La séance est reprise. Monsieur le 1er Ministre Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, après l'étape du Tour de France, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement, je vous rappelle que la science est retransmise en Direct sur France 3 Public Sénat sur le site internet du Sénat comme d'habitude, je sais que chacun aura à coeur à respecter les valeurs essentielles au Sénat, le respect des uns et des autres et une valeur plus en Lhermet mais le respect du temps, la parole est immédiatement à Monsieur Vincent Capo Canellas dans le groupe de l'Union centriste. le président de la République s'est exprimé ici même au Sénat, lors de la conférence des territoires sur l'avenir des collectivités locales, il a confirmé la suppression de la taxe d'habitation pour 80 pourcent des des foyers et annoncé 13 milliards de réduction des dépenses, le président de la République alterner les annonces pour certaines positives pour beaucoup inquiétante pour nos collectivités afin de lever toute ambiguïté, nous confirmez-vous que la suppression de la taxe d'habitation pour 80 pourcent sera compensée par voie de dégrèvement, ce qui permettrait de compenser la perte réelle de recettes en calculant ce que la taxe d'habitation aurait effectivement rapporté aux collectivités, ce système de dégrèvement est important car il garantirait une forme de neutralité financière et surtout vous engagez-vous en ce cas, à ce que ce système de dégrèvement soit maintenu par la suite. S'agissant des 13 milliards de baisses des dépenses infligées aux collectivités locales, ce qui est considérable, le président a déclaré qu'il n'y aurait pas de baisse des dotations en 2018, mais que les collectivités seraient appelés à baisser leurs dépenses selon le mécanisme dit intelligent non défini en fonction de la baisse constatée, les dotations serait donc réviser, dès lors, comment envisagez-vous de fixer un objectif de baisse des dépenses par collectivité selon lequel un guide indicateurs et quelles modalités, enfin l'effort attendu du monde territoriale suppose des choix forts s'agissant de la, de l'architecture d'ensemble de nos collectivités derrière la formule de niveaux de collectivités en-dessous de la région, quelle est votre vision stratégique en évitant le Big bang institutionnel allez vous verrez une disparition des départements en zone urbaine ou, au contraire, souhaitez-vous que le couple communes, intercommunalité devienne le pivot quasi fusionnel de cette réforme pas ces questions seront au centre des futures discussions mais le Sénat chambre des collectivités écoutera avec attention vos réponses. Merci, la parole est à monsieur Gérald armada de l'action et des comptes publics pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur

c'est à peu près, enfin un peu moins de 9 milliards le vide vers 2008 milliards CAD, d'après nos calculs, cette tranche de 80 pourcent sachant sachant que, vous le savez, il y a déjà 12 millions de foyers un peu plus de 12 millions de foyers qui sont déjà exonérés qui ne payent pas cette taxe d'habitation publication donc oui ce sera un dégrèvement, deuxièmement vous poser la question pour l'avenir, l'avenir, le président de la République a tracé devant vous et le 1er ministre le matin même de cette grande journée, monsieur le président du Sénat de la conférence nationale des territoires, posant la question de manière générale, de la fiscalité locale en conservant l'autonomie fiscale des collectivités et entend rendant des impôts plus justes, juste parce que si je prends effectivement les, les taxes, l'habitation qui sont dans la commune du Bourget par hasard, je vois que pour 2 adresses qui sont très sensiblement différente, mais pour le même revenu même couple avec un enfant avec une valeur locative identique et une surface absolument identiques même appartements, la personne qui vit dans le quartier, politique de la ville payent aussi cher que la personne qui n'habitent pas dans le quartier, politique de la ville de votre commune, tout le monde constate en effet. Qu'il y a ici une injustice et notamment une injustice sociale et en plus, comme le dit monsieur le 1er ministre vous n'y êtes pour rien puisqu'il s'agit d'un impôt injuste socialement pour les collectivités locales, mais aussi pour la compréhension des Français pour leur fiscalité avec monsieur le ministre d'État, nous parlions d'ailleurs ce midi encore de ce que nous allons proposer comme discussion aux élus et bien sûr aux parlementaires, et particulièrement aux sénateurs, parmi les pistes il peut il y a, effectivement, il y avoir un certain nombre d'initiatives notamment. Quand on sait que 150 pour 100 100 50 des plus grandes collectivités représentent 60 pourcent de de la dépense publique, peut-être faut-il faire davantage au jardin à l'anglaise, qu'à la française mais dans une viendront avec Monsieur le Ministre d'État devant vous, je vous le promets. La parole est à monsieur Dominique de neige pour le groupe, les républicains et pour 2 minutes. Seul. Monsieur le 1er Ministre Mesdames et messieurs les minutes, chers collègues, sans doute parce que j'appartiens à l'ancien monde, j'ai quelques difficultés à comprendre comment on peut en même temps et j'insiste sur le en même temps annulé 850 millions d'euros crédits du budget de la Défense, déclaré que cette décision ne perd en rien les capacités opérationnelles de la France, et en même temps, a encore déclaré que la loi de finances sera exécuté à l'Euro près : auriez-vous l'obligeance Monsieur le 1er ministre de bien vouloir m'indiquer de façon concrète comment on résout c'était équations et, plus particulièrement, quels sont les programmes d'équipement des forces qui sont annulés, quel engagement dans ce contexte, prenez-vous pour assurer l'intégralité du financement des OPEX, et enfin, envisagez-vous de débloquer les 2 milliards Pour vous répondre la parole. Quand Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des armées. armées. Le président, mesdames les sénatrices Monsieur mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur de linge, bon, vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le Sénateur la situation difficile dans laquelle nous avons trouvé les finances de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir également que nous prenons des engagements auprès des pays que nous essayons de respecter 850 millions d'euros ont effectivement été proposés à la suppression du budget des armées qui seront oui, un moment difficile pour nos armées, mais la ministre des armées, prendra les décisions utiles pour en limiter la portée et les moyens opérationnels, ainsi que sur la base industrielle de défense, elle sera avisée à surveiller de près l'exécution du budget 2017 afin que nos armées, l'exécution de cette le exécution budgétaire pardon soit à la hauteur de l'engagement, je voudrais vous peur parler d'avenir proche, monsieur le sénateur, l'avenir proche, c'est l'annonce qu'a faite le président de la République et qu'il a réitéré à Istres aujourd'hui où il se trouve, d'une augmentation inédite du budget des armées pour l'année 2018 augmentation d'1 qui portera ce budget à 34,2 milliards, ce qui en fait un budget le un des seuls Budgets qui augmentera, a dit le président de la République à Istres dans l'année 2018 et nous comptons sur vous sénateur pour nous aider à porter ce budget à cette hauteur et enfin l'engagement budgétaire pour 2025 à appelé ce sont des promesses qui seront respectés, 2 pourcent du du PIB 60 50 milliards d'euros, le budget des armées sera respectée et nous y veillerons avec vous, mesdames et messieurs les sénateurs. Madame la Ministre, heureusement que nos militaires sont plus précis dans le Tir des missiles que vous dans votre réponse à ma question. Pourtant, tout avait bien commencé, une descente ou une remontée des Champs-Élysées en commande, car une visite à Percy des victimes civiles et militaires, une visite sur les OPEX, et voici qu'à la veille du 14 juillet de façon symbolique, un arbitrage plus inspiré par un inspecteur des finances sans doute que par Jupiter rend cette excusez-moi, mais tout ceci nous éloigne des images que nous avait données le président de la République garant et gardien de la souveraineté nationale, il porte la responsabilité de cette atteinte à la souveraineté. La parole est à notre collègue Alain Bertrand pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen, vous avez la parole un collègue. Monsieur le président du Sénat, Monsieur le 1er Ministre Mesdames et messieurs les Ministres, Monsieur le ministre à la cohésion territoriale cela dit ici même au Sénat, le président de la République, Emmanuel Macron en fait plusieurs annonces lors de la conférence des territoires, j'ai trouvé modestement dans ces propos une partie du très modeste rapport que j'ai commis sur les pères ruralité. Il a dit je cite le président de la République que la réalité ne faisait pas l'aumône, qui souhaitaient un moratoire sur les fermetures d'écoles, zones rurales. Ou encore qu'il faut donner plus à ceux qui en moyenne. Là où les élus ne souhaitent, il veut une plus grande liberté d'organisation oui mais c'était Portal pour la ruralité de développement de mutualisation, il veut privilégier chaque fois que les élus, a décidé l'efficacité, la recherche de synergies pour optimiser le fonctionnement et favoriser le service aux territoires, aux citoyens, tout en maintenant l'investissement avait-il annoncé et c'est très important la création du linge à elle seule de cohésion des territoires. Nous avons donc cap pour les zones difficiles, une stratégie claire toutefois je souhaite je souhaiterais j'aimerais je participerai pour obtenir d'autres avancées sur 3 points : Monsieur le Ministre, premièrement, je souhaite que le gouvernement met en avant le rôle d'un hinterland que jouent les territoires ruraux parce qu'il faut faire reconnaître que la ruralité et créatrice d'une partie importante de la richesse et de l'âme pourra qui a fait de sommes comptabilisées dans les métropoles et les grandes agglomérations. Deuxièmement, Cannes est-il précisément si on peut dire ici lundi métropolisation entendez-vous mettre fin à l'entassement de tout dans les métropoles les capitales de région et les grades des agglomérations il y a toute une tarée grandes institutions d'entreprises d'administrations qui peuvent être décentralisées vers des territoires ruraux perd une roue en difficulté pourquoi par exemple ne pas placer l'agence de cohésion des territoires à Lozère ou dans la Creuse ou dans les Vosges ou dans le Jura. Pensez à votre question pour terminer. Vrai, pouvez-vous également me confirmer que sur le plan d'investissement de 5 à 2 milliards d'euros, une partie sera affectée aux zones les plus fragiles, parmi lesquels les zones rurales, monsieur le Président. Pour répondre à la parole est à Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires pour 2 minutes 30. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, monsieur le sénateur Bertrand. Vous êtes le chantre ici de l'hyper-ruralité, c'était donc une hyper question d'abord, je voulais vous dire : j'étais particulièrement heureux que la 1ère conférence nationale des territoires se passe au Sénat. Dans cette maison qui, au terme de l'article 24 de la Constitution représente les collectivités territoriales, ceci étant, rappelez vous avez raison de dire que, depuis de nombreuses années, une partie, une partie de la ruralité a profondément souffert chez lui une partie parce que je ne suis pas de ceux qui opposent systématiquement les territoires urbains et les territoires ruraux, il y a des il y a des territoires fragiles. Dans les villes, dans les quartiers périphériques et aussi dans nos territoires ruraux, il y a donc. Il y a donc, par rapport à cela, une vraie, une vraie politique à mener avec quelques axes fondamentaux à mettre en place, je pense au numérique au nous avons, nous sommes en train de lancer une action forte qui ne sera pas forcément facile parce que nous connaissons le poids des opérateurs et nous l'avons encore lui ce matin, dans certaines déclarations, mais il y a une vraie volonté du gouvernement de la République d'aller vite et fort sur le haut débit, le très haut débit dans nos territoires, il y a aussi, il faut le dire, l'accessibilité à nos territoires, il y a bien sûr la question des services publics, les maisons de santé, les maisons de service public et puis notre agriculture et en ce moment un débat important et lancée avec les états généraux de l'alimentation, c'est donc toute une politique qui doit se tourner vers ces territoires mais une politique qui aura pour pour but fondamental aussi de faire travailler ensemble les collectivités locales et l'État avec cette vision qui ne doit pas simplement, et ça c'est une question de fond : être une politique axée sur les problèmes démographiques, il y a des territoires qui ont peu de population, ils ont des problèmes spécifiques et nous devons en tenir compte, voilà ce que je veux dire un dernier mot sur ce que vous avez dit sur les délocalisations, ce qu'avait lancé avec courage une 1er ministre qui était Madame Cresson et souvenez-vous des réactions qui avait eu lieu, c'était une politique courageuse, ambitieuse, qui a été abandonné, parce que ce qui devait quitter la région parisienne pour s'installer en province, réagissez, de manière très corporatiste, voilà ce que je voulais vous dire sachez en tout cas que je serai à vos côtés pour mener cette politique. Merci monsieur le président. Oui, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le 1er ministre. Lundi dernier, comme nous le savons, lors de la conférence nationale des territoires, le président de la République. à porté sur les fonts baptismaux ce pacte Girondins audacieux qu'il veut construire entre l'État et les collectivités territoriales. Pour les esprits chagrins qui voudrait faire croire que les territoires constituait une sorte d'impensé présidentielle, c'est une déception. Mais pour les élus, profondément attachés à la défense des territoires, c'est une grande satisfaction. Le président de la République nous a présenté une autre qui témoigne de sa conscience aiguë des défis territoriaux auxquels notre pays doit faire face, l'écart entre France 2, métropole et France périphérique, l'importance du levier territoriale pour réussir les transitions numériques écologique, le besoin de simplification, sinon de simplicité, la nécessité de combattre les inégalités de richesse, c'est-à-dire les égoïsmes et l'indispensable refonte de la fiscalité locale, le président a su éviter le piège du grand soir territoriale et des annonces tonitruantes sans lendemain. Il a été concret sur les transports du quotidien, les déserts médicaux l'offre nouvelle dans le logement, le haut débit pour tous, oui, ces engagements ont été clairs et sans calendrier précis. Au nom des sénateurs qui se reconnaissent dans la majorité présidentielle, je veux saluer cette feuille de route ambitieuse et cette méthode pragmatique pour construire une France des territoires qui reste proche et qui voit loin, monsieur le 1er ministre. Pouvez-vous nous préciser comment le gouvernement entend mettre en oeuvre le pacte le nouveau pacte de confiance et de responsabilité que le président de la République veut sceller entre l'État et les collectivités territoriales. Merci pour vous répondre la parole. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, Monsieur le Sénateur, Berson, je salue votre enthousiasme. et je vous en remercie et je vais vous dire que nous y sommes tous ici très sensible. Comme vous le constaterez, nous voulons établir un pacte de confiance, il ne vous a pas échappé que c'est un changement. Et que, aujourd'hui, en nous adressant aux collectivités locales à tous les élus. De la nation nous voulons effectivement travailler autrement. Ne pas imposer discuter écoutez la conférence nationale des territoires L à cet objectif fondamental de ce maître de se mettre autour de la table de faire le bilan d'un certain nombre d'actions parce que nous avons tous des responsabilités dans ce qui s'est passé depuis des années quant à l'aménagement du territoire, quant à la vie de nos collectivités, c'est une responsabilité collective et nous entendons au niveau du gouvernement utiliser la Commission, cette conférence des territoires pour dégager un certain nombre d'orientation oui je vous entends quand vous dites 13 milliards mais il y a une différence, c'est que pendant plusieurs années, ça été des baisses de dotations imposée que sur les réformes territoriales pour certaines, on n'a jamais consulté les collectivités territoriales et nous entendons qu'il soit procédé différemment par la concertation par les côtes pour essayer de trouver ensemble les moyens de faire avancer nos collectivités sur tout le territoire avec plus équilibrée avec plus de justice, il y a des efforts à réaliser, il y a encore des possibilités sur les feux sur les charges de fonctionnement, c'est la réalité, il y a des 2, il y a des collectivités et je le sais, qui aujourd'hui ont des difficultés considérables, il y en a d'autres qui ont encore des moyens de faire des efforts, nous allons en discuter ensemble 12 allant travailler ensemble sur la simplification, nous allons travailler ensemble dans la concertation, sans faire de Big bang imposé pour essayer de faire mieux, de faire plus. Et monsieur Assouline vous pouvez citer des chiffres, mais je vous ai entendu accepté bien d'autres, il faut conclure dans les collectivités territoriales ne donnez pas de leçons aujourd'hui. La La parole est maintenant. à Madame, Brigitte Gonthier-Maurin pour le groupe communiste républicain et citoyen et pour 2 minutes 30. Merci Monsieur le Président, Madame la ministre de l'enseignement supérieur 87000 bacheliers sans affectation et 331 millions d'euros de crédit que vous venez d'annuler, voilà le résultat des politiques menées depuis la LRU que vous ne remettez pas en cause Dumont Current est criant de moyens pour répondre à la demande de poursuite d'études, de tous les étudiants et à l'enjeu de démocratisation de l'enseignement supérieur, au prétexte de mettre fin à la pratique honteuse du tirage au sort, vous annoncez votre intention d'instaurer des pré-requis à l'entrée à l'université, cette introduction d'un mode de sélection à l'université constitue une remise en cause du droit d'accès pour toutes et tous à la poursuite d'études comme inscrit dans le code de l'éducation, de plus, elle est en contradiction avec les principes de l'Astra naissent la stratégie nationale de l'enseignement supérieur, adopté en 2015 par le gouvernement en faveur d'une société à prenante, à prenante, au contraire, Madame la Ministre, il faut bannir pré-requis et sélection face à la gravité de la situation, je vous demande avec mon groupe de mettre en place un plan du jeu d'urgence qui ne considère plus l'université, l'enseignement supérieur, comme un coup mais bien comme un investissement indispensable pour l'avenir de nos jeunes et le développement du pays. Monsieur le président, Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Gonthier-Maurin, vous avez raison, le fait qu'autant d'étudiants autant de candidats souhaitent aujourd'hui sans affectation l'enfer saignement supérieur est un véritable gâchis, un gâchis qui a été le fait à la fois du tirage au sort de la non prise en compte de l'augmentation démographique des étudiants et de la non prise en compte du fait que cette année 100000 étudiants supplémentaires utilisent le système Admission post-bac pour se réorienter. Le véritable gâchis humain, c'est celui de ces étudiants qui échouent à l'université actuellement plus de 60 pourcent des des étudiants qui s'inscrivent dans un cycle de licence générale n'obtiennent pas de diplôme au bout de 4 ans, le véritable gâchis social, c'est que nous soyons en capacité de faire échouer autant d'étudiants alors que nous consacrons nos moyens à l'enseignement supérieur et enfin le gâchis est aussi un gâchis financier puisque lorsqu'il s'agit d'investir entre 8 et 10000 euros par étudiant dans l'enseignement supérieur lorsque ces pour les faire réussir et leur permettent de trouver un emploi, évidemment que la nation salue cet investissement mais lorsque c'est pour les faire échouer et leur donner un sentiment d'inutilité, alors la nation ne remplit pas ses devoirs, c'est pourquoi j'ai proposé et le 1er ministre a confirmé la création d'un contrat de réussite avec les étudiants, qui à l'aide d'une meilleure orientation de ces étudiants en étant en capacité de leur dire la vérité sur leur capacité à réussir en fonction des filières et en les accompagnant vers cette réussite en proposant des cours de remédiation devrait nous aider à limiter ce gâchis humain, social et financier, je vous remercie. Madame Gonthier-Maurin Madame même. Madame la ministre, la situation est grave puisque 15 univers. Cité ont été jugé dispendieuse par la Cour des comptes parce qu'elles avaient simplement décidé distribuer les moyens nécessaires à leur mission à leur mission et ce que je voudrais vous dire, c'est que nous n'avons de cesse d'avancer des propositions pour remédier à l'état de difficultés dans lequel nous nous trouvons et de ne plus considérer l'enseignement supérieur comme un coût mais comme un investissement et extraire le ces dépenses du calcul des

oui, il faudra mobiliser des moyens aussi pour changer le système d'orientation pour qu'il ne soit plus un système qui va trier mais qui les aide à réussir et il faudra évidemment mobilisés pour des passerelles

Merci, la parole. Monsieur questeur Dominique Bailly pour le groupe socialiste et républicain, vous avez la parole. Ma question s'adresse à monsieur le 1er ministre ministre actuel 1er ministre la suppression de la taxe habitation pour 80 pourcent des des ménages est annoncée pour 2018, je serais tenté face à cette proposition de vous dire chiche d'impôt est injuste, de l'avis général, injuste socialement injuste, Thierry Torii allemand pour reprendre les propos du président de la République qu'il a tenus ici au Sénat, lors de la conférence des territoires lundi. Et je pourrais même vous dire, Monsieur le 1er ministre doublement chiche, nous pourrions envisager de supprimer la taxe d'habitation pour 100 pourcent des cet impôt étant tellement injuste et d'ailleurs nous pourrions reprendre la proposition de Lionel Jospin qui, en 2000 l'avait proposé, malheureusement, il n'a pas pu aller au bout de sa volonté politique et s'est arrêté à la suppression de la part régionale de cette taxe d'habitation, mais si nous supprimons 80 ou 100 pourcent si si vous prenez ma proposition date exaltation la question essentielle : la question politique, c'est l'autonomie financière des collectivités locales, cette taxe d'habitation est aujourd'hui le pilier, donc si vous la supprimer si vous fragiliser cette autonomie financière, vous mettez en difficulté, le principe de libre administration des collectivités locales, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous le confirme, les élus locaux qui sont inquiets, ils sont très inquiets et c'est normal, j'ai entendu que vous allez procéder par dégrèvements d'accord mais je pense qu'il faut aller plus loin, vous l'avez d'ailleurs évoqué Monsieur le Ministre dans votre réponse, il faut une véritable réforme de la fiscalité locale pour durablement rassuré les écuries, les élus locaux, il faut une véritable révolution fiscale, tout le monde en parle tous les gouvernements en ont parlé, aurez-vous la volonté politique d'aboutir, il est impossible de garantir aujourd'hui est de pérenniser des dépenses dynamiques, donc voilà Monsieur le 1er ministre est-ce que vous allez rassurer durablement les élus locaux et puis votre sentiment sur ma proposition, pour 100 pourcent des

Nous aurions peut-être aimé pour la bonne un TJ intelligibilité de débat que vous nous proposez en même temps, les économies qui allait avec cette suppression totale de la taxe d'évita, c'est ce que nous ferons-nous et j'en suis certain puisque nous allons progressivement trouver ces 3 milliards, puis 3 milliards pétrolière et, pourquoi pas, vous l'avez dit, le président de la vie que l'a dit le 1er ministre l'a dit réfléchir au renouveau de la fiscalité locale en imaginant effectivement une révolution fiscale pour la taxe habitation comme la taxe foncière afin de trouver quelque chose de plus équitable pour les collectivités de plus juste pour les citoyens, mais pour l'instant, on n'est pas proposé ces économies puisque nous sommes à peu près à moins de 9 milliards pour les 80 pourcent de de ménages concernés et plus de 12 pour les les 20 pourcent qui qui restent, ça fait quand même 20 milliards d'euros à trouver, vous avez raison de dire qu'il est injuste, parce que si je prends la commune que vous connaissez bien. Celle d'Chine pour la même maison du même nombre de m2 avec un couple sans enfant à 45000 euros de revenus annuels pour le même taux de la de la commune 1000 300 9 euros pour la maison, construite en 1920 et 938 euros pour le même ménage pour le même foyer problème revenus pour la commune, conçue pour Vous dire, Monsieur le Sénateur, que nous sommes tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur le renouveau cette fiscalité, oui, nous irons jusqu'au bout, cependant je me permets de vous corriger, s'il y a autonomie financière prévue par la Constitution et le dégrèvement comme l'exonération mais le dégrèvement que nous proposons, fait partie de la confond conforte cette autonomie financière, il n'y a pas, pour l'instant, autonomie fiscale puisque toutes les collectivités n'ont pas pouvoir de tout ce qui est le cas, notamment, des régions et que la constitution prévoit pas l'autonomie fiscale en tant que telle, il faut donc que nous travaillons sur cette question d'autonomie financière d'autonomie fiscale, sachant que nous avons déjà soigné ici, même si ce n'est pas le projet du gouvernement, il peut y avoir une grande décentralisation, il peut y avoir un état fédéral qu'en Allemagne sans d'autonomie fiscale des collectivités.

ma question s'adressant à la mainmise anciennement supérieur de la recherche et d'innovation et vous également poser Madame Amir pas mon collègue Jean-Léonce Dupont, elle rejoint un peu la question qui a été posée par Madame Gonthier-Maurin mais on peut reprendre les mêmes mélodies dans des tonalités différentes ma question porte donc sur les dysfonctionnements du portail d'admission post-bac dit APB vous avez justement justifie encore tout à l'heure de gâchis ce gâchis est d'abord humain pour les jeunes et leurs familles sans doute ce soir, nous, celles qui sont le moins code qui ont le moins le code pour utiliser au mieux l'algorithme et dans la poursuite d'études leur enfant est aussi un investissement très lourd. Si vous venez d'engager une large concertation pour éviter de telles en s'à la rentrée 2018 et préconiser des prérequis naturellement indispensable il demeure à ce jour, partout en France, quel 4 87000 néo-bachelier pour certains reçu avec mention sans affectation pour septembre prochain clim si j'ai bien compris d'un tirage au sort, voulue par vos prédécesseurs et dans l'absurdité pour c'est Pauline échappe à personne, or la plupart des universités ferment leurs portes dans quelques jours aux alentours du 20 août notre question madame la ministre est simple : comment comptez-vous dans ce calendrier précontraint veiller à ce que ces milliers de jeunes débouté provisoire du droit aux études supérieures, ne perdent pas une année que leurs familles désemparées, ne se plaint pas vers des formations nerveuse et parfois sans réelle garantie garantissez-vous que les solutions trouvées ne seront pas substantiellement éloignées de leur projet d'études initiales, comment comptez-vous faire aussi pour ces jeunes, selon leur localisation parviennent dans des délais courts à se loger dans les villes universitaires qui les accueillera quelles instructions donnerez-vous au cross en ce sens, ce sont des questions certes terre-à-terre mais qui, hier, qui appelle des réponses immédiates et concrètes et les familles vous en remercie.

Effectivement, vous avez raison, il y a encore 87000 candidats qui sont inscrits sur la plateforme Admission post-bac, mais ces candidats ne sont pas tous des néo-bachelier pour une grande partie d'entre eux, ce sont des candidats qui sont en réorientation et qui ont donc leur place dans leur dans leur filière d'origine s'il souhaite y retourner, nous y trouvons ensuite un grand nombre de candidats qui pour le moment, n'ont pas accepté de façon définitive leur choix et qui sont en attente d'un meilleur choix possible et il reste aujourd'hui environ 10000 néo-bachelier qui sont notre priorité, ils étaient 17000 il y a 15 jours, ils étaient 36000 il y a un mois, et nous travaillons jour après jour à réduire ce nombre nous entrons maintenant dans la phase, une nouvelle phase d'admission post-bac, où l'ensemble des près de 200000 places libérées dans l'enseignement supérieur pour la rentrée prochaine seront offertes à l'ensemble des candidats, de manière à ce qu'ils puissent exprimer leur choix en fonction des places disponibles, ceci dit, bien entendu, ce système reste d'une injustice absolue puisque vous l'avez souligné la capacité à utiliser ce système de manière correcte, la capacité à obtenir une information de façon correcte, n'est pas la même pour l'ensemble des candidats, c'est pourquoi nous avons souhaité supprimer le tirage au sort pour la rentrée 2018 et c'est pourquoi, au travers d'une orientation renforcée dès le lycée et au travers d'un accompagnement particulier en précisant les pré-requis et en disant comment on aide les futurs étudiants à les acquérir, nous sortirons de cette situation, je signale que la plateforme APB vient de réouvrir et quel sera ouvert jusqu'au 25 septembre à compter du 20 août l'ensemble des rectorats et des universités traiteront les cas un par un pour les néo-bachelier merci. Merci, la parole est maintenant notre collègue Cédric Perrin pour le groupe, les républicains. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le 1er ministre monsieur le 1er ministre le gouvernement ainsi qu'il a été rapporté envisage de réduire de 850 millions d'euros, le budget de la Défense en 2017, chacun est ici au fait des événements aussi inhabituel que regrettable qui se sont va dérouler et qui ont abouti hier fait rarissime, voire unique à la démission du chef d'État-Major des armées, Pierre de Villiers je veux ici rendre hommage au général De Villiers grand soldat, grand serviteur de l'État, donc j'ai pu, comme tous ceux qui n'ont côtoyé constater l'engagement sans réserve au service de la France et de sa défense s'il l'a souvent dit qu'il ne faut pas gâcher l'opportunité d'une crise, gageons que celle-ci grave et l'occasion de s'interroger sur certains faits : le 1er c'est fait, c'est que nul de sérieux ne conteste qu'il n'ait pas d'autorité plus habilité que le chef d'État-Major des armées, apporter un diagnostic sur l'état de nos forces, ce diagnostic, en dépit de son départ restent valides oui, 3 fois oui, les moyens de nos armées, vous le savez, ont été consciencieusement réduit au cours des années récentes, de quantité de nos matériels compromet non seulement l'émission mais dans certains cas jusqu'à la sécurité de nos soldats, le second c'est fait, c'est l'extrême légèreté avec laquelle le travail parlementaire a été considéré, car jusqu'à preuve du contraire, les propos tenus à huis clos par le cinéma en commission parlementaire, je mets de côté certaines expressions n'était nullement déplacée à moins qu'il n'existe désormais Monsieur le 1er ministre ce qu'il faudrait bien appeler une jurisprudence Soubelet. Dans ce contexte, Monsieur le 1er mise, j'ai 2 questions : premièrement, le gouvernement est-il sincère quand il prétend que nos forces disposeront des moyens de leur mission, alors que vous leur couper les crédits et deuxièmement, pouvez-vous prendre l'engagement que le travail du Parlement sera pleinement respecté et que les personnes, a été auditionné par les commissions ne seront pas sanctionnés en raison d'un diagnostic potentiellement dérangeants pour l'exécutif, merci. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, il y a un chef d'État-Major des armées. Il a un chef des armées. Ce sont 2 fonctions différentes, 2 légitimités différentes 2 expériences différentes. Et s'il y a un désaccord entre le chef d'État-Major des armées et chef des armées. Monsieur le sénateur dans notre République, sous la Vème République, c'est le pouvoir politique qui prévaut. Le chef d'État-Major des armées, a exprimé. Un désaccord. Avec des décisions prises par le président de la République, il en a tiré les conséquences : vous avez raison, raison, Monsieur le Sénateur de lui adresser un salut républicain au moment où il quitte ses fonctions, je m'associe à ce salut républicain je je me permets de saluer de la même façon, celui qui prend le poste le général Lecointre, que vous connaissez sûrement puisque vous vous êtes passionné par ces questions de défense. Mais encore une fois soyons clairs. Le chef des armées, dans notre pays, dans notre régime a le dernier mot en matière de choix militaires et il ne peut pas en aller autrement et il ne peut pas en aller autrement sur la question de la disponibilité budgétaire et de l'effort budgétaire consenti pour nos forces de défense. Je ne pense pas, monsieur le sénateur. Non, je vais prendre autrement, le président de la République s'est engagé à porter l'effort de défense en 2025 à 2 pourcent du du PIB, c'est un engagement qui a été pris ferme. S'il faut monter à 2 pourcent du du PIB, c'est parce que pendant de longues années, monsieur le sénateur, notre effort de défense n'a probablement pas été au niveau du danger du monde et de son instabilité et je ne crois pas, Monsieur le Sénateur, même si vous nous en faites le grief aujourd'hui, je ne crois pas que cette situation et cet état de fait date d'il y a 2 mois, je pense que malheureusement le diagnostic, je ça n'est pas la première fois que nous opérons des régulations budgétaires, c'est pas la première fois, et quand je dis nous, je prends la responsabilité, pour tous les gouvernements qui sont précédées. Donc ça n'est pas 9, je voudrais vous citer quelques chiffres, Monsieur le Sénateur, car après tout autant être précis. Le budget 2016 de la défense a été voté en loi de finances initiale à 31,8 milliards d'euros. Le budget 2017, a été voté en loi de finances initiale à 32,4 milliards d'euros, il sera d'ailleurs exécutés à peu près à 30 2,4 milliards d'euros, et vous avez raison, Monsieur le Sénateur et et j'apprécie vivement que vous mentionniez le fait que 700 les OPEX car qu'avons-nous fait et je dis encore une fois, je ne suis pas là pour dire qu'il y aurait des coupables d'responsables qu'avons-nous fait collectivement depuis plusieurs années, nous avons poussé tranquillement, année après année un report à nouveau de crédit qui se montent à 750 millions d'euros cette année que nous allons d'ailleurs descendre à 700 millions d'euros, et vous savez très bien que ça n'est pas satisfaisant comme vous savez très bien que, depuis de nombreuses années pour des raisons budgétaires qui peuvent s'expliquer, nous n'intégrons pas complètement dans le budget de la défense, le coût des OPEX, or nous savons qu'elle coûte cher mais nous trouvons depuis longtemps, monsieur le sénateur, nous ne regardons pas en face ce que coûte notre effort de défense, le président de la République l'a dit le 13 juillet il l'a redit ce matin, le budget 2018 de la Défense se montera en ressources budgétaires à 34,2 milliards d'euros pour l'année 2018 7 1,8 1000000000 d'euros de plus que la loi de finances initiale 2017, c'est un effort de plus 5,25 pourcent pour pour le budget des armées, c'est plus que la progression du PIB, c'est plus que l'inflation, ce sera le seul budget qui augmentera en volume, je me permets de dire, Monsieur le Sénateur que cet effort conséquent conséquents. Ne s'arrêtera pas en 2018. si nous voulons atteindre en 2025 les 2 pourcent du du PIB, ce qui est un effort considérable l'année après année, nous allons devoir suivre une courbe d'augmentation de la dépense et nous n'allons pas le faire pour faire plaisir à telle ou telle nous allons le faire parce que la modernisation de nos équipements, la modernisation de notre capacité de dissuasion, les engagements que prend la France à l'étranger exige que nous préparions notre outil à la satisfaction et la protection de nos intérêts, je peux comprendre toutes les polémiques, ici tout le monde aime son pays et même la politique. Mais, Monsieur le Sénateur. Regardez sur 3 mois, ce qui se passe en matière de défense alors que l'effort a été diminué depuis très longtemps, depuis très longtemps et depuis trop longtemps, et alors que nous nous sommes engagés pour le budget 2018. Au montant nous sommes engagés à quelque chose, me semble-t-il, qui n'est pas totalement au niveau des hanches, je vous remercie. La parole non madame Michelle Meunier. Pour le groupe socialiste et républicain et pour 2 minutes. lors de la campagne pour l'élection présidentielle, le candidat Emmanuel Macron ne voyait pas de justification juridique à s'opposer à l'ouverture de la PMA pour les femmes, quelle que soit leur statut conjugal ou leur orientation sexuelle, il attendait l'avis de la commission consultative nationale d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé pour s'assurer d'un débat pacifié et argumentée, cet avis est désormais connu, et l'attente est forte chez les femmes seules ou en couples ayant un projet d'enfants, il n'y a donc plus d'obstacle à ce que l'ouverture intervienne au plus tôt et mettent fin à la situation hypocrite qui pousse les femmes françaises à aller en Espagne ou en Belgique pour effectuer une assimilation artificielle avec donneur, ma question est simple Madame la ministre, dans quel délai allez-vous permettre l'ouverture de la PMA aux femmes seules ou en couples, ainsi que la prise en charge par la Sécurité sociale, merci.

l'ouverture de la PMA à toutes les femmes étaient un engagement de campagne du président de la République, il avait conditionné la tenue cet engagement à l'a rendu un avis favorable du CCNE du comité consultatif national d'éthique, cet avis a été rendu après une auto-saisine qui date de l'année 2013, cet avis est favorable à l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes qu'elles soient en couple ou qu'elles soient célibataire et la vie est négatif en ce qui concerne la légalisation de la GPA avis de du CCNE il y a tout à fait en conformité avec les engagements de campagne du président de la République et avec notre position, c'est-à-dire que nous ouvrirons effectivement la PMA, mais nous voulons avoir un débat serein et apaisé sur ce sujet avec comme boussole permanente, l'intérêt de l'enfant et en préservant les couples et les familles des insultes et des actes homophobes qui peuvent survenir lors des débats de ce type, c'est pourquoi, avec mes collègues, la garde des Sceaux et la ministre de la Santé et des solidarités, nous ouvrons en appui du CCNE les états généraux de la bioéthique et nous permettront d'ouvrir la PMA à l'ensemble des femmes à partir de la révision de la loi bioéthique de 2018 et je me permets d'ajouter que, conformément aux décisions qui ont été rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, nous favoriserons l'inscription des enfants déjà nés de GPA à l'étranger à l'état civil, en France, je vous remercie. Merci.

les débats concernant la PMA, donc plus nous serons rapide sur cette décision et mieux ce sera pour les femmes et les couples en attente, merci. Merci, la parole est maintenant notre collègue François Bonhomme pour le groupe des Républicains pour 2 minutes. Monsieur le président, Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur ministre d'État, ministre intérieur. Lundi dernier, le président de la République est venu ici au Sénat, se faire porteur de mauvaises nouvelles pour les collectivités locales, une baisse de 13 milliards d'euros de leurs dépenses, une suppression de la taxe d'habitation et une baisse du nombre d'élus locaux. D'abord une nouvelle ponction de l'État sur les Budgets locaux, des collectivités locales, viendraient s'ajouter aux déjà aux efforts déjà réalisés par celle-ci, une baisse de 11 milliards de 2014 à 2017 cette annonce vient sans contrepartie et sans réforme de fond risque assurément d'affaiblir une nouvelle fois leur capacité d'action en supprimant la taxe d'habitation, c'est aussi la volonté de substituer le contribuable local au contribuable national. C'est par la même occasion, une façon de réaliser un vieux rêve de Bercy, celui de priver les collectivités locales d'un principe qui fondent leur action, je veux parler de l'autonomie fiscale, enfin, surprise du chef, le président de la République, indique vouloir moins d'élus locaux, voilà bien annoncent tout aussi illusoire que funeste sur les 500000 élus locaux 90 pourcent ne ne sont pas rémunérés, ce sont des bénévoles au service de leurs habitants mieux ou pire ils constitue souvent le seul interlocuteur n'a été autant ruraux et forment un maillage civique qui est une chance pour notre pays, alors Monsieur le ministre, à l'heure où nous n'avons ou nous avons besoin au contraire de plus de civisme, comment comptez-vous dès lors articuler cette mesure restrictive, avec l'annonce de services de proximité et de Liam plus fort et plus étroit avec nos concitoyens. Monsieur le prion, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur François Bonhomme tout à l'heure, mon collègue Gérald Darmanin avait amené son petit cahier, moi j'ai amené mon petit compteur, c'est le niveau de la dette publique. Et vous voyez que chaque seconde, il s'accroît de 2655 euros et que donc, évidemment, nous avons à réduire la dépense publique. Alors sur ce point. Sur ce point. Mesdames et messieurs les sénateurs. S'il vous plaît à respecter le temps envie. Croyant est d'accord pour réduire la dépense publique mais chacun veut que ce soit chez l'autre, nous avons proposé une méthode que nous puissions discuter ensemble et c'est l'objet de la conférence nationale des territoires pour regarder comment ensemble nous pouvons faire baisser la dépense publique, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des collectivités publiques et ce sera une première pour l'État parce que, comme l'a justement remarqué la Cour des comptes, et c'est l'ancien élu local qui parle si effectivement les collectivités publiques ont réduit leurs dépenses, l'État jusqu'à présent ne l'avait pas fait sur la réduction sur la réduction du nombre d'élus, notre collègue Pélissard a proposé par exemple les communes nouvelles pour faire quoi pour à la fois accentuer l'action publique et en même temps pour réduire le nombre d'élus locaux moi-même lorsque j'ai fait savoir conclure j'ai supprimé 26 conseillers généraux sur 55 est-ce que ça fonctionne, moins, moins bien, non, ça fonctionne mieux.

en effet, c'est pas les les élus locaux et particulièrement les yeux communaux qui coûte cher, vous savez très bien qu'il faut un travail au quotidien qui constitue un engagement civique au quotidien et heureusement qu'ils sont là pour ça peut s'occuper de leurs habitants mais tout cela m'inspire une

parce que peut-être n'aurait-il pas fait une telle proposition, au contraire, mais il est vrai, il annonçait aussi vouloir créer un droit à l'erreur, ceci pouvant expliquer cela. Merci, la parole est maintenant. à notre collègue Jean-Yves Leconte pour le groupe socialiste et républicain. Merci monsieur le président, Monsieur le 1er, mesdames et messieurs les Miss, mes chers collègues, ce sont 55000 élèves de plus ce qu'il y a 6 ans, qui fréquentent aujourd'hui les établissements scolaires français à l'étranger sur cette période, il a fallu ouvrir quelque 1800 nouvelles pourtant autant aucun enseignant titulaire français de plus n'a été détaché à l'étranger pour la prochaine rentrée scolaire : 20 pourcent des des demandes de détachement au profit de nos établissements scolaires ont reçu une réponse négative du ministère de l'Éducation nationale depuis 2 ans, les communautés scolaires sont déstabilisés par la menace de non-renouvellement de détachement pour des personnels ayant pourtant un statut de résident et non d'expatriés aujourd'hui plusieurs établissements scolaires arrête des projets d'extension ou tente de faire cesser la croissance de leurs effectifs, car il n'espère plus recevoir d'enseignants titulaires, il ne s'agit pourtant pas d'un problème budgétaire puisque la croissance est totalement malheureusement financé par les frais d'écolage nous devons constater que les besoins des établissements scolaires à l'étranger ne sont pas pris en compte dans la planification des académies et du calibrage des concours qu'elles organisent pourtant nous n'avons pas d'autre solution pour obtenir avec certitude des enseignants titulaires, nous avons besoin d'enseignants titulaires en France à l'étranger aussi pire ce qui pourrait passer un concours pour le devenir et qui vivent à l'étranger doivent définitivement rompre avec leur pays de résidence, ils sont aujourd'hui puni dissuader d'engager cette démarche cela Monsieur le ministre n'est pas acceptable, monsieur le Ministre quelles assurances, pouvez-vous donner au z'résidents qui devront l'année prochaine, faire une demande de renouvellement de leur détachement, comment pouvons-nous intégrée à la programmation des besoins de votre ministère, les besoins des établissements scolaires français à l'étranger comment inciter ceux qui pourrait, à l'étranger, passer un concours pour devenir titulaire à le faire sans se couper de leur famille et de leur vie, comment dans toutes les prochaines semaines, pouvons-nous régler les cas individuels qui subsistent à la veille de la rentrée de septembre 2017, monsieur le ministre, nos établissements français à l'étranger sont essentiels à notre présence et à notre action à l'étranger, ils sont avec leur primordial de cet esprit de conquête que souhaite aujourd'hui incarner le président de la République, ils sont un outil important d'enrichissement et d'échanges et mérite notre mobilisation et nous avons besoin, Monsieur le Ministre de la mobilisation du ministère de l'Éducation nationale. On la parole, Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, le merci beaucoup pour cette question qui m'offre l'occasion de parler à votre suite et en cohérence complète avec votre question des lycées français à l'étranger l'enseignement français à l'étranger en général, vous avez tout à fait raison comme vous l'avez fait en conclusion de souligner l'excellence de cet enseignement qui fait honneur à la France, avec de très nombreux candidats pour être élève dans dans ces lycées, notamment au travers de des lycées de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et de la Mission laïque française, cela représente une présence française dans près de 140 pays aujourd'hui, vous avez eu raison de de souligner le le développement de la demande ces dernières années et peut-être un certain d'immobilisme notre part au cours des 5 dernières années, aussi, il faut maintenant arriver à un certain dynamisme de en en la matière et voir dans quelle mesure, d'ailleurs, nous pouvons nous inspirer de de ce succès pour non seulement développer l'enseignement français à l'étranger, mais même s'inspirer de ce succès pour des éventuelles évolutions futures en France par rapport à la question précise que vous posez, je voudrais répondre à la fois conjoncturellement est structurellement sur un plan conjoncturel, il est vrai qu'il y a des refus de détachement, j'ai donné des instructions pour que ces refus soient les moins nombreux possibles : d'abord, nous avons accepté tous les renouvellements de de postes tous, ensuite nous avons environ accepté 2 tiers des demandes, cela représente environ 414 demande dans le 1er degré 447 dans le dans le second degré et nous avons fait à peu près 250 refus ces refus se concentre dans les académies qui ont un déficit de personnel, ce n'est pas un problème de support, c'est un problème de personnel, c'est-à-dire les académies de Créteil, de Versailles et de Guyane, nous devons évidemment à Moliro ça dans le futur nous l'améliorons d'une manière structurelle en ayant une politique de recrutement d'enseignants qui se prépare à travailler à l'étranger, aujourd'hui, vous l'avez souligné ce qui sortent néo-titulaires ne sont pas ne

Monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, 641700 lycéens ou le Baccalauréat précieux sésame pour pouvoir entrer à l'université, ces résultats ont bien sûr suscité la joie et la fierté pour les familles, ainsi que pour les lauréats joie et fierté qui sont vite retombés pour certains bacheliers à ce jour, il existe une grande inquiétude des familles pour la raison que vous connaissez, Madame la Ministre, ou là vous en êtes expliqué tout à l'heure, il existe une plateforme informative APB, qui travaillent sur des algorithmes et qui a laissé 87000 élèves sur le étudiants sur le carreau ou futurs étudiants près de 15 pourcent ces ces procédures d'admission post-bac est un échec total, les algorithmes laisse sur la touche des élèves brillants à Besançon, j'avais pour preuve une étudiante qui a choisi, dans le cas de son 1er choix vétérinaire Dijon 2ème choix vétérinaire, Besançon et 3ème soit médecine c'est étudiante a eu une mention bien au Baccalauréat, actuellement, elle n'a rien donc le conseiller quoi, de partir à l'étranger de rentrer dans un établissement catholique qui ne travaillent pas sûr sauf mode de formation, en tout cas cette procédure d'admission est un scandale, elle est unique en Europe, je sais que vous n'êtes pas responsable et beaucoup d'autres d'ailleurs étudiant arrête en fin du 1er semestre donc on embolie ce quelque part aussi 6 place le 2ème scandale et vous n'êtes pas responsable mais il est dû à l'ancienne ministre Éducation nationale qui ne restera pas dans nos mémoires, c'est cette circulaire publiée entre les 2 tours de la présidentielle pour officialiser le recours au tirage au sort pour les filières à effectif contraint de questions : la première, quelles dispositions entendez-vous prendre dans un 1er temps pour pallier à ce type d'état d'urgence est la 2ème peut-être plus intéressante pour vous, nous nous en dire plus sur ces prêts requis qui existent en Europe à ce jour, ils existent dans tous les pays européens, pour nous, le mot sélection n'est pas tabou, les présidents lui son accord par contre les syndicats étudiants sont moins debout contre cette réforme. réforme. La ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, l'innovation, l'amygdale pour 2 minutes maximum. Monsieur le président, Mesdames et sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Grosperrin, vous l'avez rappelé 87000 candidats qui actuellement sont toujours sur le logiciel de gestion de candidatures Admission post-bac, 641700 bacheliers 851000 candidats inscrits sur cette plateforme qui ne traite donc pas, comme je le rappelais tout à l'heure, uniquement les néo-bachelier pour la rentrée 2017, nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des services des universités et des services académiques, de manière à ce que dans la procédure d'admission complémentaires le maximum de ses candidats puissent trouver une place, vous avez cité un exemple il y en a des centaines d'autres tous sont aussi injustes les uns que les autres. En quoi va consister ce contrat de réussite et et comment allons-nous travailler les pré-requis, je veux être clair, je suis pour que l'ensemble des élèves titulaires du Baccalauréat qui souhaite poursuivre des études dans l'enseignement supérieur puisse le faire, j'estime que c'est un droit et ça a été rappelé, mais par contre je pense qu'il est absolument indispensable que cette poursuite dans l'enseignement supérieur souhaite accompagner d'où la notion de pré-requis, d'où la notion d'attendu tout le fait que nous soyons en capacité d'indiquer clairement à un futur étudiant, quelle est sa probabilité de réussite dans une filière en fonction de ce qu'il a fait avant et si malgré tout, il souhaite intégrer cette filière que nous soyons en capacité de lui proposer un accompagnement pour avoir toutes les chances d'y réussir, un jour, il ne s'agit donc pas de répondre non à l'entrée dans le supérieur à un étudiant, il s'agit de lui dire oui, franchement tu as tous tes chances pourrait réussir en l'état ou oui, mais nous allons t'accompagner pour réussir, je vous remercie. Merci madame la Ministre, la dernière question et à notre collègue Aline Archimbaud, vous avez la parole pour 2 minutes 30. Monsieur le président, collègues, ma question s'adresse à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail, madame la ministre, nous avons été alertés il y a quelques jours par des associations de victimes de l'amiante sur le fait qu'une vingtaine de procédures pénales emblématique du scandale de l'amiante se diriger vers un non-lieu à la demande du parquet, la difficulté déterminer la date exacte à laquelle les salariés ont été contaminés et intoxiqué et donc la difficulté de savoir qui, dans les entreprises étaient aux responsabilités, à ce moment-là, justifierait ce non-lieu, il y aurait donc aucun responsable de la mort de milliers de personnes, aucun responsable de la maladie de milliers d'autres l'amiante est un matériau que l'on sait cancérigène certain depuis 1977 qu'il n'a été interdit en France qu'en 1997 20 ans après, des dizaines de milliers de salariés, artisans sous-traitants ont été en contact avec les fibres lors de leur vie professionnelle sont des milliers à avoir développé des cancers particulièrement agressifs qui ont des caractéristiques bien spécifiques et dont on ne et dont on peut donc dire avec certitude qu'ils sont liés à l'amiante ce matériau est extrêmement dangereux car, contrairement à d'autres cancérigène pour lesquels la dose fait le poison, une seule fibre d'amiante inhalées peut provoquer un cancer les experts le disent l'intoxication peut donc débuter dès la première Exposition et l'on connaît donc les dates de ses premières expositions pour tous les malades, madame la ministre, ce revirement de situation épouvantable met en avant un véritable problème, celui de la sécurité au travail, celui de la responsabilité des entreprises vis-à-vis de leurs salariés et de leurs anciens salariés madame la Ministre nous écologistes, nous nous interrogions, que fait-on lorsqu'on a des gens qui sont malades par milliers, du fait de leur Exposition sur leur lieu de travail qu'on connaît les causes de leur maladie, qu'on connaît l'enchaînement des causes qui ont conduit à ces maladies et qu'il n'y a pas de responsable d'un point de vue simplement moral, éthique aussi immiscé aucunement dans la procédure judiciaire, les pouvoirs publics ne peuvent-ils pas prendre une initiative pour donner un signal positif aux victimes et à leurs soutiens qui sont accablés par cette non-réponse. On vous répond : la parole est à madame la ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Allmerch un tout d'abord je voudrais excuser l'absence de ma collègue Agnès Buzyn, qui, en déplacement aujourd'hui nous menons ce ce dossier ensemble un évidemment puisque et la santé et le travail sont concernés. Tout d'abord, vous avez raison de dire que c'est un sujet majeur. L'année dernière en 2016, 20000 demandes d'indemnisation sont ont été adressées et sont examinés, c'est le flux à peu près équivalent des dernières années, il est en très légère baisse après des années d'augmentation, donc ce sont des dizaines de milliers de personnes au total qui sont concernés. C'est un sujet majeur aussi sur le plan financier pour la sécurité sociale, puisque les 2 milliards d'euros de dépenses annuelles sur ce sujet, représente plus de 17 pourcent des des dépenses de la branche accidents du travail professionnelles de la Sécurité sociale, autant dire que ce sujet nous concerne tous, tant sur le plan humain que sur le plan financier. Alors évidemment, nous ne pouvons pas commenter une décision de justice, vous le comprenez ça ne pas dire que nous pouvons pas agir. l'action concerne les entreprises comme il concerne l'État, de renforcer le rôle des branches dans différents domaines et pas ordonnance le sujet de la prévention de la pénibilité, le prévention des maladies Professional se rend dans les compétences fixées par la loi pour les négociations de branches, deuxièmement en ce qui concerne l'État, un plan interministériel d'action amiante a été mis en place, a été lancé pour 3 ans le 1er janvier 2016, bien évidemment, nous ne continuerons est d'ores et déjà mes services, en particulier la direction générale du Trésor et mobiliser pleinement sur ce sujet notamment sur 5 points et vous en avez évoqué certains l'amélioration de la connaissance scientifique et technique, on a, depuis l'interdiction encore améliorer la connaissance il y a aujourd'hui 3 plus de 3700 maladies professionnelles répertoriées concernés faciliter le repérage de l'amiante, car il y a encore de l'amiante, protéger les travailleurs et l'environnement qualifiés formés et contrôlés et accompagner l'appropriation de la réglementation pour que tous la connaissent, salariés et employeurs, vous pouvez compter sur l'engagement des services et mon engagement total sur ce sujet très important. Madame la ville, je vous remercie pour votre réponse précise, concrète, j'espère que cette engagement que vous nous promettez sera suivi d'effet au Sénat depuis 2005, des travaux sont menés sur ces questions et est réellement, on est devant une situation tellement dramatique, nous espérons qu'enfin des décisions concrètes seront prises. Monsieur le 1er ministre de l'Inde, messieurs les milices, merci les prochaines questions d'actualité ont lieu le mardi 1er routes sont sans doute les dernières de la session extraordinaire je vais suspende la séance qui sera reprise assez pour le débat sur l'orientation des finances publiques et le projet doivent règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2016, la séance est suspendue.

La séance est reprise et notre ordre du jour appelle le débat sur l'orientation des finances publiques et la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée le règlement du budget d'approbation des comptes pour l'année 2016, la 3 conférences des présidents, je vous le rappelle, a décidé de joindre la discussion générale, ce projet de loi au débat sur l'orientation des finances publiques et dans ce débat comment la parole est à monsieur

Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui. Les orientations retenues par le gouvernement et par le président de la République en matière de stratégie économique dans le cas de ce débat dans l'tentation des finances publiques. La situation économique aujourd'hui se caractérise. Par 3 points que vous avez tous. Parfaitement en tête, mais que je me permettrai de rappeler. Le 1er c'est une croissance qui revient dans la zone Euro à 1,7 pourcent et et dans le reste du monde. C'est en 2ème lieu une révolution technologique majeure. Qui va bouleverser le travail, les entreprises. Et les conditions mêmes de la croissance. Et c'est enfin une incertitude sur le commerce international, avec des risques de retour du protectionnisme du côté des États-Unis ou du côté de la Chine qui pourrait affecter ce retour de la croissance. Face à cette situation, quels sont les grands choix de politique économique que nous avons pris avec le président de la République le 1er ministre et le ministre des comptes publics. Le 1er grand choix. C'est de profiter de la croissance économique pour engager la transformation économique de notre nation, devant laquelle nous avons reculé depuis trop longtemps. Quand nous regardons aujourd'hui ce que la France est capable de faire en terme de croissance. Elle fait systématiquement moins bien que ses voisins européens. Et surtout systématiquement moins bien que ce qu'elle pourrait faire avec son potentiel de croissance de technologies de savoir-faire de travail d'entrepreneur. Eh bien, nous estimons que c'est parce que les choses vont mieux qu'il faut engager les transformations économiques nécessaires du pays alors que d'ordinaire, lorsque les choses vont mieux, on estime que ça permet de repousser les décisions nécessaires. La 2ème grande orientation que nous prenons. C'est le choix de l'investissement pour l'innovation. N'est pas question que nous manquions la nouvelle révolution technologique en cours comme nous avons manqué il y a une vingtaine d'années, la révolution des logiciels qui a conduit aux États-Unis à la création de grands groupes mondiaux. Tandis que la France, l'Allemagne, les autres pays européens étaient incapables de profiter à plein de cette révolution des logiciels. Aujourd'hui, nous voulons que face à cette révolution des données de l'Intelligence artificielle de la robotisation, la France, l'Allemagne, tous les pays européens puissent profiter à plein de cette révolution technologique pour gagner en croissance et gagner en emploi l'innovation sera donc au coeur de notre stratégie économique. Enfin 3ème grande orientation. C'est la défense d'un commerce équitable. Fondée sur des règles de réciprocité. Nous refusons que certaines grandes nations et accès aux marchés publics français sans que nos entreprises françaises est accès aux marchés publics de ces grandes nations, nous refusons que des grandes nations accorde des aides d'État à des entreprises dans le secteur des énergies renouvelables, par exemple, alors que nous, en France ou en Europe, nous n'aurions pas les mêmes facilités pour soutenir nos entreprises, le principe de réciprocité, le refus du dumping des règles identiques pour tous, doivent être au coeur du commerce international, toutes ces décisions. Doivent nous permettre de retrouver une croissance économique et la création d'emplois, nous avons perdu depuis trop de temps. Et elles doivent profiter à tous les Français. Sans exclusive. Il s'agit pas d'avoir d'un côté, une France qui gagne. Et de l'autre, une France qui perd. perd. S'agit pas d'avoir d'un côté, la France des métropoles des grandes universités et laboratoires de pointe. Et de l'autre une France des territoires oubliés qui ne s'en sort pas. Notre stratégie économique doit profiter à tous les Français. à tous les territoires. Elle doit permettre à chaque Français de retrouver la prospérité et le chemin du travail. La première grande orientation par conséquent sera de lancer une transformation économique de notre modèle économique et social pour nous permettent de créer plus d'emplois. Vous êtes en train d'étudier le projet de réforme du code du travail qui correspond exactement cette possibilité pour nos entreprises d'embaucher plus facilement qu'elle ne le faisait jusqu'à présent, cette refondation du marché du travail qui est porté par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, c'est la mère de toutes les réformes parce que c'est celle qui permettra de libérer la capacité d'embauche de nos entrepreneurs. Cette réforme n'est pas. La réforme définitive, à laquelle s'arrêterait le gouvernement pour les années à venir. Suivront une transformation de l'assurance chômage. Une réforme des régimes de retraite. Une transformation du système de formation professionnelle, qui aujourd'hui ne permettent pas à tous les salariés de trouver la formation dont ils ont besoin. Nous porterons également dans notre modèle économique des transformations indispensables pour faciliter la vie des quotidiennes des entrepreneurs pour simplifier leur vie pour alléger les contraintes pour éviter la sur-transposition des directives qui nuit tant à tous les entrepreneurs dans le secteur industriel en particulier mais aussi dans le secteur agricole. Nous porterons en 2018, un projet de loi sur les PME et TPE qui doit nous permettre en France de disposer d'entreprises de taille intermédiaire capable d'exporter et de retrouver un esprit de conquête sur les marchés extérieurs, ce projet de loi, je vous invite à y participer tous toutes les propositions. Toutes les suggestions. Toutes les idées nouvelles qui permettront à nos entreprises de grandir et de franchir le seuil critique qui leur permettra d'exporter, nous les retiendrons dans ce projet de loi et entre septembre prochain et décembre prochain j'ouvrirait la voie à une grande consultation avec les parlementaires avec les acteurs économiques, avec les entrepreneurs, avec les représentants syndicaux avec les chercheurs avec tous ceux qui veulent construire avec nous un tissu d'entreprises de taille intermédiaire aussi solide et aussi durable que celui qui existe en Allemagne. Enfin, nous engagerons un plan favorisant l'innovation de rupture, financée par la cession d'actifs de l'État. Nous engagerons à partir de septembre prochain. La cession d'actifs de l'État dans une entreprise du secteur concurrentiel, pour un montant de 10 milliards d'euros. Parce que j'estime que l'argent de l'État. Et mieux placé dans l'innovation et en particulier dans l'innovation de rupture, plutôt que dans des entreprises pour toucher régulièrement des dividendes qui ne participe pas à la croissance et la création d'emplois dans notre pays, nous avons besoin de financer innovations de rupture, celles qui coûtent trop cher aux entreprises, celles qui nous permettra de forcer les portes de l'avenir, ce qui nous permettra de rattraper notre retard sur les nations les plus innovantes, comme les États-Unis ou comme la Chine. La 2ème grande orientation. Ce sera la réduction de déficit pour répondre à nos engagements européens, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin détaillera pour 2017 et les années à venir, les décisions qui ont été prises en matière de dépenses publiques, je tiens simplement à rappeler, dans le cas de notre stratégie économique, pourquoi cette décision politique était essentiel, j'entends bien ce qui nous disent : il faut absolument préserver la dépense publique dans tous les secteurs, parce que elle est un facteur de croissance est un facteur d'emplois. Mais si véritablement la dépense publique était un facteur de croissance est un facteur d'emplois. La France qui a le niveau des dépenses publiques le plus élevé de tous les pays européens auraient la croissance la plus forte et le chômage le plus faible, alors qu'il y a le chômage, le plus haut et la croissance parmi les plus faibles, il est temps de changer de stratégie, parce que nous avons vu au cours des 20 dernières années, plus de dépenses publiques ne se traduit pas par plus employes et plus de croissance, mais par moins de croissance et toujours autant de chômage pour les Français. La 2ème, raison pour laquelle nous voulons baisser la dépense publique. C'est parce que nous tenons à respecter enfin nos engagements européens et c'est vrai qu'il aurait été beaucoup plus facile pour Gérald Darmanin pour moi-même, pour le 1er ministre, le président de la République de faire comme il a toujours été fait dans les années passées, de dire : mais regardez les horreurs. Car fait le précédent gouvernement, le précédent président de la République, c'est tellement lourd, c'est tellement difficile, nous ne pouvons pas respecté pour 2017 nos engagements européens et nous renvoyons cela aux calendes Cette méthode de fuite et de lâcheté qui consiste à se tourner vers le passé, alors que c'est l'avenir qui intéresse les Français, je refuse que nous nous engagions dans cette dans cette voie, nous avons décidé de tenir nos engagements européens en 2017, nous avons décidé de respecter les 3 pourcent et et nous le respecterons parce que c'est la condition de la crédibilité de la parole politique de la France sur la scène internationale. Tous ceux qui nous disent. Que ce n'est pas important. Ce sont les mêmes qui nous supplient de modifier la directive sur les travailleurs détachés. Bien sûr qu'il faut modifier la directive sur les travailleurs détachés, bien sûr que cette directive provoque du dumping social affaibli le secteur du transport affaibli le secteur du bâtiment et des travaux publics, mais comment voulez-vous que la parole de la France souhaite entendu sur la modification de la directive travailleurs détachés, si d'un autre côté, nous ne sommes pas capables de tenir nos engagements européens les plus élémentaires, comme la réduction de la dépense, réplique et la réduction de notre dette, nous tiendrons donc nos engagements, nous réduirons notre difficile budgétaire en 2017 comme en 2018, Geraldo Darmanin précisera les économies de 4,5 milliards d'euros que fera l'État sur son seul budget. Cette décision elle est majeure. C'est une décision fondatrice et c'est une condition de la crédibilité de la parole politique française sur la scène européens. Nous estimons en même temps que nous pouvons réduire la dépense publique. Et réduire les prélèvements obligatoires. Et que faire les 2 en même temps, dès 2018 est la condition du rétablissement de la confiance des entreprises comme des ménages ne pourront pas demander des efforts, c'est la réduction de la dépense sans simultanément baisser la pression fiscale qui insupporte les Français. Tous les engagements. Pris par le président de la République seront tenus. Nous en sommes avec Gérald Darmanin les comptables. Les engagements sur la baisse de la dépense publique, ils seront tenus. Les engagements sur le respect. De nos règles européennes, ils seront tenus. Nos engagements en termes de trajectoire budgétaire, ils seront tenus. Dans tous les secteurs. Notamment le secteur de la Défense et des armées. Le président de la République a fixé un objectif de 2 pourcent de de la richesse nationale pour le budget des armées d'ici 2025, avec un effort qui portera ce budget à 50 milliards d'euros d'ici 2025 nous sommes ici les comptables de cet engagement, la trajectoire sera tenu et les engagements vis-à-vis des armées seront rigoureusement respectée. Au-delà de ces réformes fiscales. Il faut donner le sens des décisions que nous prenons. Le 1er sens que nous donnons à ces transformations fiscales, c'est d'abord la valorisation du travail. Vous tous ici, qui a été représentant des territoires tous les jours vous rencontrez de ces hommes et de ces femmes qui partent travailler le matin, de ces femmes seules qui doivent faire garder leurs enfants qui doivent payer pour la garde de leurs enfants qui prennent leurs voitures qui vont travailler, qui rentrent le soir, qui touche 1200 ou 1300 euros Net par mois et qui vous disent : nous ne supportons plus de savoir que si nous étions restés chez nous sans travail et sans faire garder nos enfants sans dépenser de l'argent pour nous transporter, hé bien nous aurions mieux vécu des revenus de l'assistance, plutôt que des revenus de notre travail. Un pays dans lequel. Il vaut mieux rester chez soi, plutôt que de partir travailler est un pays qui n'a pas d'avenir. Nous voulons avec tout le gouvernement, faire en sorte que le travail paye. La suppression des cotisations maladie les cotisations chômage à partir de 2018 pour tous tous les salariés de France est une façon de lancer un message politique clair le travail en France doit payer. Cette baisse des prélèvements obligatoires, elle vise aussi à favoriser la situation des ménages notamment, avec la suppression de 80 pourcent de de la taxe d'habitation qui sera engagée dès 2018. Elle vise en 2ème lieu à favoriser la compétitivité des entreprises françaises, parce que oui, ce sont les entreprises qui créent les emplois, pardon d'avoir enfoncé cette porte ouverte, oui c'est en améliorant la profitabilité des entreprises n'hésitent pas à le dire qu'elles pourront investir, innover et créer les emplois que nous sommes incapables de créer depuis trop longtemps nous baisserons donc le taux de l'impôt sur les sociétés qui sera réduit progressivement pour atteindre 25 pourcent,, à la fin du quinquennat et rejoindre donc la moyenne de taux d'impôt sur les sociétés dans les autres États européens nous supprimerons le CICE à compter des salaires versés en 2019 pour le le transformer en un allégement de charges pérenne et immédiat, plus facile et plus simple pour toutes les entreprises, la contribution de 3 pourcent sur sur les revenus distribués, il a été récemment condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne sera supprimé. L'ISF. Qui décourage investissement. Pour des recettes limitées à 4 milliards d'euros sera supprimée et remplacée par un impôt pesant uniquement sur les valeurs immobilières de façon à encourager l'investissement, l'innovation, l'audace et la prise de risque. Un prélèvement forfaitaire unique de 30 pourcent sur sur les revenus du capital sera instaurée en lieu et place des dispositifs actuels qui sont trop complexe et illisible, cela favorisera aussi l'attractivité d'autres territoires pour l'investissement et donc le financement de l'innovation. Enfin, la dernière grande orientation de ses choix fiscaux. C'est faire avancer la transition écologique et réviser la fiscalité énergétique. La composante carbone de la TI CPE sera donc augmenté de façon plus ambitieuse que ne le prévoit la loi sur la transition énergétique et nous ferons converger le prix du gazole avec le prix de l'essence parce que je ne vois pas au nom de quoi le gazole aujourd'hui aurait une fiscalité plus favorable que celle de l'essence cette convergence ou la feront progressivement, nous le ferons en tenant compte de la situation des territoires ruraux et en continuant à soutenir les transporteurs et les agriculteurs et nous la ferons en aidant les ménages les plus modestes pour qu'ils ne soient pas affectés par cette mesure. Enfin, en termes de calendrier, je tiens à dire que nous souhaitons avec Gérald Darmanin avec l'ensemble du gouvernement avec le 1er ministre avancer vite. Figureront donc dans le projet de loi de finances 2018 qui vous sera soumis la suppression du CICE en 2019 la trajectoire de baisse du taux de l'impôt sur les sociétés jusqu'en 2022 pour le le ramener à 25 pourcent,, la suppression de la contribution sur les revenus distribués, la suppression de l'ISF et son remplacement par l'IFI, le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, la première réduction de la taxe d'habitation, l'extension du Champ d'application des régimes d'imposition simplifié et la hausse des tarifs de TI CPE et de TI CGN nous voulons aller vite, nous voulons aller loin, nous voulons aller fort parce que, comme je vous le disais en ce début d'intervention, c'est parce que la croissance frémit et parce que les augures sont un peu plus favorable qu'il faut en profiter pour accomplir la transformation économique, notre pays devant laquelle nous avons trop longtemps reculé, je vous remercie. Merci monsieur le ministre. La parole est maintenant monsieur Gérald armé d'un ministre de l'action et des Comptes publics.

nous avons à la fois étudier mesdames et messieurs les sénateurs, le débat dans Action des finances. Public et en même temps, si j'ose dire, la loi de règlement, nous aurons donc à étudier en même temps, le passé et l'avenir, à nous éclairera, j'en suis sûr pour retenir les mauvaises leçons du passé afin que l'avenir soit plus radieux que nous dit le passé de dit cette loi de règlement je m'arrêterai à 3 éléments : un déficit

a annoncé des montants dans son 1er discours mais donc je me suis ceux qui étaient devant la commission des finances, et je remercie d'ailleurs votre commission des finances, monsieur le rapporteur général d'avoir validé ses décrets d'avance et plus détaillé possible, même si nous avons tous regretté avoir prendre ces mesures de régulation en milieu de mandat

Et à stratégie que propose au gouvernement pour l'avenir, c'est le cas du texte que nous vous avons proposé, c'est à la fois de considérer qu'il faut dépenser moins, dépenser beaucoup moins et trouver dans les impôts et de taxes, non pas le refuge notre lâcheté mais les diminuer afin bien sûr de relancer l'économie et le pouvoir d'achat de nos concitoyens, nous allons donc mettre en place ce double choc voulue par le président de la République et le 1er ministre à la fois une baisse très importante de la dépense publique et je vous rappelle que le 1er ministre a rappelée à chacun des membres du gouvernement mais aussi dans ce discours de politique générale 0 pourcent ce ce qui n'est jamais arrivé sous aucun gouvernement avec le président de la République cet après-midi encore, dans son adresse aux armées a évoqué que seul le budget des armées cette augmentation, qui a évoqué tout à l'heure aux questions d'actualité, Monsieur le Président, le 1er ministre et en même temps, nous allons pouvoir diminuer ses impôts et ses textes nous a viendront nous pensons tous qu'il faut diminuer le déficit non pas pour faire plaisir à je ne sais quel hydre bruxelloise et parce que le problème, c'est le déficit, voilà des années que nous avons considéré maintenant quasiment 40 ans que le déficit était normal. Qu'il était normal de vivre en déficit, imagine-t-on un chef d'entreprise, une famille pendant 40 ans vit avec des recettes qui du coup voient pas ses dépenses et qui peut vivre éternellement en déficit c'était évidemment impossible ce déficit creuser notre dette notre dette qui, désormais, malgré des taux d'intérêt très bas, cela a été rappelé notamment par la cour une dette et des intérêts qui sont le 2ème poste de l'État bien avant, désormais, le budget de la défense et qui, bien sûr, pose à notre pays des difficultés très forte et devait par malheur devoir affronter de nouvelles crises et des remontées des taux d'intérêt moins dépensent moins d'impôts et de taxes, moins de déficit et pour demain, moins de dettes, c'est l'engagement du gouvernement dans le débat dans un sur les finances publiques d'aujourd'hui alors, ces engagements sont chiffrés, monsieur le rapporteur général, vous pourrez le vérifier à la fin du mandat, moins 3 points de dépenses publiques, moins 5 points de dettes et moins de points de déficit, nous avons des engagements extrêmement me semble-t-il, ambitieux et dès la loi de finances 2018 que gouvernement proposera, vous pourrez constater que ces baisses de dépenses et ces baisses de paiement obligatoire seront au rendez-vous, nos engagements sont simples, mais en même temps, difficile à tenir, puisque beaucoup de gouvernements ont essayé de les mettre en place, sans jamais pouvoir y y arriver complètement, mais je m'engage devant vous, monsieur le président du du Sénat, mesdames et messieurs les sénateurs, que nous présentons la finance sincère qui ne connaît pas les ASUS des sous-budgétisation

mais nous devons aussi considérer que, en sa série en ce budget les efforts d'économie sont d'autant plus grand que nous devons tenir ce 0 pourcent par par rapport à la loi de finances 2017 ici et je suis prêt en répondent devant les commissions des finances détail par détail présenteront noix finances sincère, selon les prévisions du gouvernement, en dehors des aléas qui pourraient toucher notre pays comme une retouche des pays malheureusement à travers le monde mais nous ne ferons pas de sous-budgétisation, deuxièmement, nous nous engageons à ne pas présenter de décrets d'avance devant les assemblées, ce que nous savons tous ce que le rabot, surtout lorsqu'il est-ce agit d'rabot de fin d'année est une mauvaise gestion, cet engagement est très important, très ambitieux, et en tout cas c'est une adresse que nous apportons, en tout cas, nous partons avec ce principe se rapportant général pour t-on pas faire cette mauvaise manière, même si elle est prévue par la LOLF nous aurons pas l'occasion de revenir vous voir en commission des finances sur ce sujet, troisièmement, nous pensons que la consolidation budgétaire reposera uniquement sur les dépenses et sur les baisses des dépenses, nous ne pensons pas que c'est la fiscalité ou d'autres mesures qui pourront régler cette consolidation budgétaire et nous aurons donc à trouver, c'est le chiffre me paraît difficile à tenir aujourd'hui mais quelques milliards pour ne pas dire plus de baisses de dépenses dès le projet de loi de finances 2018 pour tenir tenir cette consolidation budgétaire. La 4ème engagement que nous voulons vous dire ici devant l'assemblée des territoires, c'est que c'est l'État qui en 1er fera ses efforts, tout le monde fera des efforts, mais l'État en 1er et l'État fera plus de 50 pourcent la la diminution de la dépense publique l'année prochaine pour atteindre un peu plus de 40 pourcent les les années suivantes, nous avons bien compris les collectivités locales ont fait leurs efforts souvent contraints par les baisses de dotations, nous avons bien lu le rapport, la Cour des comptes qui expliquait dernières années c'était l'État qui n'a pas fait ses efforts, nous allons faire plus de 50 pourcent des des efforts, le budget de l'État même si, bien sûr, toutes les autres administrations, y compris les collectivités locales, nous en avons parlé tout à l'heure, feront une partie de de cet effort, enfin, nous ne pensons pas que la stratégie du rabot soit une bonne stratégie et désespère les ministres, les parlementaires, qui contrôle l'action du gouvernement et considère que finance n'est pas respecté et directeur de programme, les agents publics même et nous souhaitons faire des réformes structurelles, c'est le cas, monsieur rapporteur général pour la sécurité sociale et pour l'ensemble des questions de santé et de maladie ou d'innovation, de nous permettre de changer profondément notre système de santé tout en garantissant la sécurité sociale aux Français mais aussi des la réforme de la loi du travail qui a été évoquée par le ministre Bruno Lemaire mais également le logement, la formation professionnelle, l'université a été dite par Abidal, ainsi que diverses interventions sociales, c'est pas des réformes structurelles que nous éviterons la politique du rabot et que nous trouverons nos économies durablement ses conséquences et je voudrais en terminer par là, Monsieur le Président, Bruno Le Maire l'a évoqué, je voudrais essayer de redire, c'est une baisse sans précédent de la fiscalité, je rappelle que dans le budget 2018 c'est 11 milliards 3 de dépenses fiscales décidées par les anciennes majorité que nous tiendrons comme promesse bascule du CIC reviendra bien sûr l'année d'après, mais déjà 6 à 7 pour le le CICE, une partie de l'impôt sur les sociétés et puis les promesses fiscales du président n'applique seront accomplis, nous l'avons évoqué sur la taxe d'habitation, une première tranche dès l'année prochaine 3 milliards d'euros, mais aussi la question de l'ouverture de la fiscalité locale et de son avenir, l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les sociétés pour passer à 25 pourcent le le prélèvement forfaitaire unique et bien d'autres, a évoqué monsieur de mise, Économie et finances, sans oublier l'exonération des heures supplémentaires dans les prochaines années, de ce mandat, tous les projets fiscaux du président de la République seront tenus par mauvaise des cultures ou peut-être par critique un peu facile du gouvernement que ce sont des mesures pour les riches, je voudrais vous dire que l'ambition sociale du gouvernement est extrêmement forte, notamment pour les classes populaires et les classes païenne nous allons augmenter l'année prochaine la location adultes handicapés en à-coups pour plus de 100 euros par mois, ce qui n'aura jamais été fait et qui sera je crois une bonne politique, à la gare de nos concitoyens qui connaissent malheureusement un handicap et un empêchement de travailler à cause de son handicap, le minimum vieillesse sera puisqu'il prévoit aussi une augmentation de 100 euros la prime si j'ose dire, au travail, comme l'évoquait, Bruno Le Maire, c'est 260 euros pour un ouvrier au SMIC, qui va connaître par an, de pouvoir d'achat grâce à la baisse des cotisations sociales 500 euros pour un indépendant qui gagnerait 3000 euros grâce à cette même rénovation pour les cotisations, la prime d'activité, c'est 80 euros par mois supplémentaires pour ce qui la toucheront et la suppression de la taxe d'habitation pour 80 pourcent c'est en moyenne 550 euros de pouvoir d'achat supplémentaire à la fois gouvernement qui dépensent moins, qui dépensent moins pour moins d'impôts et qui dépensent pas mois, en faisant moins d'impôts pour qui est effectivement plus de gens au travail et que ce travail puisse étayer voici tout à stratégie du gouvernement, je vous en remercie. je vais maintenant donner la parole au rapporteur général de la commission des finances Monsieur Albéric de Montgolfier.

examiné l'exécution l'année 2016 et en même temps, débattre lors de son nos finances publiques pour l'avenir et il est vrai que, cette année, ce débat présente un caractère un petit peu particulier car de constituer l'occasion pour le gouvernement, et nous avons eu à l'instant, allons développement l'occasion développer les grandes orientations des finances publiques pour la législature, je voudrais d'abord revenir très brièvement sur l'année 2016 mon temps de parole est très limité, et je vous renvoie au rapport écrit qui est très détaillé néanmoins l'an passé, la croissance était levée, vous le savez, à seulement 1,2 pourcent c'est c'est un résultat qui est très décevant au regard des prévisions, la loi de finances initiale qui était de 1,5 pourcent mais mais aussi des parts performance de nos partenaires de la zone Euro qui ont enregistré une croissance de aviez autre contre-performance tient essentiellement à la contribution très négative du commerce extérieur, nous avons non seulement des difficultés en termes de compétitivité coût mais aussi en termes de compétitivité hors coûts et c'est un point crucial : j'ai entendu ce qu'à dit Bruno Le Maire le garnement doit s'attaquer pour que la France tire tout le profit possible du redémarrage de la croissance internationale, j'en viens maintenant à la situation des comptes publics en 2016 et sur ce plan, le diagnostic est sans appel la légère amélioration du déficit public masque un relâchement de l'effort public des comptes de redressement des comptes publics en effet ramener le déficit à 3,4 pourcent correspondait dans la recommandation du Conseil à une réduction de 0 6 point de PIB par rapport à 2015, finalement, cette réduction n'a été que de 0 2 points, c'est-à-dire 3 fois moins,

en 2016, les collectivités territoriales ont ainsi porté 60 pourcent de de la réduction du déficit 3,1 milliards alors qu'en comptabilité nationale, le déficit de l'État s'est dégradé la baisse très modérée du déficit budgétaire de l'État, soit avec 5 milliards d'euros résulte d'économies de constatation sur les prélèvements sur recettes et sur la charge de la dette, la dette publique qui continue d'augmenter et notre écart de niveau d'endettement avec l'Allemagne c'est démontré pour les collègues de la commission des finances s'élève désormais à 28 points de PIB je revois également un rapport sur l'analyse des recettes et en viens pour les dépenses au respect de l'autorisation budgétaire. Les principaux déplacements dépenses portent sur des missions que nous connaissions bien travail emploi défense solidarité enseignement scolaire agriculture ces sous-budgétisation avait été largement pointées par les rapporteurs spéciaux du fait de ses insuffisances 2016 a été marquée par un usage intensif des outils de régulation budgétaire comme la mise en réserve de crédits toujours plus élevés, les annulations, les ouvertures par voie évidemment de décrets d'avance ou encore les reports qui pèseront sur 2017, en conclusion, la loi de règlement qui nous est présenté pour 2016 traduit une gestion passée, dont la responsabilité incombe au Président de gouvernement, nous ne pouvons Speer et que ce nouveau gouvernement, en tire les leçons pour mieux préparer l'avenir tant d'efforts de redressement de Spinoza, finances publiques que de sincérité budgétaire et j'ai bien entendu Monsieur ministère Starmania les engagements quant au décret d'avance, mais là, je demande à voir, en tous les cas on on entend aujourd'hui ça engagement passons justement à l'avenir pour 2017 l'hypothèse de croissance révisé à la hausse

pour la suite du quinquennat le scénario retenu est de de croissance me paraît raisonnable en 2018 Compte-tenu de ce que nous connaissons déjà, mais plutôt optimiste pour 2019, 2022, en tous les cas par rapport aux prévisions de la Commission européenne de même s'agissant des hypothèses de croissance potentielle et des Cars de production que la précédente majorité avait fortement surestimée, il faut se féliciter que le garnement reviennent à des estimations plus prudentes, comme vous le savez, le 1er défi du garnement consiste à contenir le déficit public à 3 pourcent du du PIB afin d'ouvrir la voie à une sortie de la France du volet correctif du pacte de stabilité dans cette perspective, le garnement annoncé la mise en oeuvre des mesures correctrices 4,3 milliards d'euros, dont aujourd'hui je note que seulement 3,5 milliards d'euros sont documentés il retient une élasticité plus forte des recettes à la croissance lourdement espère sans doute une bonne nouvelle du côté des recettes, ce n'était pas au rendez-vous des mesures de régulation supplémentaires devraient être prises, faute de quoi nous notre réveillon pas les 3,1 pourcent Pour 2018 le garnement souhaite désormais mettre en oeuvre immédiatement et ça nous a été confirmée à l'instant, les baisses d'impôts annoncées lors de la campagne présidentielle, tout en assumant l'héritage fiscal mais là, c'est un bon héritage de la présente majorité aussi il entend procéder an à à une baisse des impôts pour un montant qu'il estime à 0,6 point de PIB en 30 ans, je note qu'une telle baisse des prélèvements n'est observée qu'à 3 reprises, du fait de ces contraintes, le redressement des comptes publics serait donc très progressif sur la première partie du quinquennat le déficit structurel se maintiendrait donc à 2,2 pourcent du du PIB en 2018 avant de se réduire lentement ses trajectoires semble néanmoins difficilement compatible avec nos engagements européens, de même le critère de dette ne serait pas respecté en 2021 quand il deviendrait pleinement applicable à la France et nous devrions donc connaître une nouvelle art divergence de nos taux d'endettement avec l'Allemagne. J'en viens maintenant à une question centrale : en effet, compte tenu de la nécessaire diminution des prélèvements obligatoires à la stratégie de redressement des finances publiques repose ce nous était confirmée à l'instant exclusivement sur la maîtrise des dépenses publiques, concrètement, ce sont donc 82 milliards d'euros d'économies qui devraient être réalisées sur l'ensemble du quinquennat dont 20 milliards d'euros sur chacune des années 2018 à 2020 c'était serait inédit 2011 et c'est la seule année au cours de laquelle une quasi-stabilisation de la dépense publique, a-t-il pu être observés, j'ai entendu tout à l'heure en effet comme vous aux questions d'actualité, le 1er ministre qui a dit : stabilité, sauf pour le ministère de la Défense, même dans le scénario dérapage limité de dépenses, le déficit dépasserait évidemment largement les 3 pourcent du du PIB en 2019 années de lait au cours de laquelle le CCE doit être transformé en baisse de charges je vous ai d'ailleurs interrogé Monsieur Mini-je viens maire mis à l'instant, la lettre de réponse sur l'impact en points de PIB de cette mesure, je comprends qu'à ce stade les les taux qui sera retenu et les effets du retour d'impôt sur le super ne sont pas encore pleinement arbitrer et la peur en tout état de cause, indispensable d'adopter sans tarder une stratégie crédible de maîtrise de la dépense publique et donc vous s'efforce de dresser les contours à cet égard, 3 grandes orientations semble particulièrement pertinente, il faudra d'abord ciblé les politiques publiques pendant laquelle la France dépense significativement plus que ses voisins et en effet je suis d'accord avec vous la logique du rabot ne pourra pas suffire pour, a-t-il niveau d'économie si on compare simplement les ratios, dépenses publiques de la France avec l'Allemagne et peut-être noté que 3 secteurs, explique l'essentiel de l'écart, les retraites, le chômage et le logement, bien évidemment, cela ne doit pas conduire à laisser penser que, dans tous les autres secteurs, aucune économie ne pourraient être réalisées. En complément, il sera également sans doute difficile de faire l'économie d'une réforme visant à maîtriser la masse salariale de l'État et à cet égard, je tiens à vous rappeler les propositions formulées par le Sénat lors de l'examen, loi de finances pour 2016, nous avions fait des propositions à cet égard en matière de temps de travail dans la fonction publique en matière de jour de carence y a déjà une annonce Monsieur Michel ministère maintenant et il est en effet indispensable de mettre en place une gouvernance enfin adapté pour associer l'ensemble des acteurs de la sphère publique à l'effort de la Redoute des premières annonces ont été faites en ce sens, j'ai assisté aux états généraux des comptes de la nation, l'autre jour à Bercy, j'ai assisté aussi à la conférence nationale des territoires ici même monsieur présent du Sénat mais il faudra veiller à ce que ces structures ces instances ne deviennent pas des instances purement formel ou le gouvernement viendrait uniquement présenté des décisions déjà actée en tous les cas, nous y serons vigilants, je vous remercie.

monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires des finances monsieur le président de la commission des affaires sociales, rapporteur général des finances, chers collègues, avant d'évoquer plus précisément les comptes sociaux, je voudrais indiquer que la commission des affaires sociales partage votre appréciation, Monsieur le Ministre sur selon laquelle il est nécessaire de nous projeter prioritairement dans l'avenir. Mais il me semble néanmoins nécessaire aussi de consacrer du temps à l'examen de la gestion passée, c'est particulièrement vrai. Pour les lois de financement de la Sécurité sociale, qui sont des exercices de prévision et pour lesquels l'exécution et rapidement évoqué dans les textes relatifs aux exercices suivants ou hors du Parlement dans le cadre très formel et plutôt dater date de 1979 de la commission des comptes de la Sécurité sociale. faut rénover ce cadre, monsieur le ministre et l'intégrer, selon l'expression consacrée, dans un schéma j'vertueux qui se décline depuis les engagements européens de notre pays dans le cadre des assauts les administrations de Sécurité sociale jusqu'au régime général de la Sécurité sociale, qui fait l'objet du Plfss les régimes à gestion paritaire, les hôpitaux, l'effort en faveur des personnes âgées et handicapées ne doivent plus constituer des angles morts de nos finances publiques dont les comptes ne serait être retracée dans aucun texte alors que notre pays s'engage aussi sur les résultats de ces entités. Je vois l'intérêt, comme cela est évoqué dans le document préparatoire de ce à ce débat, qu'il pourrait y avoir à renforcer le lien entre les vols et recettes des des différents textes financiers, même si à la suite des réformes des efforts récents la TVA demeure la seule recette partagée entre l'État et la sécurité sociale, je m'interroge toutefois sur les modalités de ce renforcement dans l'état actuel des textes organiques et dans la séquence actuelle des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, au-delà des rapprochements qui pourrait s'opérer, il existe bien une spécificité des finances qui tient notamment à la pas encore très majoritaire que prennent les cotisations sociales dans le financement de ses prestations pour en venir au comptes sociaux, le gouvernement a fixé à un horizon de retour à l'équilibre du régime général en 2020, cet objectif nous semble à la fois réaliste exigeant réaliste parce que la marche à franchir qui est de 5 milliards 5 d'euros n'est pas si élevé est sans commune mesure avec le déficit de l'État. Mais cet objectif est exigeant, parce que la dynamique des dépenses dépenser forte tandis qu'à qu'très court terme, les baisses de recettes sont d'ores et déjà engagés. Pour 2017, le déficit devrait se réduire, moins que prévu mais sa réduction devrait attaquer si les dépenses ne connaissent pas d'accélération au second semestre. Pour 2018 l'équation paraît difficile, les résultats 2016 et 2017, moins bons que prévu, se reporteront sur l'exercice, tandis que les les temps que des tensions sont d'ores et déjà prévisibles. En recettes la prévu la révision de l'hypothèse d'évolution de la masse salariale que vous avez signalé devrait se traduire par de moindres recettes d'un 1000000000 4 d'euros auxquels s'ajoutent les effets des mesures nouvelles crédit d'impôts, de taxes sur les salaires, contrecoup des acomptes de ces 3 et de taxes sur les véhicules de société. Ce qui fait un total de un en dépenses, la nouvelle convention médicale pèsera encore davantage sur l'Ondam soins de ville, tandis que le protocole peut PCR augmente les charges des hôpitaux publics, au total ce sont près de 4 milliards 5. Il faudra trouver en recettes ou en moindres dépenses à cet égard le document préparatoire nous informe que chacun des sous-secteurs devra contribuer à la baisse de la dépense publique pour la part des dépenses qu'il représente dans le PIB pour les assauts, si mes calculs sont exacts, cela représente 32 milliards d'euros sur 5 ans dont 8 milliards dès 2018. La commission des affaires sociales a formulé des propositions, notamment sur l'assurance maladie ou des gisements d'efficience restent à exploiter dans l'organisation des soins, mais sur ce point, le document ne nous en ne nous informe pas davantage, il trace en revanche quelques pistes qui suscite de notre part des réflexions et des sujétions monsieur ministre je voudrais ainsi évoqué l'assurance chômage, dont le gouvernement souhaite étendre le bénéfice aux travailleurs indépendants, certains indépendants souscrivent déjà de telles garanties à titre volontaire pour des montants et des durées d'indemnisation variable avec des cotisations éligible un à des avantages fiscaux. La définition crucial de la privation involontaire d'emploi est en général entendu assez strictement redressement judiciaire, liquidation ou cession judiciaire fusion-absorption Restructuration profonde révocation ou non-reconduction du mandat social pour ne citer que quelques cas. Le projet du gouvernement semble beaucoup plus large. Pourriez-vous nous éclairer Monsieur le Ministre, sur son calendrier, ses contours et le cadrage général de son financement. Qu'envisagez-vous sur la question de la dette de l'assurance chômage qui s'élève d'ores et déjà à 30 milliards d'euros. Sur la question et qui sera certainement de de pas loin de 40 milliards à la fin de l'année sur la question des retraites : le Sénat s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur d'une réforme systémique et de l'instauration d'un régime par points plus équitable, plus facile à piloter, nous sommes donc sur ce point, en accord avec les évolutions annoncées par le gouvernement, au-delà de cette question d'organisation, la commission des affaires sociales a également alerté au cours de chacun des derniers Plfss sur la nécessité de reporter l'âge légal pour tenir compte de l'augmentation de l'espérance de vie et garantir la soutenabilité de notre système de retraite et la confiance des jeunes générations. Après la publication des nouvelles prévisions du COR, qui font état déséquilibre profond et persistant à court terme, le comité de suivi des retraites a préconisé la semaine dernière que des maires, des mesures correctives soient prises, elles sont sur ce sujet des retraites, les intentions du gouvernement. C'est sur ces jeunes générations que nous reportons le poids de la dette sociale, en prévoyant de le faire supporter demain des économies ou les impôts que nous ne souhaitons pas aujourd'hui, nous savons tous que la solution de portage des déficits de régime général par l'Acoss, ne peut être que transitoire la distribution ira-t-elle jusqu'à l'augmentation de la CRDS est une question Monsieur le Ministre, CRDS éventuellement gagées par la baisse d'autres prélèvements avec l'engagement ferme bien sûr de la restituer aux Français à l'échéance de 2024 qui a été confirmé par le gouvernement voici Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les principales observations et interrogations que je souhaitais formulée au nom de la commission des affaires sociales dans ce débat d'orientation merci beaucoup. Merci, monsieur le rapporteur général, avant de passer à la suite de la discussion générale, je vais donner la parole à notre collègue Claude Raynal. Monsieur le Président pour une rectification de vote sur le vote du projet de loi relatif à la sécurité publique, je vais vous indiquer que notre collègue Roger Madec avait entendu voter pour. Et nous vous donnons acte de votre mise au point qui sera publié au Journal officiel et figurera dans le lit politiques du scrutin dans la suite de la discussion générale, notre collègue Richard Yung

Monsieur le président, messieurs les Ministres, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Commencerait par la loi de règlement et je rappelle que la discussion sur la loi de règlement, c'est de regarder d'évaluer comment la loi de finances initiale éventuellement modifiées par les différentes lois de finances rectificatives et autres comment cette loi de finances, a été exécuté, c'est pas un débat sur le contenu de la loi de finances elle-même comme on voit parfois, on le voit, mais c'est une c'est une déviation de ce que doit être le débat et c'est ça qui nous intéresse parce que c'est au fond la façon de mesurer, d'essayer de mesurer l'efficacité des politiques mises en oeuvre,

l'inflation reste faible, ce qui est dommage puisque nous essayons nous avions pour ambition d'atteindre 2 pourcent d'inflation mais l'inflation la mais un peu à part, parce que ce n'est plus tellement entre les mains du gouvernement français c'est la Banque centrale européenne qui est active en la matière. Le point faible, le point le plus faible, je dirais, je crois que tout le monde le le sang, c'est toujours le commerce extérieur et en particulier la faiblesse de nos exportations et nous savons tous que ceci est dû non pas tellement à des ou à des raisons générales, on invoque les intempéries, on a invoque le ralentissement du commerce international, mais tout ceci, les autres pays aussi le vivent non c'est dû au fait que notre tissu de PME, ça a été légèrement touché par le ministre-n'est pas orienté exportation n'est pas orienté vers la productivité vers une productivité suffisante, nous rêvons tous au milieu, le stand allemand mais enfin comme tous les rêves, c'est quelque chose qui relève plutôt du souhait que de la réalité. Les dépenses sont couvertes par les recettes de façon tout à fait prévu

c'est-à-dire celui qui que l'on calcule en dehors de toutes les influences conjoncturelles extérieure de 1,6 pourcent et et ça, ça reste très élevé, ce que je vous rappelle que l'objectif communautaire le objectif du fameux traité et de 0 5

vous devriez donner un petit satisfecit à cette à cette amélioration sur les dépenses, je rappelle que la France est en déficit en procédure de déficit excessif depuis 2009 depuis 2009, ça fait presque 10 ans et chaque année il y a un débat avec la Commission, la commission est bonne fille en il y a un débat avec la Commission, qui dit : bon, vous avez pas encore tout à fait réaliser ce que vous aviez dit que vous alliez réaliser donc on vous donne une année de plus, c'est ça qui se passe comme comme des disputes familiales, je pense que le moment est venu d'agir de façon beaucoup plus, beaucoup plus sérieuse en la matière sur la question de la sous-budgétisation, nous en avons parlé avec lors du du rapport de la Cour des comptes.

C'est pas tout à fait nouveau, tous les gouvernements le font où l'ont fait, depuis, depuis 20 ans, c'est pas une raison pour continuer, c'était avant, ça c'est vrai que c'était avant et je suis sûr que ce nouveau gouvernement est décidé à prendre dans cette question à bras-le-corps et à faire en sorte qu'il n'y aura plus de sous-budgétisation. Une des questions qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on évalue cela une des discussions qu'on avait avec la Cour des comptes vous rappeler, c'est-à-dire bon il y a la Haute autorité qui a été créée, qui évalue les hypothèses de croissance, d'inflation, etc qui, semble-t-il, donne satisfaction et ce qu'il faut envisager que cette haute autorité ou une autre institution économique, au fond, donne un avis sur la butte les budgétisation qui sont proposés, c'est un des débats, je pense qu'il faut qu'on est et enfin je termine par une chose qui me tient à coeur, c'est s'effacer ces fameuses réserves de précaution ces fameuses réserves de précaution qui à mon avis, vide les discussions budgétaires de son sens, tout ce que nous faisons ici pendant 3 semaines à discuter les programmes de façon détaillée ne sert plus à grand chose puisque, comme vous savez,

donc moi je proposerai, je propose, puisqu'il y a plusieurs sujets de débat et d'ailleurs vous le vous le mentionnez dans le rapport sur les le le le chemin à moyen terme, je proposerai que nous ayons table ronde ou une façon de de consulter, de travailler ensemble pour revoir l'ensemble de ces procédures, à la fois d'élaboration du budget et d'évaluation, parce que je pense que la démocratie est à ce prix. Sur le, sur le chemin d'orientation à moyen terme de 2 3 choses : je crois que les hypothèses de croissance sont prudentes crédible 1,6 pour cette. Vous avez vu que le FMI vient de moindre, le gouvernement français de sa bénédiction pour l'année en cours, probablement pour les années qui viennent, donc. Nous nous réjouissons à Lille

une soudaine progression des recettes fiscales, ça c'est une bonne nouvelle, semblerait que le taux d'élasticité malheureusement notre ami François Marc, le spécialiste de l'élasticité fiscal n'est pas là mais les lester la liste ici fiscal, je vais y arriver. Et recalculé à la hausse. Donc nous respecterons, semble-t-il, les 3

vous demander de de préciser au moins les grandes lignes de votre plan de de réduction des dépenses, vous avez, vous prenez un implant de 60 milliards en 5 ans 25 milliards pour l'État c'était 17 13 milliards maintenant pour les collectivités territoriales et 25 milliards pour la sphère sociale, je dois dire que ça c'est quelque chose qui est quand même assez, assez gros, comme on dit, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur qu'est-ce qu'il y a dans dans ces dans ces différentes masses voilà mais sous sous réserve de ces, de ces observations nous considérons que mon groupe considère que le il peut approuver le plan à moyen terme. si on cherche relève. La parole est maintenant au président Thierry Foucaud pour le groupe communiste républicain et citoyen, il a 5 minutes.

Il faut sans tarder, sans faiblir, réduire la dépense publique, il faut sans IT avec le courage nécessaire : réduire la dépense publique, mais les 97000 bacheliers que je me permets de féliciter ici d'avoir si brillamment conclu lors scolarité secondaire qui se retrouvent dans la nature, par la faute d'une autonomie des universités, devenue une machine à exclure ou bien alors parlons des enfants qui ne verront jamais en classe d'école communale la dès 6000 enseignants qu'il n'y a pas été nommé depuis 5 ans, ou encore que les usagers des transports parisiens confrontés à peu près chaque jour aux pannes du matériel roulant, usure du réseau ou bien aux défaillances de la signalisation mais allons bon, il faut réduire la dépense publique, la chose est acquise et c'est la soi-disant la seule solution, malgré une baisse de la dépense locale en 2016, les collectivités locales vont devoir prendre à leur charge 13 milliards d'euros de baisse de la dépense publique, outre la disparition programmée de 80 pourcent de de la taxe d'habitation, rajouter aux 10 milliards de baisses de de de dotation sur la DGF ces dernières années, quoi de pire quoi de pire pour les collectivités, alors que j'entendais tout à l'heure aux questions d'actualité, un ministre réponde à une question à dire qu'il fallait encore diminuer les dépenses de fonctionnement, lorsque l'on sait que les dépenses de fonctionnement, c'est le gosse, électricité, c'est l'essence mais c'est surtout la masse salariale pour environ 50 à 60 pourcent des des collectivités que ces collectivités contre 5 millions de salariés, c'est un appel, c'est un appel à la réduction des des effectifs donc un chômage croissant pour la France, et en même temps, a annoncé, service public, qui puisse être assurée pour les populations alors la mesure est clair et lisible et le choix laissé aux élus locaux n'est que celui de la peine qu'ils auront en conscience décider de s'appliquer à eux-mêmes, avec ses 13 milliards quel formidable avancée

en fait environ 17 heures et demie de production de l'économie nationale et peut-être 35 heures de rendement des prélèvements fiscaux et sociaux, les engagements donc nous avions souscrit la auprès des instances européennes, l'insécurité invoqué des comptes publics ne fait d'ailleurs penser. Au collectif budgétaire de 2012 dans le dans le dossier, l'été, dit je cite il nécessaire de procéder à une rectification des prévisions de recettes, d'une part en raison de la révision à la baisse de la prévision de croissance. Et d'autre part, afin de corriger les erreurs manifestes de prévisions du gouvernement précédent, tels que 11 quel telles qu'elles ont été soulignés dans le dites rendu par la Cour des comptes, cela conduit à réviser à la baisse des prévisions de recettes publiques de manière significative, fin de citation ces observations, mes chers collègues, figurait donc en toute la dans le dossier de présentation du collectif budgétaire d'août 2012, que le gouvernement Hollande avait fait voter devant l'impasse des 7,1 milliards d'euros, je dis bien 7,1 milliards d'euros de pertes de recettes fiscales lors de son installation alors ne comptez pas sur nous, ne comptez pas sur moi pour accorder un brevet de bonne gestion des comptes. Public à l'équipe Hollande que le suffrage universel a été suffisamment sévères à cet endroit ne comptait pas plus sur nous pour donner quitus au choix que nous propose le gouvernement actuel, livre de recettes éculées qui, en 30 ans, on fait la preuve de leur inefficacité, oui nous sommes pour la baisse de la dépense publique, quand il s'agit par exemple de financer de financer. à fond perdu un crédit d'impôt, compétitivité, emploi, où chaque emploi coûte 200000 euros pièce, oui nous sommes pour la baisse de la dépense publique quand elle finance un crédit d'impôt recherche qui n'a nullement, relancé le budget recherche et développement des entreprises. Et qui n'a pas permis de créer de l'emploi, oui nous sommes pour la baisse de la dépense publique quand elle paie la ristourne dégressive sur les bas salaires, dont une une récente d'ailleurs publication de France Stratégie dit et là encore, je cite, en France, les travaux d'évaluation de la politique d'exonération de cotisations sociales patronales sur les bas salaires ont surtout cherché à mesurer son effet sur le volume de l'emploi, ils aboutissent globalement à conclure que la première vague d'allégement de 93 à 97 a permis de créer ou sauvegarder de de Delors de 300000 emplois et la 2ème vague environ 350000 emplois les effets de la 3ème vague de 2003 2005 serait quasiment nul, fin de citation alors que vous vous apprêtez-vous à faire Monsieur le ministre, car la Gendak fiscal du gouvernement comprend un certain nombre de dispositifs dont l'orientation est fondamental fondamentalement totalement exclusivement libérale rétablir un prélèvement libératoire pour les revenus du capital encore plus intéressant que celui qui avait disparu sous la gestion Hollande au demeurant quand on est de gauche que l'on soit communiste, socialiste progressiste, comment peut-on approuver une telle mesure qui va permettre à quelques dizaines de milliers de contribuables de se partager 1,5 milliards de baisses d'impôts. Pour les 280000 foyers fiscaux les plus riches la réforme fiscale macron Philips et 15000 euros de baisses d'impôts en 2018, rien à voir avec les 2 ans Euro moyen de baisse de la taxe d'habitation inscrit dans votre réforme quand on est de gauche progressiste, on ne peut pas admettre une quasi-liquidation de l'impôt de solidarité sur la fortune, au motif de financement des PME quand on compare ISF-PME 1 1000000000 par an Odon et montant Net des patrimoines impose à Bali, ISF, plus de 1000 milliards d'euros, quand on est de gauche progresse, ils sont se refuse à une politique fiscale qui va accroître les inégalités de Patrimoine financier et immobilier ou l'orientation budgétaire de 2018 celle donc de l'austérité, encore et toujours l'austérité, c'est-à-dire qu'en lieu et place d'une désintoxication de la dépense publique comme des prélèvements sociaux et fiscaux, nous allons avoir une fois encore la mise en cause du service public d'État comme du service public local, la dégradation de la qualité de vie des agents. Dont le traitement d'ailleurs va être gelé, et les droits attaquer celle des réponses apportées aux attentes des citoyens, c'est-à-dire que nous allons encore. Constaté des retards pris dans la réalisation des grands projets structurants dont notre pays a besoin pour avancer sur la voie de la transition écologique également, c'est-à-dire que nous n'allons pas engager des sommes nécessaires à l'indispensable prévision de la sortie du nucléaire, qui appellent des investissements spécifiques pour modifier notre gamme de production d'énergie, c'est-à-dire que nous n'aurons pas les moyens. Pour mener le vaste plan de mise à niveau des performances thermique des immeubles d'habitation attendue par nombre de familles modestes, soucieuses de leur facture de chauffage, c'est-à-dire que nous n'allons pas mettre en oeuvre le plan de réalisation d'équipements universitaires indispensable à la réalisation des capacités d'accueil des 3 millions d'étudiants qui seront inscrits dans les 10 années qui viennent, outre que nous ne voterons pas la loi de règlement du budget 2017. Nous ne pouvons que désapprouver la ligne imprimée à la gestion des deniers publics pour ce qui est de 2018, d'autant qu'entre cadeaux fiscaux aux plus riches et réduction du service public pour les autres, elle conduira à la récession.

Madame la présidente, monsieur Les ministres messieurs les rapporteurs, chers collègues, ce 1er débat budgétaire du quinquennat au coeur de l'été n'aurait sans doute eu que peu d'écho, si elle ne s'inscrivait dans le contexte des mesures prises par le nouvel exécutif et qui ont fait couler beaucoup l'homme ces dernières semaines, si, en l'absence de loi de finale ça rectificative, le parlement a peu de prise sur les mesures concernant l'année en cours, il n'en garde pas moins le droit d'en débattre les économies annoncées, parfois drastiques, notamment dans les grands ministères régaliens pour faire face à certaines dépenses inéluctables, sans dans toutes les têtes, la commission des finances, a rendu hier son avis sur les projets de décrets d'avance et d'annulation qui concernaient des sujets hélas urgentes telles que la recapitalisation d'Areva ou le financement des opérations militaires extérieures, les OPEX, le règlement du budget l'année passée, n'est quant à lui que la constatation d'un résultat, mais sur ce point, vous l'aurez compris leur ce a dans sa grande majorité soutenu l'action du précédent gouvernement approuvera également dans sa majorité, ce projet de loi de règlement en 2016, le produit intérieur brut s'est accru de 1 Birchwil 2 pourcent soit soit un résultat légèrement décevant par rapport aux projections établies en loi de finances initiale, mais aussi un loi rectificative mais c'est 0 1 point de plus que la croissance constatée en 2015 amélioration donc modeste mais réel, qui confirme la reprise constatée dans la seconde moitié du quinquennat Hollande

pendant la première moitié de 2012 à 2014 a connu une reprise modérée sur la seconde moitié le déficit public s'établit à 3,4 3,4 points de PIB, c'est là aussi un résultat légèrement décevant par rapport à la prévision moyenne 3,3 points en loi de finances initiale, mais qui reste malgré tout très proche. Au total, les déficits se sont réduits de façon continue depuis 2012 alors que la situation, faire de la France s'était beaucoup dégradé à la suite de la récession 2008 2009, sans toutefois atteindre l'objectif annoncé de retour en dessous des 3 pourcent et et de réduction du poids de la dette, le gouvernement votre gouvernement, Monsieur le Ministre, parviendra-t-il à sortir la France de son interminable crise de langueur, une crise qui combine depuis tant d'années de faible croissance, déficit contenu chômage est levé et forte pression fiscale, c'est en tout cas. L'ambition qui est affichée et je la salue l'encourage la même la soutient, car le défi à relever est immense Laurent douce compris, à ce titre, les mesures d'économies de 4,5 milliards d'euros annoncés par le ministre de l'action et des comptes publics

toutefois, on peut constater que les économies frappe émission considéré jusqu'à présent comme prioritaires, comme la sécurité ou la défense à effet les le ciseau budgétaires qui affectent, on le sait, la défense mais aussi des missions importantes comme l'aide au développement, budget budget sur lequel je suis particulièrement attentif, posant un problème à court terme, c'est pourquoi il doit permettre un redressement des comptes publics à moyen et long terme et je ne doute pas que ce soit la volonté des ministres à côté des mesures touchant des ministères : Bercy a pris d'autres mesures d'économie, gel du point d'indice, le rétablissement du jour de carence dans les fonds de la fonction publique, la réduction du nombre des contrats aidés et les mesures d'économies budgétaires sont toujours impopulaires, nous le savons, mais encore une fois, elles peuvent peut-être être rendu plus acceptable dans la perspective, le groupe globale de rétablissement des comptes pour 2018, le gouvernement l'affiche des objectifs non moins ambitieux 2 milliards d'euros d'allégements fiscaux qui dans le passé, notamment par la poursuite de la baisse de l'impôt sur les sociétés initié l'année dernière, nouvelle réduction des cotisations sociales, un resserrement inédit de l'assiette de l'Yacef la suppression de la taxe sur les transactions financières intra-journalières et bien sûr la 1ère étape de la suppression de la taxe d'habitation pour 80 pourcent des des ménages réforme

ces mesures s'accompagneront à l'inverse de certaines hausses de prélèvements, ceux de la CSG, des taxes sur le diésel, le tabac ainsi que de mesures non fiscales accroissement des recettes comme des cessions de participations de de l'État à hauteur de 10 milliards d'euros annoncée par monsieur le maire, toutes ces mesures risquent de frapper de façon différente, les ménages aisés, les ménages modestes, il est donc essentiel de s'assurer du service économique de ces mesures, autre point, le président de la République a décidé de reporter d'un an la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, il est vrai que les questions techniques mais aussi de déontologie imposées par cette réforme sont plus importantes qu'on ne pouvait l'imaginer au premières bord en commission des finances, tout ça ne nous avait pas échappé d'ailleurs son adoption dans la dernière loi de finale celui précédent un canard d'ailleurs quelque chose de surprenant mais tout aussi surprenant le choix du texte pour adopter ce report dans le projet de loi d'habilitation d'ordonnances sur le code du travail, n'aurait-il pas eu davantage sa place dans le collectif budgétaire, il est vrai que l'agenda resserré la priorité donnée à la réforme du marché du travail rendent messieurs les Ministres difficile examen tels texte à Millau d'année tout est question de priorité, le gouvernement souhaite c'est une demande de la population de réduire la pression fiscale sur les entreprises et surtout, surtout sur les ménages, mais il ne doit pas moins poursuivre, me semble-t-il, les efforts menés par la précédente majorité pour lutter contre la fraude fiscale qui est toujours estimée selon certains à 80 milliards d'euros par an qui était énorme de ces quelques remarques je retiré l'idée que si le gouvernement n'apparaît dynamique et sincère dans sa volonté de réduction des dépenses de la pression fiscale et de redressement des comptes publics, il manque peut-être une vision de plus long terme de ce vers quoi il entame nous mener à l'horizon des années prochaines ainsi le grand sujet de la redéfinition des missions et du périmètre de l'action publique doit être abordé le débat d'orientation des finances publiques et me semble-t-il le moment privilégié pour cela puisque nous avons le recul et l'expérience des exercices passés et du temps pour la réflexion, avant le dépôt à l'Automne, du projet de loi finance je vous remercie de votre attention. la parole est maintenant à monsieur Claude rénal pour le coup peu socialiste et républicain. Et vous aurez la parole pour 13 minutes maximum.

Madame la présidente, messieurs les Ministres, Monsieur et les rapporteurs, mais, mais, cher collègue, quelques mots tout d'abord au au nom de Yves Daubigny pour le budget des comptes sociaux, puis je compte poursuivre et par le sujet qui nous occupe ce rôle, la loi de règlement pour 2016 et les recettes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse se compose pour l'essentiel des 205 milliards de cotisations sociales de 89 milliards de CSG de 46 milliards d'impôts, taxes et autres contributions cette diversité des ressources ne saurait tout de fois remettre en cause la spécificité des finances sociales si elles conduisent comme toutes les finances un équilibre de dépenses et de recettes sont liées à la recherche à la science, à la prise en charge des accidents de la vie aux solidarités et donc profondément à l'humain et un autre vivent ensembles 3 caractéristiques distinguent la France a matière de finances sociales la première et le niveau d'engagement financier pour 2015 la couverture ou la réparation des risques sociaux ont atteint le montant de 700 46 6 milliards d'euros, soit 34 pourcent du du PIB sur un montant total de dépenses de 1000 la 2ème caractéristique et le faible niveau de reste à charge supportée par nos compatriotes en matière de dépendre santé la variabilité de ce reste à charge, suivant le type de soins sa progression en valeur absolue, les frais optiques et de prothèses dentaires génère en ressenti éloigné de cette comparaison, pourtant favorable avec les autres pays de l'OCDE, la dernière caractéristique, il convient d'évoquer ici et l'existence d'une dette sociale unanimement considéré comme insupportable car concernant nos dépenses courantes de protection sociale, par ailleurs, la dégradation constatée de un virgule 3 milliards d'euros de la situation financière 2000 17 du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse par rapport à la prévision de fin 2016 ne doit pas masquer la maîtrise des dépenses et à trajectoire de réduction du déficit de la Sécurité sociale, sur la période 2012, 2017, le déficit du régime général était de 13,3 milliards d'euros en 2012, il est de 4,1 milliards d'euros en 2016 et devrait se réduire à 1,6 1000000000 en 2017, le déficit global, régime général font solidarité vieillesse était de 17,5 milliards en 2012 et devrait se réduire à 5,5 milliards 2017, la branche accidents du travail, maladies professionnelles affiche un solde positif depuis 2013, la branche retraite après plus d'une destinée de déficit est redevenue excédentaire en 2016, la branche famille retrouvera un excédent en 2017 pour la la première fois depuis 10 ans, l'inquiétude persiste pour le Fonds de solidarité vieillesse dont le déficit malgré une baisse sensible de ses charges en raison d'une forte baisse de ses recettes, assises sur les revenus du capital s'aggraverait à nouveau en 2017 atteignant 4 milliards d'euros ainsi notre pays éprouvent de grandes difficultés à équilibrer sa branche maladie qui a vu en 2016, la mise en place de la protection universelle maladie branche dont le déficit s'est réduit d'un 1000000000 en 2016 mais devrait encore dépasser 4 milliards en 2017 la santé mentale, la prise en charge des cancers, des maladies cardio-neuro-vasculaires et du diabète constituent les pathologies qui engagent les plus importantes, prise en charge après les hospitalisations ponctuelles, un nombre croissant de personnes vivent avec une ou plusieurs pathologies chroniques, parfois en situation de dépendance ou de handicap, notre système de santé doit donc évoluer pour mieux accompagner ces personnes dans leur lieu de vie, leur fournir des soins de qualité coordonné continue dans le temps, il s'agit d'un défi organisationnel majeur qui appelle une restructuration profonde de l'organisation des soins, relever le défi de l'équilibre de la branche maladie de la Sécurité sociale n'est pas affaire d'experts mais nous concerne tous, patients, professionnels de santé, responsables politiques, quand l'exercice médical et soignant mais toujours la vocation médicale de l'homme, selon Emmanuel Lévinas, comme l'impossibilité de passer son chemin lorsqu'il s'agit de solitude, de souffrances et de morts, selon Alain Cordier. Voilà ce que souhaitez nous dire mon collègue Yves Daudigny qui au dernier moment, n'a pu être. Nous complétons je voudrais compléter maintenant son propos par quelques mots sur le projet de loi de règlement et sur le débat de l'orientation des finances publiques, l'examen de ce projet de loi de règlement doit d'abord être l'occasion de répondre à 2 questions essentielles : quelle est l'évolution des finances publiques d'exécution exécution des objectifs fixés par le législateur, ont-ils été atteints, force est de constater que ça en 2016, le déficit des administrations publiques comme le déficit budgétaire de l'État diminue, ce dernier se situant comme cela a été dit à 3,4 pourcent du du PIB ces bons résultats ne doivent pas nous étonner les ministres s'appelle Eckerd nous ont habitués depuis le projet de loi de finances pour 2013 à tenir les engagements de la France,

en 2016 sur ce dernier chiffre, notons qu'il est exactement conforme au niveau recommandé par le Conseil de l'Union européenne du 10 mars 2015 dans le cadre de la procédure de déficit excessif, notons aussi que cette baisse constante des déficits s'est accompagnée d'un allégement des prélèvements obligatoires de 44,8 pourcent en en 2013

que cet objectif de contrôle de la dépense publique n'est donc pas l'apanage mais c'est les ministres de votre seul gouvernement. Dès lors, pourquoi avoir pris le risque d'ouvrir une bien mauvaise hé bien stérile polémique sur les comptes publics, suite à l'audit de la Cour des comptes, la Cour aurait identifié un risque d'exécution, compris entre 8 et 9 milliards d'euros sur un total de 322 milliards d'euros, ce risque a mis à nu est-il nouveau il étaient entre 6 et 10 milliards en 2012 et d'ailleurs les parlementaires que vous étiez, messieurs les ministres, à l'époque nous ce n'était pourtant guère ému, il était encore de 7 à 8 milliards en 2015, 2016, vous le savez bien, et vous l'avez dit, d'ailleurs les régulations de l'été servis chaque année à permettre d'atteindre les objectifs budgétaires et d'ailleurs, votre ami, monsieur Woerth, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, la réponse la redit et rappelé récemment en fait à l'issue de ce travail que tout gouvernement quel qu'il soit aurait réalisé notre déficit public sera comme la France est engagée, inférieur à 3

et d'ailleurs 2 fois, hein, c'est l'objectif que vous fixez pour les 5 prochaines années, vos prédécesseurs l'ont réalisé tout en permettant le final, le financement des politiques qui nous paraissait prioritaires, éducation, justice des forfaits sécurité notamment au fond de ce point de vue, celui de la baisse du déficit public, vous mettez vos pas dans ce qui vous ont précédés, vous le voyez, vous le voyez cher Éric Doligé, vous le voyez, cette petite polémique stérile, n'avait pas sa place dès l'instant où nous partageons avec vous cette la nécessité de poursuivre dans la restauration, des comptes publics je gage d'ailleurs que le rapport de la Cour des comptes, pourtant sur l'exécution de l'année 2 1000 18 premières exercice sous votre entière responsabilité sera bien moins commenté poursuivons maintenant notre réflexion sur le rapport préparatoire au débat d'orientation des finances publiques de façon générale, votre gouvernement propose de poursuivre des prélèvements obligatoires dans la voie de la baisse pardon des prélèvements obligatoires de la dépense publique du déficit du budget de l'État pour réduire in fine et le poids relatif de la dette, l'amélioration de la situation économique, fruit notamment des dispositions prises par vos prédécesseurs devrait vous y aider, je note d'ailleurs que l'estimation de croissance pour 2017 et de cinq 5, qualifié par le Haut Conseil des finances publiques fin 2016 d'optimiste devrait être atteintes voire dépassées si nous pouvons partager vos orientations dans leur principe, leur application rappelle cependant de nombreuses remarques sur l'effort de 13 milliards d'euros demandés aux collectivités territoriales, outre la coïncidence malheureuse entre cette annonce et l'affirmation un peu contradictoires de la volonté d'une négociation entre l'État et les collectivités territoriales, il n'est pas tant que durant les dernières 4 années, la baisse du déficit public et d'abord à mettre à l'actif des collectivités pour la seule année 2016 notre rapporteur général, chiffre à 3,1 milliards la contribution des appels à ce résultat, l'explication en est connue, nous l'avons régulièrement dénoncés dans la participation des collectivités est une perte sèche pour elle, la contribution de l'État n'est qu'une moindre augmentation des dépenses, comparé à l'évolution tendancielle c'est pourquoi avant de proposer de nouvelles coupes dans les services publics de proximité, commençons par établir la réalité des efforts certains par exemple, à compter de 2013 en appliquant, comme vous le proposez à l'avenir un calcul sur les dépenses en vous, nous trouverions alors sans difficulté les efforts non réalisés par l'État mais que vous nous demandez maintenant une 2ème fois aux collectivités non mais je note nous notons également que d'une part vous demande à l'ensemble des collectivités à nouvelle, fort de 13 milliards d'euros et que notre pas vous supprimez la taxe d'habitation pour 80 pourcent des des foyers français pour un montant évalué sur 3 ans à 9 milliards d'euros si la volonté de réduire la est intéressante, compte tenu d'acteur inégalitaire de cette taxe, vous proposez en réalité que le financement de cette décision sur par les économies générées par l'ensemble des collectivités territoriales sur cette mesure, enfin il me semble que pourrait encourir la censure du Conseil constitutionnel pour rupture d'égalité devant l'impôt, dès lors, ce ne serait plus de 9 milliards d'euros et 21,5 il faudrait trouver, il faut d'ores et déjà nous y préparer et penser dès aujourd'hui au remplacement de cette taxe par une part d'impôt national suffisamment dynamique comme la proposition avait été faite par le président de la République en ce qui concerne les prélèvements obligatoires, vous faites vôtre des mesures déjà décidées par l'ancien gouvernement, autant de 7 milliards d'euros, je n'y reviens pas, je reviendrai pas non plus sur les 3 1000 milliards d'euros nécessaires en 2018 pour engager engager la baisse de la TH par compte, comment pouvez-vous dans une situation de nos comptes publics, qualifié par vous-même proposer une transformation de l'ISF, il y a un coût budgétaire je comprends de 3 milliards d'euros en 2018 je refuse pour ma part de voir un quelconque lien de cause à effet entre la réintroduction tardive de cette mesure et l'augmentation parallèle, la contribution des collectivités de 10 après 7 milliards d'euros par ailleurs comment pouvez-vous affirmer dans le même temps que vous touchez pas vous impôts alors que l'augmentation des taxes sur le tabac comme sur le deviennent dizaines de Fribourg au final 2 5 milliards j'en reviens pas seuls, a été dit par certains collègues sur l'avis de nombreux économistes sur ceci : elle aurait un impact très significatif pour les ménages les plus riches correspondant au 10ème décide de l'impôt et donc et socialement pour les plus aisés, l'OSCE la pouvez voilà je j'emmène tout simplement sur la conclusion, si vous me permettez, tout ceci amène notre groupe à vous demander d'ici la présentation du PLF 2018 d'intégrer ces quelques remarques et de retravailler en profondeur votre trajectoire des finances publiques, vous nous avez d'ailleurs montré très récemment que vous étiez capable de très grande agilité pour intégrer en catastrophe quelques milliards de dépenses nouvelles, pour conclure, le groupe socialiste républicain votera la loi de règlement et vous souhaite Monsieur Monsieur le Ministre, un été studieux pour revenir à la rentrée devant nous avec une trajectoire des finances publiques plus affiner et peut-être plus convaincante. Merci mon cher collègue, la parole est à monsieur David de Rachline pour le groupe de non-inscrits et moins chers collègues, vous avez la parole pour 3 minutes. Merci madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, je vais pas m'étaler en ce qui me concerne, sur les comptes 2016 : vous connaissez tous, si c'est notre position sur les orientations budgétaires et vous connaissez tout autant notre nous se mettre à l'austérité imposée par Bruxelles, mais rappelez-vous : bien que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est du fait des politiques menées depuis des décennies que les choses soient très claires, tous les gouvernements dans cette affaire portent une lourde responsabilité, je l'ai dit ici avant hier, mais je considère que pourcent imposés imposés par l'UE passe après la sécurité des Français, c'est l'objet de mon propos ici et qu'est-ce qui peut stopper les attaques contre notre pays, pourcent ou ou un équipement correcte de nos forces de sécurité, croyez-vous que les familles des morts du Bataclan Denis et celle des soldats morts pour la France en ont quelque chose à faire de la règle des 3 or oui, le fait de diminuer le budget du ministère de l'Intérieur diminutions entraînant par exemple la fin des recours au réserviste au sein des forces de police comme ces cas, dans le Var et même dans ma ville, alors que la saison touristique bat son plein, le fait de diminuer le budget de la défense, alors nos soldats luttent contre nos ennemis dans des matériels hors d'âge, les vagues d'ailleurs dans lesquelles nos soldats font la guerre au Sahel en moyenne plus de 31 ans, je n'ose pas vous demander la moyenne de 2 voitures fonction alors oui, le fait de diminuer ses Budgets remet en cause la sécurité des Français au-delà des chiffres, cette actualité budgétaire est très inquiétante sur le fonctionnement de notre République et sur la dérive autoritaire que nous voyons poindre l'article 24 de la Constitution de la Ve République, dispose que le Parlement vote la loi, le contrôle l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques quant à l'article 45, il précise : le Parlement vote le projet de loi de finances, or pour voter la loi pour contrôler l'action du gouvernement et pour évaluer les politiques publiques, les parlementaires ont besoin de recevoir des informations et d'interroger ce qui sur le terrain même ces politiques publiques obéissent au gouvernement et utilise l'argent public pour nos institutions fonctionnent correctement, il est indispensable et normal et je dirais même il est 5 les personnes notamment Les Hauts fonctionnaires qui s'exprime devant les commissions parlementaires puissent le faire en toute franchise et en cas de sujets sensibles, c'est bien évidemment le cas des affaires de défense les auditions se font à huis clos et n'ont donc pas vocation à être rendus publics ces personnes entendues par les commissions ne sont là que pour répéter les éléments de langage préparé par leur autorité de tutelle ou pour sur ordre caché la vérité, voire mentir alors plus besoin de perde son temps à les auditionner mais alors on change la Constitution car c'est pour contrôler l'action du gouvernement vous avec la parole du ministre-cela va pas être facile évidemment et si le pouvoir législatif n'équilibre plus pouvoir exécutif on change alors de régime et on quitte le système démocratique, le Sénat a récemment obtenu la condamnation d'un homme pour avoir menti devant une commission d'enquête, c'est bien la preuve que nos institutions ne fonctionnent que si la parole est libre, vrai et sincère devant le Parlement, qui je le rappelle, représente le peuple souverain alors je conclurai par les mots de George Orwell dans les temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire et je suis sûr que le Vendéen Pierre Deville qui a servi la France pendant 43 années avec honneur et fidélité sera ému d'être passé du côté des révolutionnaires. Merci, moi j'ai collecté par l'État Monsieur Vincent Delahaye pour le groupe Union centriste et mon cher collègue, vous avez la parole pour 12 minutes maximum.

Madame la présidente, messieurs les Ministres Monsieur monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs, sénatrices et sénateurs tout d'abord le passé, la loi de règlement, c'est vrai que j'aurais préféré qu'on puisse en débattre avec d'autres ministres assez bon avant la présidentielle, ça m'aurait semblé tout à fait normal de pouvoir faire le bilan d'un quinquennat avant la présidentielle, et je pense que dans le changement de pratique qui est souhaitée par le président de la République, il faudra y réfléchir parce que c'est pas normal qu'on arrive en fin de quinquennat et qu'on étudie finalement les comptes 2016 le 20 juillet avec de nouveaux ministres qui sont non pas la responsabilité de ce qui s'est passé alors sur la loi de règlement, monsieur Claude Raynal qui la trouvent très très bien qui va la voter, nous n'allons pas la voter, nous n'allons pas la voter, d'abord parce que nous n'avons pas voté la loi de finances initiale pour moi, c'était un des éléments, mais de 2ème élément, c'est que pour nous. Ces comptes ne sont pas sincères, ces comptes ne sont pas sincères, la Cour des comptes l'a relevé, puisque on a 12 vers 5 milliards de reports de charges de 2016 sur 2017 et 12,5 milliards sur un déficit monsieur rénale qui est supérieur au déficit de 73 ans, retraité, parce que si on retire les éléments exceptionnels de 73 2013, 2016, le déficit est supérieur, les 76 milliards et si vous prenez 12,5 milliards sur 76 milliards c'est 16 pourcent du du résultat qui n'est pas bon

l'augmentation considérable des frais de personnel de l'année 2016, 2016, c'est l'équivalent des 5 des 5 années précédentes en terme d'augmentation de Damas salariale plus l'endettement, quitte à son maximum 2200 milliards, c'est-à-dire 7 années et demie de recettes fiscales, il faut quand même chose mesurer ces 7 années et demie d'impôts de TVA, de l'impôt sur les sociétés d'impôt sur le revenu, donc tout ça c'est, c'est la loi de règlement, malheureusement, elle montre une situation extrêmement dégradée de nos finances publiques qui n'est pas une découverte pour nous a ici au Sénat au sénat on a refusé de d'examiner la loi de finances initiale 2017 je pense avec raison et avec sagesse toujours la sagesse qui mène aux travaux ici au Sénat, et c'est vrai que on a pensé que cette loi de finances, à juste raison était insincère et on a bien fait de pas l'examiner et moi je considère que ses comptes annuels de 2016 sont eux insincère sincère et dans aucune entreprise privée, on aurait un report de charges accepté de cette dimension-là, donc c'est vrai que c'est un mauvais cadeau pour le nouveau gouvernement. Je nuance serait un petit peu les positions qui ont été affirmé tout à l'heure en disant que c'est une situation qu'on découvre. Vous étiez député, Monsieur le Ministre, nous sommes sénateur et cette situation, on ne la découvre pas si vous reprenez mon intervention sur la loi de finances initiale à l'Automne dernier, ce qu'a dit la Cour des comptes, il y a quelque temps, là je l'avais déjà annoncés, c'est d'ailleurs qui manquait 11 à 12 milliards dans les dans les dépenses de l'État et c'est pas une découverte, c'est quelque chose que nous savions mais c'est vrai que ça plombe forcément les années 2017, 2018 et comme nous sommes là à la fois pour la loi de règlement sur le passé, mais surtout pour réfléchir à l'avenir, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble. Il est évident qu'il faut un affaiblissement de nos comptes publics, alors messieurs les ministres, vous nous présentez une trajectoire ambitieuse. C'était déjà le cas il y a 5 enfants soit Hollande quand il est arrivé, nous a présenté une trajectoire très ambitieuse puisque, en 5 ans, il devait revenir à l'équilibre, on a vu ce qui est advenu. On est très très loin de l'équilibre à la fin 2016, moi j'ai peur, j'ai peur que vous fixez un objectif trop ambitieux, je vous le dis, moi, je pense qu'il faut se donner plutôt 8 ans pour revenir à l'équilibre des finances publiques que 5 5 ans 5 ans ça me paraît trop court, compte tenu de la distance qu'il y à parcourir pour revenir à cet équilibre des finances publiques qui était souhaitable pour notre pays, donc ça c'est la première remarque la 2ème remarque, c'est que je pense qu'il faut arrêter quand même d'être trop optimiste et que quand on fait un budget, il faut être prudent

Si on regarde les 10 dernières années, messieurs les Ministres, les 10 dernières années, la croissance moyenne en France, c'était combien. Personne n'a la réponse dans l'hémicycle 0 9 sur les 10 dernières années, c'est 0 9 pourcent donc donc on peut pas dire que 1,6 avec sur 5 ans, ça soit quelque chose qui ne soit pas qu'ils soient prudents, donc moi j'avais déjà fait cette proposition auparavant à vos prédécesseurs, ils ne l'ont pas suivi, mais j'aimerais bien que. ça, soit peut-être une position de principe qui soit retenue, c'est-à-dire que on prennent comme hypothèse de croissance, le consensus des économistes : moins 0 5 pourcent.. Et j'avais proposé qu'on fasse ça de façon à ce qu'on est plutôt des bonnes surprises et moi j'aime bien les Budgets, avoir des bonnes surprises, plutôt que de mauvaises, donc moi je dis, je dis qu'aujourd'hui je pense que vous êtes un peu optimiste avec l'an dernier, si ça virgule 7 pourcent et et que il serait souhaitable de partir sur des hypothèses plus basse. Ensuite, il est nécessaire effectivement de faire des économies et de faire de vrais économique

c'est-à-dire que les dépenses augmentent quand même, je sais bien que ça n'a jamais été fait, je sais bien que ça n'a jamais été fait, j'ai entendu ça, ceci étant, moi je suis pour une véritable baisse qui nécessitent des réformes de structure et j'attends ces réformes de structures parce qu'on nous les a annoncé c'est dans vos documents et j'espère que d'ici à la fin de l'année, on y verra plus clair sur ces réformes de structure, parce que pour moi, ils sont indispensables, donc moi je souhaite une vraie baisse de la dépense publique et sur les économies que vous annoncez, vous annoncez 82 milliards vous annoncez 20 milliards en 2018 et vous annoncez 80 2 milliards sur la durée, le président de la République avait annoncé 60 milliards 10 milliards pour les collectivités, là, on est passé à 82 milliards pourquoi pas. Et on est passé de 10 à 13 milliards pour les collectivités, alors moi j'aimerais vous entendre dire quelle va être la répartition des 82 milliards parce que c'est important, il faut savoir quand même que le déficit de l'État, c'est 95 98 pourcent du du déficit de l'ensemble les collectivités locales étaient en excédent de 3 milliards à la fin 2016 donc ça veut dire quand même que en part de déficit, c'est quand même les dépenses de l'État qui marque le plus Au-delà même de 50 pourcent vous vous avez indiqué tout à l'heure, moi j'aimerais avoir la répartition complète des 82 milliards et j'aimerais surtout parce que c'est ce qui nous a beaucoup gênés dans le quinquennat précédent et j'aimerais pas qu'on recommence sur cette base là, c'est que le calcul des économies pour les collectivités locales et pour l'État, soit le même voilà si on dit que l'État à 0 pourcent en en volume fait des économies, à ce moment-là on dit pour les collectivités locales, c'est la même chose, c'est-à-dire que, à 0 pourcent en en volume pour les collectivités, on fait aussi des économies et on est dans le discours du président de la République, qui souhaite un discours de confiance réciproque et donc la confiance à ce n'est pas que ces combats ce partie sur les mêmes bases, et pour moi c'est très important parce que on est en début de quinquennat et si on veut pouvoir travailler ensemble, et moi je souhaite que le Sénat travaille avec le gouvernement et aide à redresser la situation et qu'on fasse des propositions, je pense qu'il faut être sur les mêmes bases Je parle en mon nom, bien sûr, mais je parle au nom de du groupe de l'Union centriste et je voudrais dire que le groupe d'union centriste a envie de vous faire confiance, messieurs les ministres et envie de faire confiance au gouvernement, mais le crédit qu'on peut vous accorder ne sera pas éternelle et que pour que ce crédit dure dans le temps et que cette confiance se maintiennent, il faut absolument qu'on ait un discours commun et ce que je viens de dire à la fois sur la prudence et sur le calcul des économies, je pense qu'il faut que ça soit précisé en début de de mandature et qu'on puisse vérifier sur la suite Par rapport à tout cela, je dirais que la loi de finances 2018 va être forcément une épreuve de vérité, j'espère que ça va être une opération vérité j'ai entendu dire qu'il aurait pu, de sous-budgétisation donc ça, ça va être le 1er marqueur effectivement s'apercevoir que le budget est sincère et que l'on a pris en compte toutes les dépenses qu'on peut connaître lorsqu'on prépare le budget, c'est-à-dire en septembre, octobre, toutes les dépenses à me dire qu'on peut connaître connaissez pas de sous-budgétisation mais je souhaiterais également que vous engagiez sur les réserves, la réserve de précaution parce que j'entends les ministres Sapin les ex-ministre Sapin Eckerd qui nous disent : oui, vous avez 11 milliards de nouvelles dépenses mais en avait 13 milliards de réserve de précaution. Mais pour moi la vraie réserve de précaution, c'est celle qu'on peut vraiment gelé, quand on voit que dans la réserve de précaution, on a des dépenses qui sont des dépenses de de rémunération de pensions et autres, on sait très bien qu'on va devoir y faire face, donc c'est pas une vraie réserve de précaution, donc moi j'aimerais avoir une vraie réserve de précaution et avoir une provision pour dépenses imprévues, ça peut être pour les obsèques, ça peut être pour eux chose mais qu'on est clairement une provision pour dépenses imprévues, on sait que c'est une réserve, mais là on du coup on est, on est vraiment dans dans le dans quelque ne permettent pas d'y voir clair et moi j'aime bien y voir clair, j'aime bien la transparence, j'aime bien la clarté, j'aime bien l'honnêteté et dans les comptes publics, ça me paraît quelque chose de très important donc. De la prudence. Des objectifs peut-être un petit peu moins ambitieux mais qu'on peut étaler un petit peu plus dans le temps mais contiendra parce que moi ce qui me paraît important, c'est tout dire ces objectifs et le 3ème point. Le la loi de finances 2018 soit une vraie loi de vérité et de clarté. Alors pour aller un tout petit peu plus loin sur cette loi de finances, j'ai entendu le discours du président de la République cet après-midi qui a dit que le seul budget qui augmenterait, ça serait le budget de la défense.

j'ai entendu, madame la présidente, je sais que vous êtes très rigoureux sur les horaires et moi aussi, donc elle a raison, elle a raison, mais moi j'aime bien aussi la rigueur, je pense que dans les comptes publics, c'est important aussi d'avoir la rigueur donc dans les priorités, moi, je serai très vigilant à ce qu'il n'y a pas une dizaine de priorité dans le passé, on a vu ça très régulièrement sur des Budgets, on a vu dès 10 priorités et quand on a des priorités, on en a plus une seule, donc moi j'entends votre priorité à la défense, j'espère qu'elle sera respectée et j'espère surtout que, on verra qu'il y a 2 ou 3 priorités : voilà pour conclure, je dirais qu'on a envie de vous faire confiance, on espère que vous allez agir vite, fort, que vous allez agir avec courage et discernement, messieurs les Ministres et que vous le serez aussi dans la transparence et dans l'honnêteté vis-à-vis des parlementaires que nous sommes, je vous remercie. La parole est à présent à notre collègue Philippe Dallier pour les républicains et vous aurez moins chers collègues 14 minutes maximum. Madame

le président de la République avait annoncé pendant la campagne électorale, vouloir demander un audit des finances publiques dans la foulée de cette élection, cet auditeur, nous l'avons alors démarche classique, diront certains, tout nouvel élu quel que soit le poste, cherchant toujours à charger la barque de son prédécesseur, c'est ce que n'ont pas manqué d'dire Michel Sapin et Christian Eckert, qui nous manque aujourd'hui, je dois vous le dire mais que Claude rénal a essayer de remplacer en nous servant les mêmes arguments, mais pour nous comme pour tous ceux qui s'intéressent un peu aux finances publiques, il y avait besoin de cet audit, parce qu'il y avait nous savions et nous savions tous et je suis persuadé qu'à Bercy, il ne savait il y avait des cadavres dans le placard.

comportait des éléments d'insincérité connu connu, elle le dit la Cour qui rendait absolument inatteignables, l'objectif affiché de 2 8 pourcent alors alors je ne vais pas trop insister sur les résultats de l'année 2016 puisqu'il s'agit du bilan de vos prédécesseurs, monsieur le ministre, mais tout de même en 2016, la croissance de l'économie française a été médiocre 1,2 pourcent c'est c'est à peine mieux qu'en 2015, 1,1 pourcent et et surtout et surtout, c'est très loin de ce que les autres pays européens ont fait 1,8 en Allemagne et dans la plupart des pays européens, alors pourquoi ce décalage, c'est bien là la question que nous devrions nous poser est pourquoi la France est-elle à la traîne depuis maintenant un certain nombre d'années elle a décroché la France et c'est bien cela qui devrait nous inquiéter et pour nous, c'est la conséquence directe des politiques qui ont été conduites depuis 2012 parce que nous n'avons pas fait les réformes structurelles nécessaires, notamment sur le marché du travail. De même, le déficit public c'est très faiblement réduit l'an dernier, il est passé de 3,6 pourcent du du PIB à 3,4 pourcent et et cette amélioration peu significative doit en outre être relativisée, d'une part, il n'est pas inutile de rappeler que, en 2012 à peu près à la mais l'époque le gouvernement qui ne s'installer nous annonçait le retour à l'équilibre des comptes publics pour 2016 voilà, retour à l'équilibre, on est à 3,4 et d'autre part cette lente amélioration est essentiellement due à des facteurs autres que la bonne maîtrise des dépenses de l'État, elle est principalement dû ça été rappelé à une charge de la dette inférieure de 3 milliards d'euros à celle observée en 2015, du fait d'une nouvelle diminution des taux d'intérêt, tant mieux, tant mieux, mais c'est tout-à-fait conjoncturelle et cela aura une fin, elle est due également pour moitié à l'amélioration des comptes des collectivités territoriales qui par leurs efforts ont dégagé un excédent de 3 milliards d'euros en 2016, malgré ou à cause de la réduction des donations de l'État, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais cela, il faut le rappeler cache aussi une réalité qui finira par nous rattraper, c'est d'abord l'investissement public des collectivités locales qui baissent et que lorsque nous obtiendrons, nous aurons tiré sur l'entretien des bâtiments et de la voirie, on sait bien que tout cela se paiera un jour, alors j'appelle d'ailleurs votre attention, Monsieur le Ministre, alors que vous voulez imposer 13 milliards d'économie aux collectivités locales, après les 11 milliards de baisse des dotations de l'État du quinquennat précédent sur le fait que ces dernières ont déjà fait des efforts de gestion important et je suis heureux, Monsieur le Ministre, que vous l'ayez noté parce que c'est vrai que dans le climat actuel est depuis une dizaine de jours, on aurait l'impression en écoutant les journalistes que les collectivités locales sont responsables de tous les malheurs budgétaire de ce pays, c'est loin d'être le cas et il est quand même bon que ça soit rappelé et un exemple, la progression de la masse salariale des collectivités territoriales,

alors oui, nos collectivités ont pris déjà une part importante dans la réduction du déficit public et il est bon de le rappeler, quant au budget de l'État, le déficit mais a été réduit que de 1,5 1000000000 d'euros en 2016 à 69,1 milliards et encore la Cour des comptes, le dit, c'est au prix d'accommodements critiquable avec la comptabilité budgétaire, vous avez en effet augmenter l'aéroport de 900 millions d'euros par rapport à 2015, ce qui n'est pas rien et la Cour pointe aussi la sortie du périmètre du budget de l'État d'1,9 milliards d'euros de dépenses, donc ça ce sont des petits habillages qui permettent d'améliorer la situation, mais qui ne sont pas la vérité des chiffres, et la Cour des comptes, et c'est peut-être le plus le plus grave, note hors éléments exceptionnels et investissements d'avenir, en fait, depuis 2013, le déficit ne s'est pas réduite rien depuis 2013, alors mon cher collègue rénale, on a du mal à se laisser convaincre par vos arguments, ben, c'est dommage, mais effectivement préfère effectivement la Cour des comptes, ça nous semble un tout petit peu plus comment dire à la loupe à être sérieux. Mais je pense que c'est la la critique la plus sévère, qui est portée contre la majorité précédente, de surcroît, le déficit public de la France demeure en 2016 très supérieur à celui de la moyenne européenne et de la zone Euro 1,7 et 1,5 pourcent et la France et d'ailleurs avec l'Espagne, le seul pays qui reste maintenue dans la procédure de déficit excessif. Rappelons également que notre tour dépense publique atteint 56,4 pourcent de de la richesse nationale et que nous détenons la le record d'Europe

les dernières années du quinquennat Hollande devait être celle de la baisse de la fiscalité, alors c'est vrai qu'il y a eu une baisse de l'impôt sur le revenu pour les ménages les plus modestes et des allégements pour les entreprises, mais aucune balle là au global, la fiscalité n'a pas diminuer les prélèvements obligatoires n'ont pas diminué, enfin, la dette publique, elle a atteint 2147 milliards d'euros, elle passe de 95,6 pourcent du du PIB en 2015 à 96,3 se rapprochant inexorablement de 100 pourcent de de la richesse nationale et, là aussi sans l'artifice primes d'émission, le gouvernement a largement utilisé en 2015 comme en 2016, alors là, on peut effectivement mais utiliser ces primes d'émission c'est facialement diminuer la dette aujourd'hui mais c'est reporté le coup sur les années à venir, moi vous savez en politique, mon maître, ce général De Gaulle, et il disait : il ne faut jamais sacrifier le long terme au court terme. tous ces résultats et je reviens à la dette sont d'autant plus inquiétant que les taux l'intérêt central remonter les OAT à 10 ans retrouvé son Andral remonter en 2016, vous avez eu un trou exceptionnel, ils ont retrouvé leur niveau de 2015 et chacun sait que c'est Olympe RFI n'iront pas remonter et nous sommes heureux de constater que le gouvernement a dans ses prévisions, anticiper cette remontée des taux à un niveau important mais cela ne fait pas disparaître pour autant le risque et ce risque, il pèse effectivement sur le budget et dans les bacs dans des proportions importantes. Alors nous détenons plusieurs records en Europe, médaille d'or de la dépense publique, médaille d'argent du déficit public et nous sommes sur le podium pour notre niveau de prélèvements obligatoires, notre déficit budgétaire et le dos de la moyenne de nos voisins, sans parler de l'Allemagne, je sais que ça énerve toujours quand on parle de l'Allemagne mettait, elle est en excédent budgétaire depuis 2014, la comparaison sur le déficit structurel est tout aussi désavantageuse pour nous l'avait publique française a augmenté de 0 7 points en 2016 alors que la dette a diminué en moyenne de 1,4 points dans l'Union européenne et 1,1 point dans la zone Euro, la divergence avec l'Allemagne et presque de 30 points le rapporteur général a rappelé contre 10 points en 2012, c'est-à-dire que l'écart s'est très largement creusé et je rappelle que la dette allemande était pourtant légèrement supérieure à celle de la France avant la crise économique, la divergence avec l'Union européenne et de 13 points le décrochage s'est bien opéré en 2012 et la divergence avec la zone Euro et de 7, le décrochage est apparue en 2014. La Cour des comptes et donc parfaitement fondé à affirmer que la situation de nos finances publiques est médiocre et je trouve que le terme de médiocre et 30 corps trop faible, je crois que on peut utiliser le terme de situation alarmante, ça me semble tout à fait convenir ce qu'on s'en est pourtant pas nouveau, nous l'avions déjà dressé en novembre dernier à l'occasion de la discussion budgétaire, nous avions organisé une conférence de presse avec nos collègues de l'idée, un groupe centriste à l'époque et certains journalistes apparaissait alors quelque peu incrédule, pourquoi pas dire narquois dubitatif, nous avions pourtant pointée du doigt à l'époque, les mêmes éléments d'insincérité que la Cour des comptes, aujourd'hui ce qui nous avaient conduits à adopter une posture que vous aviez condamné sur les bancs du Parti socialiste, nous avions choisi la question préalable, après une longue discussion générale qui avait entraîné le rejet du budget que n'avions-nous entendu alors pour certains au Parti socialiste pour qui sont passés chez en marche aujourd'hui, hé bien, 7 mois plus tard, la Cour des comptes reprend exactement nos critiques et notre rapporteur général a rappelé notre hypothèse de 3,2 pourcent du du déficit en 2017 à la police a été effectivement validée par la cour, alors nous reconnaissons bien volontiers que notre seul tort fut d'avoir eu raison trop tôt, alors le gouvernement enfin aujourd'hui couvrir la situation mais quand même, messieurs les ministres, nous trouvons que la ficelle est un peu grosse à l'époque d'ailleurs pas inutile de rappeler qu'Emmanuel Macron a été à Bercy jusqu'à l'été 2016, donc sur les comptes 2016 il y a quand même constat de la situation et quand on sait comment comme fonctionne la mécanique de merci à La Hague, en août 2016, le budget 2017 était bouclé chacun, ça va, et je crois que la commission des finances, a récupéré quelques documents qui montrent que des notes du Trésor alertait en disant attention en 2017, ça va être beaucoup plus difficile que ce que vous affichez tout le monde savait, chers collègues, tout le monde savait seulement on n'a pas voulu dire à l'Assemblée nationale nationale était pas député mais Bruno Le Maire était député Gilles Carrez avait également alerté comme nous ici et je pense que personne ne mettait en doute la qualité de l'analyse de J. K. alors la découverte du mauvais état des comptes publics s'apparente un peu à une mise en scène qui permet de revenir sur certaines annonces de campagne tout ce qui est dans le rapport de la Cour des comptes étaient connu mais voyez au moi j'ai un point d'accord avec Claude rénal c'est sur la mise en scène, c'est dommage que ça s'arrête là. La Cour des comptes avait recommandé en cas dérapage des comptes de soumettre au Parlement un projet de loi de finances rectificative malgré l'état des finances publiques que vous semblez des ou vous de vous semblez découvrir vous mes chers collègues, que j'ai pas bien compris la réponse que le 1er ministre ma fête lors du débat sur la politique générale il manie, on ne fait pas de loi de finances rectificative parce qu'on aurait été dans l'obligation d'augmenter les impôts, alors sur le coup, j'étais un peu surpris, je me suis mais qu'est, est-ce que c'est que cette réponse donc on a fait vérifier si quelqu'un peut me démontrer que la LOLF impose que dans une loi de finances rectificative, on augmente les impôts, on a on a juste les dépenses et les recettes en fonction de la nouvelle situation ça permet effectivement d'avoir un débat au Parlement, alors qu'avec vos décrets avance mais effectivement le débat est très limité, eu dans en commission des finances, on en discute un peu, on vote pour votre compte, mais ça ne permet pas au Parlement, effectivement comme dans une mode finance rectificative de modifier les chiffres et de faire bouger, de faire alors vous procéder par décret d'avance pour 3,3 milliards d'annulations de crédits et ses annulations touchent notamment la défense avec les conséquences que l'on sait, et c'est vrai que c'est assez regrettable mais aussi la justice, la sécurité et l'enseignement supérieur et la recherche, les collectivités territoriales, ça a été rappelé par peu de monde ou supprimer 209 millions d'euros de crédits pour le fonds de soutien à l'investissement local et pour les contrats de développement ruraux, bon 209 millions et la justification dans le document de Bercy, c'est-à-dire pas la phrase est tellement tourner qu'on a impression qu'il y avait pas dossier les collectivités locales, j'en doute, je pense qu'il y avait des dossiers mais vous réduisez effectivement cette subvention à nos collectivités territoriales, par les temps qui courent, c'est malvenu, je vois que le temps passe, alors je vais peut-être accélérer avant que madame la présidente, non le fasse remarquer, alors oui, vous avez profité de cette mise en scène sur la découverte de l'État, nos comptes publics pour changer votre fusil d'épaule en matière de politique économique et budgétaire et c'est un peu regrettable en 2012, François Hollande a fait une grave erreur, il a cru que la croissance allait revenir toute seule, il a matraqué fiscalement les particuliers, entreprises, il a tué la croissance, il y avait au moins un point sur lequel je pense que nous étions d'accord pendant la campagne électorale, il fallait un choc de compétitivité tout de suite mais ce choc de compétitivité vous décalé si voulez si voulez décalé dans le temps de ce ministre, effectivement il fallait redonner à la fois aux particuliers valse-hésitation sur la taxe d'imitation valse-hésitation sur l'ISF et du coup vous avez décaler certaines mesures de compétitivité, j'espère, et c'est aussi que je forme en terminant que ce n'est pas là une grave erreur que vous paierez plus cher, trop tard, la croissance semble être en train de repartir, il faut vraiment saisir l'occasion pour relancer la mécanique, peut-être que c'est ce que vous ne faites pas assez, j'espère que nous n'opérons pas vous. Mon cher collègue, je crois que messieurs les ministres veulent une petite suspension de séance, donc je vais suspendre la séance, nous la reprenons voulez combien de temps Monsieur 5 minutes nous reprenons : moins 25, si vous le voulez bien donc la séance est suspendue.

La séance est reprise pour répondre à la question de certains de mes collègues, il n'y a pas de séance ce soir donc, nous vous allons terminer ce débat c'est aujourd'hui cet après-midi, si je puis dire, donc si on doit déborder on débordera ça ne tient qu'à vous. J'ai répondu à votre votre question, c'est parfait, monsieur Rénald vous n'aviez pas posé la question mais vous l'avez pensé tellement fort que j'avais entendu donc la parole est à Monsieur François Marc, pour 7 minutes au nom du groupe socialiste et républicain. Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous avons écouté avec grande attention l'intervention de Claude rénal et elle a été saluée sur tous les bancs, donc je vais me contenter de quelques précisions additionnelles à son propos, le contexte, on le connaît le cadrage nous a été présenté le contexte de déficit d'endettement et à la nécessité d'efforts budgétaires, tout le monde, je pense, en convient, mais l'élaboration d'une stratégie gouvernementale ne peut pour autant ignorer la situation inquiétante tenantes à l'accroissement des dîners galite et en France. Nos gouvernants évoque régulièrement et à juste raison, les principes républicains de liberté, de fraternité, on a entendu à Versailles. Ils doivent aussi porter une attention soutenue au principe d'égalité, il ne pourra y avoir aucune vraie mobilisation collective du pays si la recherche d'une plus grande égalité n'est pas au coeur des préoccupations des autorités publiques. Quel constat peut-on faire en 2017, au sujet des inégalités en France, hé bien, selon l'Observatoire des inégalités, les écarts de revenus entre les plus pauvres et les plus riches continuent d'augmenter selon l'INSEE, je cite, la pauvreté et les inégalités ont encore progressé, même si en 2015, plusieurs mesures fiscales, baisses d'impôts pour les faibles revenus, modulation des allocations familiales ont permis d'atténuer en partie s'agit égalité, Le contexte général étant l'jugé très inquiétant, il y a 10 ans, le capitalisme perdait pied et toutes les analyses ont pointé l'accroissement des inégalités de revenus comme l'une des causes majeures de cette catastrophe financière. Et la situation créée dangereux à 2 titres : tout d'abord, elle creuse le lit du populisme qui se nourrit du ressentiment économique pour rejeter en bloc les études, les économiques et intellectuelles, mais aussi les étrangers et les minorités en général par ailleurs à l'bloque la croissance économique en empêchant une partie de plus en plus important de la classe moyenne d'accéder à plus de consommation, il y a une éducation de qualité, il ne pourra donc il y avoir, à mes yeux de prospérité durable sans réduction des inégalités. S'agissant du débat d'orientation budgétaire de ce début de quinquennat il doit bien sûr et de l'occasion d'évoquer les principes d'action essentielle à partir des seront déclinés les mesures financières et fiscales de la programmation à venir et je souhaite pour ma part exprimé ici une triple conviction. Oui, la réduction du déficit budgétaire est une impérieuse nécessité. Oui, les mesures budgétaires et fiscales doivent en particulier visait à lutter contre les inégalités dans notre pays. Oui, l'assainissement de nos finances publiques doit veiller à préserver l'esprit de la décentralisation dans notre pays. S'agissant tout d'abord de la trajectoire du déficit. Rappelons que celui-ci, qui s'élevait à 50 milliards en 2007. à grimper à 148,8 milliards en 2010, soit 7,7 pourcent du du PIB, on a entendu tout à l'heure, quelques interventions sur la vertu budgétaire nécessaire je souligne que le déficit qui était de 148 milliards en 2010 est passé à 75 milliards en 2016 soit une division par 2, n'est pas négligeable. S'agissant de la programmation pluriannuelle des finances publiques adoptée sous l'ancienne majorité, elle prévoyait, quant à elle un retour sous la barre des 3

messieurs les Ministres, j'ai noté que les intentions annoncées par le gouvernement s'accordent peu ou prou avec ses projections et nous sommes non nous convenons donc il convient de poursuivre dans la trajectoire annoncée. Deuxièmement, la politique budgétaire et fiscale doit contribuer à la réduction des inégalités, jeudi. Le président de la République l'a rappelé à Versailles ne peut y avoir de développement équilibré de la France et chacun ne trouve pas sa juste place dans la société. Tendre vers plus d'égalité entre les Français doit me semble-t-il, constitué un fil conducteur de la politique budgétaire à conduire dans les prochaines années. Et n'oublions pas que c'est le début du quinquennat qui donne toujours le signal politique majeur qui ne se souvient en la matière du début calamiteux du quinquennat Sarkozy en 2010 en 2007, le fameux paquet fiscal, dotée d'un bouclier renforcé avait conduit à distribuer de l'argent aux plus riches, et le gouvernement du se résoudre à une piteuse marche-arrière avant la fin des 5 ans du quinquennat. Je vous propose, je vous posais ici la question messieurs les Ministres, est-il vraiment si est impératif, alors que la France a encore un déficit budgétaire annuel de 70 milliards d'euros de réduire aujourd'hui SF de 3 milliards. De réduire la fiscalité de l'épargne des plus fortunés avec la flat axe de 30 pourcent est est-ce vraiment le moment d'adopter une stratégie identique à celle que nous avons mieux mettre en oeuvre en 2007, Ma 3ème conviction qu'il faut conforter la décentralisation en réservant collectivités territoriales des moyens suffisants et équitablement répartis 2 chantiers ont été engagés durant le quinquennat précédent, celui d'un nouveau mode de répartition de la DGF, d'une part, et celui de l'indispensable révision des valeurs locatives, d'autre part, quels sont aujourd'hui les intentions du gouvernement pour aboutir à une DGF plus équitable en entre communes et intercommunalités, c'est une question et s'agissant des valeurs locatives foncières, une première étape a été franchie avec la mise en application de la révision des valeurs des locaux commerciaux dès cet Automne et quant à la 2ème étape, elle est également engagée avec les principes qui ont été adoptées, l'expérimentation grandeur nature qui a été menée, et là aussi, la question est posée au gouvernement, y a-t-il une véritable volonté politique de mettre en oeuvre cette révision des valeurs locatives d'habitations, c'est je crois une question fondamentale : si on veut en vers plus d'équité et une véritable justice fiscale entre contribuables locaux, je vous remercie. Merci mon cher collègue, la parole est à monsieur Serge Dassault pour les républicains, mais mon cher collègue, je vais vous donner bien volontiers la parole pour 7 minutes maximum.

le président président ont privilégié l'État-providence, multipliant les dépenses de protection sociale sans prévoir leur financement, ils oublient le risque grandissant de l'ensemble du système financier j'aussi effondrée connaîtront tirer augmenteront

tout système social que caution aujourd'hui s'écroulerait, la France ne peut se résoudre à faire faillite, le gouvernement doit pas des clients qui risquent de méfiance, de nous investisseurs

économise encore flou, alors l'annonce de dépenses nouvelles et la suppression de recettes non financées, se multiplient 450 millions supplémentaires pour les contrats aidés qui coûte déjà 2 milliards 5 par an, à quoi ça sert et et c'est pas ça qui va réduire le chômage, de même la prime d'activité 4 milliards si vous souhaitez doublé, c'est de la folie, ça ne sert à rien et c'est pas ça qui vont faciliter l'embauche silicieux financé par 15 milliards d'emprunts,

l'affaire aussi l'Allemagne pour baisser le coût du travail en réduisant le périmètre de l'État-providence, ça suffit, l'État-providence, par exemple en développant le système par capitulation Lazic social et non par répartition, invitant les salariés à prendre les assurances personnelles pour financer leur retraite la santé Jean-Marc, c'est comme ça dans tous les pays, et ça ne coûte rien à et ça marche très bien, on pourrait réduire ainsi d'autant les charges sur salaires et baisser le coût, il travaille l'apprentissage aussi efficace pour faire avec le collège unique que nous subissons en France depuis 15 ans, ça ça me suis habitué à enseigner le même programme à tous les enfants sans aucune formation professionnelle produit en réalité 150000 chômeurs par an, tout le monde en fait

et pas des départements et les dépenses de à ça, à tous ces dépenses, ce qui fait qu'aujourd'hui les pardon en faillite et il faut quand même arriver à réduire ça monsieur, c'est maire et les présidents départementaux sont très inquiets sur leur gestion,

écoutez, taux d'imposition progressif sur le revenu, supprime toute possibilité d'enrichissement pour les contribuables parce que plus ils sont

et pour cette doivent rassurer la décret lui-même qui le désirent, droit de gauche mais pour tous et ne sera jamais assez remercier d'avoir mis en place un gouvernement d'union nationale et le supprimer, il y a 16 merci. Il vaut cher collègue, la parole est à monsieur Jean-François Husson pour le groupe, les républicains qui j'vais demandé de bien vouloir respecter son temps de parole.

madame la présidente, monsieur le Ministre Monsieur messieurs les les rapporteurs généraux, le rapporteur général, mais mes collègues Philippe Dallier, à l'instant, Serge Dassault, l'ont rappelé la situation budgétaire de la France est très dégradée, pour ne pas dire alarmantes, il apparaît en effet totalement incongru qu'une des 2 locomotives de la zone Euro et de l'Union européenne soit aujourd'hui le seul pays européen avec l'Espagne qui a connu pourtant une crise autrement plus violente à être sous le coup d'une procédure pour déficit excessif. être le champion de la dépense publique, avec pourtant une croissance plus faible que les autres pose question : la France, qui devrait être un exemple en Europe a une dette en effet plus élevé de 13 points que la moyenne européenne, il est donc temps de se redresser si José d'inverser la courbe. Et de vouloir équilibrer nos comptes en diminuant notre dette, cela passe assurément par des économies avant toute chose, mais ou faire les économies là est toute la question et si messieurs les Ministres, je l'ai vu vous partagez diagnostic peut-être divers journaux sur la Poste, je m'attacherai plus partir, a évoqué la situation Des collectivités locales puisque nous avons eu la chance d'accueillir le 1er, le président de la République de nombreux ministres, à la conférence nationale des territoires ce lundi au Sénat une conférence au cours de laquelle le président Macron a demandé aux collectivités de réaliser 13 milliards d'euros d'économies en 5 ans sur les 60 milliards d'euros de baisse annoncée de la dépense publique, je rappelle pourtant que les économies étaient initialement réparti différemment 10 milliards pour les collectivités et puis 25 milliards à parité pour l'État et les dépenses sociales. Dans son discours, si l'effort sur les dépenses, le le les collectivités locales, passe de 10 à 13 milliards c'est tout de même, excusez du peu, 30 pourcent d'efforts supplémentaires qui est demandé aux collectivités le montant global d'économies demeure à 60 milliards du du PIB, conformément au programme présidentiel l'effort supplémentaire au nom de la nouvelle situation dégradée des finances publiques ne serait donc portée que ou en grande partie par les collectivités territoriales de surcroît prendre comme référence la part dans la dépense publique, c'est oublier que la dépense des collectivités est très spécifique, ce sont certes des dépenses de fonctionnement, mais c'était avant tout des dépenses d'investissement qui représentent 70 pourcent de de l'investissement public en 2017, dont on sait qu'il est un catalyseur indispensable pour soutenir la croissance, mais c'est oublier également que la section de fonctionnement de Budgets de nos collectivités à l'obligation d'être à l'équilibre, sans capacité ni possibilité de recourir à l'emprunt, c'est oublier également que contrairement à l'État, le budget global des collectivités est excédentaire depuis 2015, grâce aux efforts qu'elles ont consentis et ça a été rappelé 3 milliards d'excédent en 2016, c'est oublier également que les efforts d'économie des collectivités ont déjà contribué pour moitié pour moitié à la réduction du déficit public en 2015 et 2016, c'est oublier enfin que leur part dans la dette publique est inférieure à 10 En réalité, 13 milliards c'est demander aux collectivités un effort encore plus important que celui qu'elles ont consentis dans le quinquennat précédent, certains ont appelé ça le régime de la double peine, alors même que nombre de collectivités sont exangue et ont déjà serré la ceinture au maximum le rabot ayant fait ses effets, vous leur proposez aujourd'hui et prenons-y garde de l'éleveur, vous leur proposez les effets du garrot hé bien attention parce que ça vient également avec des changements incessants d'échelle depuis plusieurs années, imposé par l'État pour gouverner, pour modifier les périmètres des territoires autant de réformes qui entravent la bonne gestion financière et qui donc. Ne donne pas, ni la visibilité ni la prévisibilité nécessaire au budget de nos collectivités alors pour, si j'ose dire, faire passer la pilule, le président de la République annonce que c'était fort ne passera pas par une baisse des dotations mais par un engagement des collectivités à baisser leurs dépenses de fonctionnement dans une, je cite : logique de confiance sans baisse de dotation, il ne peut en effet imposer cet effort sens heurté au principe constitutionnel, ça a été dit de libre administration des collectivités, cela passerait donc peut-être par une forme de contractualisation, sauf qu'il a ajouté que si l'effort demandé n'était pas respecté par certains, hein, je cite, mécanisme de correction serait mis en place à les suivantes le piège se referme l'emballage, l'emballage et 9 et plus mais le contenu reste la même, ce mécanisme de correction va de surcroît pénaliser les collectivités qui ont déjà fait des efforts, les années passées et peut-être favoriser les moins regardants tous les plus laxistes qui auront de ce fait davantage de marge de manoeuvre pour remplir les objectifs de réduction des dépenses. La seule réelle avancée a annoncé par le président Macron est la contrepartie à cet effort d'économies dans le cadre d'un pacte girondin, il est proposé en effet davantage de pragmatisme, de liberté, de flexibilité, d'expérimentation, la revue générale des normes avec la suppression de la règle du 2 pour 1 c'est une demande à laquelle évidemment le Sénat souscrit puisque il a fait partie de cette des institutions qui l'ont proposé l'augmentation également du temps de travail dans la fonction publique territoriale et le décrochage du point d'indice par une gestion différenciée des fonctions publiques, tout ça va dans le bon sens enfin, le président public promet une commission de travail autour de la réflexion sur une fiscalité locale mieux adapté et modernisé, nous ne pouvons que souscrire à cette proposition. Mais une telle mesure ne pourrait compenser la suppression annoncée de la taxe d'habitation, les élus locaux ne pourrait alors décider du taux de l'impôt national, il faut rappeler que le transfert d'une part de TVA aux régions visait à compenser la suppression de leur DGF une ressource dynamique remplaçait une dotation de surcroît la piste avancée par le président de la République et surprenante en proposant le transfert d'une part, disait-il, de siéger ou de CRDS qui serait de fait une perte en plus de financement pour la protection sociale, enfin si le selon le président République la taxe d'habitation et je partage est un impôt injuste et obsolète, alors pourquoi le maintenir mais nous l'avons déjà dit pour 20 pourcent des des Français qui serait d'ailleurs montré fustigé comme étant les privilégiés où les riches la réforme de la taxe d'habitation, pourrait, en outre, enfin et surtout contrevenir au principe constitutionnel d'autonomie financière des collectivités locales en faisant perdre 36 pourcent des des ressources propres du bloc communal

Nous pouvons nous interroger finalement sur la réalité de la décentralisation, aujourd'hui, avec des contraintes plus fortes imposées par l'État. Je veux faire le pari du dialogue confiant. Mais pas une confiance aveugle, parce que j'ai aussi entendu la vision macronienne de la République décentralisée qui pourrait s'apparenter par certains des propos entendus à celle d'une 3ème République où le maître d'école depuis l'Élysée demanderait aux élus locaux de rendre chaque année leur copie avec une punition à la clé, il n'était pas satisfait évidemment vous comprenez, je n'ose le penser surtout je l'espère pas le défi à relever est trop important pour notre pays, il nécessite de se faire confiance. Tous ensemble, et notamment aux élus. Pour lesquels l'engagement n'est pas une faute, mais une à motifs de fierté et je pense qu'il n'y a pas trop d'élus. L'engagement des élus aujourd'hui cet engagement pour servir à la fois sa commune et la République, c'est aussi pour servir la France, hé bien, faisons le pari du chemin du redressement de la France qui a besoin de tous et toutes ces bonnes volontés pour réussir demain et se construire un avenir meilleur, je vous remercie. Merci Simon chers collègues dans la suite du débat commun, la parole est à Monsieur François Marc, en remplacement de Madame Michèle André, présidente de la commission des finances à qui j'adresse mes très sincères condoléances en ce moment. De deuil familial, vous avez la parole monsieur Marc pour 5 minutes. Merci madame la présidente, effectivement, je prends la place de Michèle André, à sa demande pour vous lire l'intervention qu'elle souhaitait faire étant retenu donc dans sa famille en raison d'un deuil madame la présidente, monsieur, les milices, chers collègues, un débat conjoint sur la loi de règlement et les orientations des finances publiques est une bonne idée, car c'est à la lumière de l'expérience des exercices passés, qu'il faut analyser les orientations pour l'avenir, notre débat est bref mais je vous rappelle que les travaux du Sénat les travaux législatifs comme les travaux de contrôle ne se limite pas au débat en séance publique. Tout à l'heure, nous consacrons à moins d'une heure à la convention fiscale avec le Portugal, elle a pourtant donné lieu à énormément de travaux préparatoires de la commission et surtout du rapporteur, et je vous renvoie à son rapport. L'examen de la loi de règlement de lieux un lourd travail du rapporteur général mais aussi de tous les rapporteurs spéciaux et je vous invite à vous reporter au recueil de leurs observations qui sont autant de recommandations adressées au gouvernement en vue de la budgétisation 2018. Au terme de ces 3 années à la présidence de la commission des finances Michel-André pensent que le gouvernement a raison d'évoquer dans son rapport, la question de la procédure d'examen des lois de finances au Parlement car nous examinons les textes de loi de finances, mais aussi le collectif de fin d'année dans des conditions d'urgence déraisonnable, alors même que, contrairement à ce que j'entends ces dernières années, loi de finances n'est pas une prévision mais l'autorisation donnée par le Parlement au gouvernement de lever les impôts et de dépenser. La législation fiscale comme l'examen des propositions du gouvernement en matière de répartition des dépenses entre politiques publiques nécessitent un examen serein et approfondi dans la première condition et la disponibilité des ministres et de leurs administrations pour répondre aux interrogations des parlementaires et transmettre tous les documents utiles. Le débat politique porte aujourd'hui sur la stratégie budgétaire du nouveau gouvernement et à cet égard, il est utile de regarder l'exécution de 2016, on peut la résumer à grands traits, en constatant que le déficit public a continué de diminuer de 0 2 point de PIB. Si l'on regarde quelle a été l'impact des mesures décidées par le gouvernement, indépendamment de la conjoncture, ce que l'on appelle l'effort structurel. Il peut être constaté que les prélèvements obligatoires ont été diminué de 0 1 point de PIB donc de 2 2 milliards d'euros et que des économies dépenses ont été réalisés à hauteur de 0 4 point de PIB des économies ont été réalisées, tout en dégageant par ailleurs des moyens nouveaux pour la sécurité et la justice, les créations de postes dans l'éducation ou encore le service civique. On peut penser qu'une dizaine de milliards d'euros d'économies, ce n'est pas assez. Pour sa part, la présidente, pensent que la politique budgétaire a été bien doser suffisamment d'économies pour permettre une réduction du déficit, pas trop de coupes dans les dépenses pour ne pas casser la reprise de la croissance. ce qui conduit aux orientations pour 2018 et les années suivantes. Il y aurait lieu de d'appeler l'attention des uns et des autres sur la préservation des intérêts patrimoniaux de l'État. Vous voulez céder 10 milliards d'euros de participation pour financer l'innovation c'est louable, mais faites vos calculs pour l'État, céder des participations, plutôt que de s'endetter revient dans le contexte actuel a abandonné un rendement annuel de près de 4 pourcent sous sous la forme de dividende pour s'épargner le versement chaque année d'un taux d'intérêt proche de 0, est totalement rationnel. Sur la trajectoire des finances publiques. Michèle André, a observé que le gouvernement se fixe l'objectif d'évolution des dépenses le plus ambitieux de l'histoire de nos finances publiques 0 pourcent d'augmentation en volume pour l'ensemble des administrations publiques et ce, alors même que les précédentes cible moins ambitieuse dont jamais été atteint. Ne vous sera pas reprocher d'être ambitieux mais selon André voudraient des précisions sur la durée, quel montant annuel d'économies implique cet objectif et qu'elle serait à court terme, l'impact sur la croissance de l'art, il y a, Sion de ce programme d'économies. Ainsi, sur la nécessité de bien calibrer l'arbitrage entre réduction du déficit et préservation de la croissance, car il faut avoir une approche économique et non comptable des finances publiques, l'objectif principal, dans le respect de nos engagements européens, bien sûr, c'est la croissance et surtout l'emploi. Monsieur le ministre du Budget, qui est le gardien de l'unité du budget de l'État. La construction du d'un budget qui ne soit pas que l'addiction de sanctuaire sera d'autant plus ardu que vous avez insisté en commission sur la notion de sincérité vous avez indiqué vouloir ne plus recourir à ce que la Cour des comptes appelle des billets de construction. En citant les souvenirs Djezzy et recettes surévaluées, quels sont les autres billets auxquels vous avez décidé de ne plus avoir recours. Par exemple, allez vous vous interdire de reporter des dépenses sur l'exercice suivant pour piloter la fin de la de gestion. De mobiliser des crédits extrabudgétaires comme ceux du pays, a pour compléter le financement budgétaire d'un projet. D'inscrire des autorisations d'engagement sans prévoir les crédits de paiement de décaler les dates d'indexation pour gagner un peu de trésorerie. Allez-vous toujours rattachés les fonds de concours suffisamment tôt pour qu'il soit consommé dans l'année. Plus fondamentalement, et au-delà des arrangements budgétaire qui permet de tenir le déficit allez-vous toujours distingué dans vos annonces les économies de constatation et celles résultant de vos efforts et toujours explicité le référentiel en fonction duquel vos calculs rêve aux économies.

pas avoir peur de la transparence sur les choix que vous vous préconisez aux Français, ce sont les conditions de leur adhésion, de la vitalité du débat démocratique et pour le coup de la confiance dans l'action publique. Merci Merci beaucoup moins cher collègue, la parole est au président Alain Milon, président la commission des affaires sociales, monsieur le président, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues qu'il abhorre, une petite phrase que vient de me dire Serge Dassault c'est vrai que de ce côté-ci, quand on est là et qu'on garde l'hémicycle, on se rend compte que nous ne faisons pas recette et c'est bien dommage quand on parle finances dans ce débat d'orientation budgétaire d'orientation plutôt des finances publiques, je serai bref, monsieur le ministre, sur le bilan de la gestion passée que je résumerai en 3 points : un choc fiscal sans précédent, un changement de pied aux effets tardifs et des déficits persistants, le gouvernement a donné l'écho nécessaires à une situation désormais bien connu de tout ça et puis encore du Sénat dans ce débat, la question est plutôt celle de l'après, en matière de finances sociales, le gouvernement a annoncé une hausse de la contribution sociale généralisée, la CSG, pour un montant de 22 milliards d'euros et pour laquelle je voudrais tenter, comme c'est l'usage en matière de médicaments, une analyse bénéfice risque le bénéfice attendu est une hausse du pouvoir d'achat des salariés par la suppression des cotisations salariales d'assurance-maladie et d'assurance chômage pour un montant total de 17 milliards d'euros par an, mais risquent quant à eux sont nombreuses, rappelons que la CSG porte à 70 pourcent sur sur les revenus d'activité, c'est donc bien un prélèvement ainsi très majoritairement sur le travail, il y a bien sûr une assiette sur les revenus du capital, mais le gouvernement a annoncé qu'il ferait l'objet d'un prélèvement forte

augmenté le taux de la CSG, c'est prendre le risque d'un processus de mitage comparables à celui qu'a connu l'impôt sur le revenu, dont le produit 72 milliards est aujourd'hui inférieur de 26 milliards d'euros à celui de la CSG et se concentre sur les dette sur les de rémunération d'ores et déjà, le débat se porte sur les compensations, ils sont en effet bientôt à n'en pas douter sur les dérogations que faire pour les travailleurs indépendants dans la CSG porte sur le revenu, majoré des comptes, ils assurent social et qui ne paye pas de cotisations d'assurance chômage, que faire pour les fonctionnaires qui n'acquittent ni cotisations maladie ni cotisations chômage alors qu'il est par ailleurs indispensable de maîtriser la masse salariale publique que faire pour les retraités qui bénéficient d'un taux réduit de CSG et ne paye pas de cotisations salariales très récemment, les praticiens et auxiliaires médicaux se sont avisés que leurs cotisations étaient prises en charge par l'assurance maladie va-t-il falloir inventer pour le système spécifique de compensation, le gouvernement a annoncé en forme de compensation pour les retraités, une suppression de la taxe d'habitation pour 80 pourcent des des contribuables. L'expérience de la suppression de la demi-part des veuves nous enseigne que les compensations indirect de tout jamais exactement le même, il un élargissement du Champ des bénéficiaires de l'assurance chômage dans le régime aurait accumulé une dette de 40 milliards d'euros à l'horizon 2020 et qui seraient également, bien qu'il s'agisse d'Harris contributif, financé par une affectation de CSG, messieurs les ministres, le financement de la protection sociale est loin d'être un jardin à la française avec des prélèvements, simple, clair et compréhensible par tous, dans un paysage à fiscal d'une rare complexité ou impôts et cotisations se confondent dans leurs modalités leurs objectifs, les prélèvements ne seront légitimes et accepter que s'ils sont compris les impôts financent la solidarité les cotisations, les risques contributifs là quand transformation annoncée du CICE offre une occasion de mettre en oeuvre ce principe par la suppression des cotisations famille qui pèsent encore sur les salaires, la CSG dans le produit devrait être de 98 milliards d'euros cette année répond aux critères de la recette idéale produits stables assiette large

vous aurez compris, Monsieur le Ministre, que pour une diversification des ressources, la protection sociale, notre préférence va à une taxation de la sur la consommation, une assiette qui s'est toujours maintenu pendant la crise, un prélèvement progressif grâce au taux réduit de TVA et une taxation des produits importés alors que l'offre de 9 très 9 très économique peine à répondre à la demande des consommateurs, je vous remercie. Dimanche son en colère. Le débat est clos, nous passons à la discussion des articles du projet de loi, sauf si les ministres veulent répondre mais je vous en prie, monsieur, monsieur le ministre. Prétendant intervention de grande qualité, madame la présidente, après tant d'intervention de grande qualité, madame la présidence serait dommage que. Le ministre des comptes publics et moi-même nous ne répondions pas à certaines observations certaines remarques, je vais essayer d'être rapide parce que le temps est bref et laisser la parole ensuite Gérald Harman, un mot d'abord sur les observations très juste d'Albéric de Montgolfier, sur la question de la compétitivité coût et hors coûts dont dépend évidemment notre balance commerciale extérieure. Toutes les décisions que nous prenons, elle vise justement à rétablir aussi bien la compétitivité coût hors coûts de nos entreprises, pour améliorer le solde de la balance commerciale quand on décide de ramener le taux d'impôt sur les sociétés à 25 pourcent de de 33 aujourd'hui sur 5 ans, c'est un effort considérable, mais qui va améliorer les marges des entreprises leur profitabilité et donc la compétitivité coût. Quand nous décidons de financer massivement innovation en maintenant le crédit impôt recherche, en mettant en place un fonds de 10 milliards d'euros financés par des cessions d'actifs de l'État dans les entreprises du secteur concurrentiel, nous permettons à nos produits de monter en gamme d'intégrer l'innovation donc d'être plus compétitifs, enfin, je rappelle que le projet de loi PME TPE que nous porterons 2018, il vit justement à transformer nos entreprises en entreprise de taille intermédiaire capable d'aller sur les marchés extérieurs conquérir de nouveaux marchés, donc nous avons vraiment conscients, je crois, de l'importance de rétablir cette balance du commerce extérieur, de ne pas se reposer sur nos acquis, c'est-à-dire d'un côté, l'aéronautique, de l'autre, le vin et en 3ème le luxe et puis de continuer à tourner en rond comme ça, comme si avec 3 filières d'excellence en France, il y en a des dizaines d'autres, il suffit de leur donner les moyens d'exporter dans de bonnes conditions, un mot également sur les questions de croissance potentielle et de rétablissement des soldes structurels côté soulevée par plusieurs intervenants, nous avons fait un choix avec Gérald Herrmann avec le 1er ministre avec le président de la République qui est un choix très novateur, qui est de ne pas surévaluer la croissance potentielle dans la trajectoire quinquennal, je rappelle que précédemment sur les toits, même chose, c'est-à-dire qu'on établit une croissance potentielle très au-delà de ce que nous pouvons réaliser 1,5 le plus souvent, et puis à la fin de l'année, on s'aperçoit que la réalisation n'est pas à la hauteur de ce qui était espéré et il faut réviser par conséquent la réalisation budgétaire bien là, nous avons fait un choix très différents, nous mettons une croissance potentielle à 1,25 pourcent,, c'est-à-dire exactement ce qu'estiment les plus grands centres d'évaluation étrangers internationaux et européens, je pense que pour le coup, c'est un gage de sincérité et d'honnêteté de la trajectoire budgétaire que nous avons retenus. Un mot également sur le prélèvement forfaitaire unique et sur le Livret A pour bien préciser, toute la question était posée à plusieurs reprises que le prélèvement forfaitaire unique concernera les intérêts, les dividendes et les plus-values mobilières et je dirais à Serge Dassault, je pense avoir eu l'occasion de lui dire : une bonne centaine de fois que ce prélèvement forfaitaire unique qui n'est pas très éloigné de la flat axes qu'il défend aussi souvent par ailleurs j'estime qu'avoir de la progressivité dans l'impôt, c'est un gage de justice et que la justice, c'est ce qui rend les prélèvements obligatoires acceptable, donc avoir un prélèvement forfaitaire unique et garder de la progressivité dans l'impôt. C'est conjuguer l'efficacité fiscale et la justice fiscale.

ne sont pas faites pour être strictement respecté, sinon ça sert à rien d'avoir des responsables politiques qu'ils soient sénateurs, députés ou membre du gouvernement, nous sommes là justement pour essayer de prendre des décisions raisonnables en fonction des indications qui nous sont données, je rappelle que nous avons des évaluations d'inflation qui sont encore moins forte que prévu autour de 0 7 pourcent en en juin, je rappelle que la rémunération dans ce contexte-là va rester attractive pour les épargnants, dans un contexte où les rendements financiers restent faibles, du fait de la politique monétaire accommodante menée par la Banque centrale européenne et je redis également à ce qui l'aurait oublié cette stabilité, elle est favorable au secteur du logement social puisqu'il emprunte auprès de la CDC, à un taux

mais nous gardons la possibilité de financer le logement social dans les meilleures conditions possibles. Enfin, un tout dernier mot mais je pense que Gérald Darmanin complétera ça beaucoup mieux que moi sur la question des génies délité jeudi, notamment pour François Marc, le gouvernement. Gérald Harman à moi-même. Nous avons parfaitement conscience que la lutte contre les inégalités, être une priorité. Et du point de vue strictement économique, je suis le 1er, convaincu que les inégalités sont défavorables à la croissance. L'idée qu'on va faire de la croissance en creusant les inégalités est une erreur. Il faut arriver à créer de la croissance et à réduire les inégalités parce que l'un va avec l'autre et qu'une croissance qui ne profiterait qu'un petit nombre de personnes d'une croissance qui serait à la fois inutile et en plus, très probablement une croissance faible, mais quand nous décidons de supprimer la taxe d'habitation pour 80 pourcent des quand nous décidons d'augmenter l'occasion pour adultes handicapés quand nous supprimons les cotisations patronales sociales sur l'assurance maladie ou sur l'assurance chômage bien nous réduisons les inégalités et je rappelle que nous avons fait aussi des choix qu'on ne mentionne pas souvent mais qui est de reprendre un certain nombre de décisions du précédent gouvernement dont nous estimions qu'elles étaient justes, même si elles étaient coûteuses. Avez le crédit d'impôt sur l'emploi à domicile. Nous avons décidé de maintenir ce crédit d'impôt sur l'emploi à domicile qui coûte près d'un 1000000000 d'euros aux contribuables, aux finances publiques françaises mais nous l'avons décidé parce que ça permet à des ménages modestes d'avoir accès à l'emploi de missiles notamment des retraités, avec un niveau de retraite très faible quand on nous accuse de taper sur les retraités, je rappelle que ce dispositif sur l'emploi à domicile, sous forme de crédit d'impôt va permettre à des retraités qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, d'avoir accès à des emplois à domicile et en plus c'est bon pour l'emploi, ce qui reste évidemment notre priorité à tous. Merci, Monsieur le Ministre d'vous avez la parole. Merci à la présidente pour compléter les propos de de Bruno Le Maire sur les question plus budgétaire d'abord évoqué la question de de cette fameuse baisse, même si peut-être les interlocuteurs ne sont pas tous présents mais compte rendu et leurs collègues le répétera la baisse du des dépenses publiques, évidemment on peut toujours en souhaitait davantage mais si on baisse le budget si l'on regarde par rapport au pourcentage du PIB, ce sera effectivement une baisse qu'on n'a jamais obtenu depuis le début de la crise économique des années 70, donc il me semble que c'est tout à fait à la fois exaltant et difficile, je comprends que les sénateurs soient désormais extrêmement exigeant avec ceux qui essaye d'être courageux en ce début d'année quinquennal budgétaire si j'ose dire, mais je pense que ce sera déjà une très grande chose, sachant qu'il y a des tendanciel qui sont déjà très. Or, l'augmentation de la la population par exemple nous pousse à faire évidemment quelques quelques dépenses de manière générale, je dois dire que je regrette même de la de la bouche même du du rapporteur général, même s'il a eu des propos tout à fait encourageant pour le gouvernement et je prends comme tels que il y avait beaucoup de listes d'économies proposées puisqu'on nous a dit qu'on faisait pas touche aux armées pas l'intérieur pas toucher la justice ne veut pas toucher les cultures pas seulement supérieur non plus, pas aux collectivités locales, c'est faire attention à la sécurité sociale, donc je voudrais savoir si c'est que sur les inspecteurs des impôts de Bercy qu'on veut faire des économies non je sais pas c'est interpellation ne soit votée en juin c'est de manière générale, je n'ai pas entendu beaucoup de propositions d'économies pourtant tout mauvais accord pour que nous fassions des économies, mais en revanche, c'est un petit peu difficile de savoir où est-ce que les parlementaires proposer ses économies voilà donc à votre bon coeur pour le débat de la loi de finances. Si vous trouvez que nous, les économies sont pas bonnes et je n'ai pas proposer les mêmes sommes ailleurs et je suis sûr que ce sera facile à à faire assez rapidement sur les collectivités locales, il est vrai que les collectivités locales et Julie moi-même cela dans le dans les secours pour être un élu local moi-même, il est vrai que les collectivités locales ont fait des efforts et les efforts importants qui sont souvent la conséquence à la fois leur bonne gestion, pas toutes, mais souvent mais aussi quand même de la baisse des dotations renforcer ces ces économies cependant sur la dépense publique, mais c'est un un constat sur la dépense publique, c'était pour entre 2010 et 2016 en tout cas plus rapide que pour l'État, ce qu'on a 06 de dépenses publiques pour les collectivités locales, on est à 0 ne me semble-t-il pour pour l'État, donc voilà, c'est notre problème à nous, c'est une preuve de dépenses publiques, même si j'entends que l'État et c'est ce que nous proposons cette année face plus de 50 de l'effort parce qu'il ne l'a pas fait précédemment dans les 2 dernières années au mois de diminution de dépenses publiques, donc il il faut vraiment qu'on regarde ces choses autant que j'entends l'argument sur le solde mais

d'autant qu'à la fin, c'est comme les Français qui vont le payer d'une manière ou d'une autre, mais j'entends l'argument et je pense qu'on a, on dit pas totalement les choses très différentes, je n'ai pas entendu leur la bouche, sénateur de gens qui disaient qu'il est pas du tout faire d'économies sur les collectivités locales, d'abord parce qu'il faut aussi faire des réformes de structure, y compris dans les collectivités locales, c'est ce que nous proposerons avec le ministre d'État en charge de l'Intérieur lors du début des des groupes de travail sur la conférence des territoires sur les dépenses sociales répondent à monsieur le rapporteur général, moi je voudrais juste dire que

avons, si nous sommes en reprise économique, c'est la croissance hé bien plus grande que que nous le prévoyions nous-mêmes, ne serait-ce que par pur bon sens et et par envie effectivement comme dit Bruno Le Maire de ne pas spéculer et faut pas voir revenir vers vous en disant trompé sur les chiffres de croissance il il faut profiter de cette embellie puisque Sion, dépenses publiques drastiquement et surbaissé, fiscalité, c'est que nous espérons quand même qu'il reprise économique conforme aux présidentielles, donc l'objectif c'est dépassé 2021 monsieur rapporteur général et puis de pouvoir a atteint des excédents. Et surtout je pense que sur les dépenses sociales, comme sur la la sécurité sociale revoir sans faire cette politique de rabot qui qui qui énerve tout le monde qui désespère aussi nos concitoyens, ça a été dit d'ailleurs par la présidente de la de la commission, je pense qu'il faut vraiment l'expliquer, elle a tout à fait raison à nos concitoyens, il faut sans doute que nous ayons de l'innovation un changement structurel, y compris sur les les sujets qui vous intéressent tout particulièrement, mais je sais, à la fois les rapports que vous commettez les propositions et ils seront bien évidemment étudiés à la semaine nationale et bien sûr dans cette maison particulièrement simplement dire une dernière chose, peut-être sur les collectivités locales devant la chambre qui représente tout particulièrement. Sur les valeurs locatives depuis et 70 la locative sont pas revus,

pour arriver à cette réforme, qui maintenant est en place, bon, donc ça c'est valeurs, elles sont nouvelles, mais elles sont désormais mais nous avons les valeurs locatives d'habitation,

il y a 15 jours a on va toujours répéter sans cesse la répétition et la pédagogie est l'art de la répétition, mais je suis certain que monsieur Dallier se souvient quand même de lui, j'ai bon, donc oui, nous allons travailler à cette question, mais cette question malgré tout pour à la fois l'affaire sera sera longue, on est aux accords qui va faire beaucoup de travail, d'abord de la part des agents de la direction générale des finances publiques, mais aussi de la part des parlementaires d'un comité des finances locales, ce qui ne veut pas dire qu'il qu'il faut arrêter et que l'unique : réforme de la fiscalité locale ne soit que les valeurs locatives, nous proposons, et ça l'a été dit par le président de la République, alors j'entends le point sur la CSG ou la CRDS, c'est un exemple qui l'a pris, il a pris une variété d'autres moyens de financer dans l'accident, ce que vous avez voté l'occurrence ce que vous n'avez pas discuté monsieur rapporteur général, mais il y avait quand même un instrument notamment pour les régions qui va s'appliquer l'année prochaine, qui consiste à donner un point de TVA en suppression de la dotation ça c'était décidé par le ce moment qui a pas été mis en place, parce que sa notation sont très dynamiques et peut-être permettrait d'ailleurs de regarder les futures compétences que nous que nous pourrions continuer à donner aux régions, aucun un gouvernement celui-ci ou d'autres envies de faire donc le président de la République a évoqué une piste de réflexion, il a demandé que l'imagination soit au pouvoir, nous allons mettre en place imagination collective peut-être est-ce un point ou 2 points de quelques impôts nationaux, peut-être que c'est pas le la bonne chose à faire, peut-être qu'il faut imaginer un nouvel impôt local qui supprimera 5 serrés et et le reste en attaque délectation là qu'il faut garder intact foncière, mais si on recentraliser RSA peut-être que c'est une question qu'on peut reposer avec les collectivités locales, enfin en cette semaine, on va pas recréer l'exacte copie vous diriez mais il y a pas de concertation, donc ce que nous avons prévues en méthode à la demande du 1er ministre et et pour mette concrètement le discours du président de la République en verve, c'est avec le ministre d'État mis à l'intérieur avec mise à cohésion des territoires pendant les 3 mois qui arrivent et le Sénat, il sera pleinement associé bien sûr dans ces groupes de travail, comme bien sûr un président de commission ne souhaite rapporteur général devant la commission des finances, nous regarderons quel est le meilleur moyen à la fois de supprimer, c'est étrange est exaltation je voudrais juste rappeler que c'est la volonté du peuple français a travaillé, qui ont prévu des élections présidentielles et les élections législatives, bon moi je n'ai cours par la TVA, mais ça pas eu un succès d'estime énorme c'est tellement vrai que lorsque la présidentielle a été perdue par François Fillon y a républicains se sont empressés de supprimer cette très bonne idée d'augmentation de points de la TVA voilà donc ça devait pas être forcément la plus grande idée fiscale du monde sinon elle aurait sans doute été présenté dans les électeurs aux élections législatives, je, je, je, faire je ferme la parenthèse bon mais nous allons donc travailler aujourd'hui à ses pistes pour pouvoir rénover la fiscalité locale pour qu'elle soit à la fois et j'en terminerai par là la présidente juste pour nos concitoyens, juste pour les collectivités locales parce que vous l'avez tous dit et nous disons à nouveau, c'est injuste, territorialement et que nous respections l'autonomie financière des collectivités locales, mais je voudrais rappeler ici qu'il n'y a pas, comme j'ai entendu tout à l'heure dans les rangs d'un de vos collègues, vous savez d'autonomie fiscale, la Constitution la constitution mais tout à l'heure, la question était : autonomie fiscale ne prévoit pas l'autonomie fiscale peut-être est-ce une évolution qu'il faut imaginer pour un certain nombre de sénateurs, mais en tout cas c'est pas le cas d'aujourd'hui et l'autonomie financière, elle est garantie par le fait que soit des dégrèvements voilà donc je l'ai dit, je suis désolé, pas répondre plus précisément aux interrogations mais il me semble des pistes et je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, on aura l'occasion de revenir sur les pistes très concrètes que le gouvernement proposera après concertation. Merci monsieur ministe.

y a-t-il des oppositions, je n'en vois pas. Donc, qui est pour l'article liminaire. Je répète ma question qui est pour l'article liminaire et je vous rappelle qu'il se vote vaudra pour tous les autres articles, donc il est pour l'article liminaire. 3, ce qui

je veux mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2016 il y a-t-il des demandes d'explications de vote. Oui, Monsieur Dominique, je vous en prie. Oui, très rapidement, merci madame la présidente, messieurs les ministres, cher collègue, souligner tout le travail de fond qui a été fait à l'intérieur, à la fois la commission des finances, la commission des affaires sociales, parce que je dirais les les 2 rapports, le tome 1 et tome 2 sont particulièrement pédagogique et c'est vrai que, à la lecture des différents rapports, qui concerne les différentes missions, on tient à souligner, je dirais aussi la complexité notre collègue Alain Milon en parler aussi tout à l'heure de complexité je confirme tout à fait et vous je voudrais aussi sur ces différents articles même principe pour le budget de l'État que pour nos collectivités territoriales, et on a fait beaucoup référence c'est la loi de de règlements, c'est ce qui équivaut aussi à à au compte administratif au compte de gestion de nos collectivités territoriales mais c'est vrai que les dépenses qui sont ce qu'elles sont, c'était, rappelez 11 milliards d'euros, avec un déficit pour l'exercice 2016, qui s'élève à 75 moins 75 milliards d'euros, la situation est-ce qu'elle est, beaucoup se sont exprimés, beaucoup de nos collègues, bon après, j'ai renoncé qu'il faut faire des efforts de maîtrise des des dépenses et, gouvernement après gouvernement c'est souvent rappeler après les recettes sont ce qu'elles sont, on a parlé aussi souvent d'insincérité en terme de de recettes mais joueurs relire naturellement à la vie de notre commission des finances en saluant aussi réellement tout le travail de fond qui a été fait aussi au sein des commissions aussi par l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs, je vous remercie. Merci, il y a-t-il d'autre demande d'explications de vote, je n'en vois pas je me vois le projet de loi de règlement du budget d'approbation des comptes de l'un des 2016 en application de l'article 59 du règlement, le scrutin public et de droit, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin sera ouvert dans quelques instants.

Plus personne ne demandera voter le scrutin clos invite les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin numéro 125 sur l'ensemble du texte compte de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs groupes politiques et notifié à la présidence, nombre de votants 333 Nombre de suffrages exprimés 187 pour l'adoption 126 7 contre 60, le Sénat a adopté définitivement. Mais, chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant la ratification merci monsieur le ministre. Nous en gardons aller 2 monsieur ministre Dormans. l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi donc autorisant la ratification de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal pendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu dans la discussion générale, la parole est à monsieur Gérald Darmanin Ministre de l'action et des Comptes publics la parole monsieur le ministre.

l'avenant signé le 25 août 2016 avec le Portugal, qui vous est soumis aujourd'hui et ciblée sur 2 catégories de dispositions prioritaires pour les autorités françaises. D'abord résoudre les difficultés de nos compatriotes qui exerce ses activités du sel de service public, au Portugal et notamment des enseignants de de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger qui participent aux Liens culturels entre nos 2 pays mais aussi et c'est le 2ème Point renforcer notre coopération initiatives de manière très opérationnelle dans l'objectif de lutter contre la fraude et d'évasion fiscale, la France et le Portugal sont liés en matière d'impôt sur le revenu par une convention fiscale de 1971 or dans le cas des réduire Sion et des pensions publiques, elle prévoit un droit d'imposer, partagée entre l'État de résidence et celui d'origine du revenu, à charge pour le 1er d'éliminer le la double imposition, je vous rappelle que les diplomates, quant à eux, obéissent à un régime différent qui leur est propre, celui de la convention de Vienne de 1961. Dès lors que le Portugal a commencé à exercer. Son droit d'imposer les rémunérations et pensions publiques versées par la France à compter des revenus de 2009 système complexe prévu par la convention fixe fiscal actuel a donné lieu à de nombreuses difficultés. Nos agents publics et notamment les enseignants et lycées français qui avaient généralement d'éclaireurs énumération et payer en impôts en France ont immédiatement exprimé une forte incompréhension face aux contrôle engagé à leur égard par l'administration portugaise, même si ces derniers étaient conformes à la convention fiscale. Le ministère des Finances français a donc engagé sans tarder des démarches à l'égard des autorités portugaises pour remédier à cette situation, la France et le Portugal étant membre de l'Organisation de coopération de développement économique, les travaux se sont appuyés sur le modèle de grand saut fiscale publié par celle-ci, l'OCDE prévoit ainsi que les re-numération et pensions publiques sont imposables est-ce que Zeev ment dans l'état d'origine du revenu ou bien dans celui de résidence, c'est les contribuables en a la nationalité ce principe d'imposition et ceux qui disparaît un état est une simplification essentiel par rapport à l'état actuel de la grande franco-portugaise ainsi de manière concrète. Dans le dispositif qui vous est soumis nos compatriotes résidant du Portugal percevant des rémunérations publiques d'origine française serait désormais exclusivement imposables par la France de plus dans le but de tenir compte notamment de la situation des établissements d'enseignement, le gouvernement portugais a accepté d'aller plus loin que le modèle de l'OCDE, il y a 2 répondent favorablement à notre demande d'étendre ce régime aux binationaux franco-portugais. Je tiens ici à remercier le Portugal ces autorités pour les pensions publiques le même principe s'appliquerait à savoir l'imposition et ce qu'il vivent dans l'état d'origine, toutefois, dans ce cas, il n'a pas été possible de déroger au modèle de l'OCDE en conséquence et personnes percevant des retraites publiques d'origine française, serait à l'exclusivement en France, sauf s'ils ont la nationalité portugaise, qu'elle soit binationale ou non, auquel cas seul le Portugal pourrait alors les imposer enfin de manière à régler d'ici. Question actuellement pendantes aucun seront centrés nos agents publics au Portugal, ces dispositions s'appliquerait de manière rétroactive. Or énumération pension versée à compter du 1er janvier 2013. Là encore les autorités portugaises ont été sensibles, il y a des métiers culturels existants note note entre nos 2 pays désormais action à nouveau. L'avenant qui vient de vous être soumis comporte un autre volet, également très important qui concerne effectivité de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale en effet l'actualise dispositif bilatéral d'échange de renseignements de la convention fiscale et il ajoute un mécanisme d'assistance recouvrement en sont conformes dans les 2 cas aux normes les plus récentes de l'OCDE, rappelons que, conformément à la directive européenne de 2014 la France et le Portugal doivent par ailleurs échanger automatiquement les informations sur les comptes financiers ici de 37 en 2017 enfin l'avenant introduit dans la convention fiscale une clause anti-abus, destiné à éviter des montages d'optimisation visant à bénéficié indument des avantages conventionnels et s'inscrit dans la lignée du projet de lutte contre l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices des fameux projet d'de l'OCDE et du G20 et anticipe en particulier sur l'accord Multina multilatéral signé dans ce cadre, le 7 janvier 2017, à Paris, monsieur le rapporteur par plus de 60 pays pour ces raisons, et sans être plus long, c'est dans l'accord de l'entrée en vigueur est très attendu que nous vous demandons de voter le Portugal a achevé sa ratification le 3 avril 2017 et interviendra dès que la France aura fait de même, je vous invite donc à approuver la ratification de cet Allemand proposé par le gouvernement qui est porteur de progrès au plan fiscal et qui permettra de faciliter la vie de nos agents et retraités public au Portugal, je vous en remercie. Merci monsieur le ministre, n'a parlé que monsieur Éric Doligé, rapporteur de la commission des finances. vous avez la parole pour 10 minutes, mon cher collègue. madame la présidente, pardon. Monsieur le Ministre, c'est-à-dire d'un gouvernement d'union nationale, comme le dirait notre ami Serge Dassault et comme ça a l'air de vous plaît, je le répète, chers collègues, nous examine aujourd'hui le projet de loi autorisant la ratification de l'avenant du 25 août 2016 à la convention fiscale franco-portugaise qui date du 14 janvier 1971 je compris ce milices de m'excuser de répéter un peu ce que vous avez dit il y a quelques instants. En soi, cela mérite d'être très signalé en décembre dernier à l'Assemblée nationale, le gouvernement avait déposé un amendement tendant à autoriser la ratification de cet accord par un simple article au sein de la loi de finances rectificative, le Sénat s'y était opposé, estimant que la ratification d'une convention fiscale n'avait pas sa place dans une loi de finances, le Conseil constitutionnel avait ensuite confirmé notre position en change sur en l'article en question, je me permets d'insister sur c'était pilote car il me semble que nous avons ainsi éviter de créer un précédent fâcheux que le gouvernement successifs aurait sans doute eu la tentation de répéter, monsieur le ministre est exemple montre si c'était nécessaire, que nous sommes attentifs et avant une certaine expertise, même si cela ne semble plus nécessaire pour un parlementaire, j'en viens maintenant au fond du présent accord, sans entrer dans les détails, celui-ci poursuit un double objectif : premièrement il vise à mettre en conformité avec le modèle de l'OCDE, les règles applicables à l'imposition des rémunérations et pensions publiques en prévoyant une imposition exclusive à la suite, la convention franco-portugaise de 71 actuellement en vigueur et dérogatoire sur ce point en ce qu'elle autorise aussi l'imposition par l'État de résidence du bénéficiaire cette particularité longtemps sans effet est devenu problématique en 2013 lorsque le Portugal, alors en pleine crise économique a engagé une série de contrôles fiscaux à l'encontre d'agent. Et de retraités de la fonction publique française résidant au Portugal, en fait, les personnels des lycées français de Lisbonne et de Porto, ceux-ci se sont à leur retrouver dans une situation difficile, l'impôt sur le revenu étant sensiblement plus élevé au Portugal les redressement portant sur plusieurs années, suite à l'intervention de la France, le Portugal a accepté de renégocier la convention fiscale et de la mettre en conformité avec les principes de l'OCDE, deuxièmement, c'est un plan vise à moderniser les dispositifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale sur 2 aspects, que vous avez cités, d'une part, les échanges d'informations. La France et le Portugal, étant précisé que les 2 pays appliquent déjà le standard le plus élevé en vertu d'engagements multilatéraux géant européen, d'autre part, l'introduction de de clause anti-abus permettant d'écarter les cas ou bénéficiaires d'un revenu dans n'est pas le bénéficiaire effectif ou lorsqu'il apparaît que l'opération un objectif principalement fiscales tous ces éléments constituent des modifications bienvenues de la convention franco-portugaise de 1971 justifie la ratification de l'avenir, je souhaiterais toutefois prendre le temps d'adresser une série de questions au gouvernement, qui ne porte pas tant sur l'avenant lui-même que sur le contexte dans lequel il s'inscrit sur le 1er sujet l'avenant prévoit que les nouvelles règles relatives aux rémunérations et pensions publiques auront une portée rétroactive à compter de 2013 afin qu'elle puisse s'appliquer aux contrôles engagés par le Portugal, c'est une disposition bienvenue mais il se trouve que dans les cas des binationaux fait rétroactivité n'est pas le même selon qu'ils soient actifs qui seront à alors imposer à la source par la France aux retraités seront eux alors imposer à la résidence, c'est-à-dire par le Portugal, ce qui était un a priori moins favorable. Les règles applicables retraités sont conformes au modèle de l'OCDE ne sont pas contestables sur le fond, ceci dit, s'agissant de dossiers en cours, elle place les quelques rares personnes concernées dans une situation difficile, alors même que les enjeux pour les 2 États sont modestes et que chacun semble vouloir faire preuve de bonne volonté, monsieur le Ministre, pourriez-vous nous indiquer s'il est envisageable que le Portugal accepte de clore définitivement ces quelques affaires par une mesure de clémence fiscale, quitte à ce que celle-ci porte sur les seuls majoration de pénalités, naturellement, une telle décision relève de la compétence exclusive du Portugal, mais pourriez-vous nous dire si la France a engagé des démarches en ce sens sur le second sujet, celui de la lutte contre la fraude élévation fiscal, vous savez qu'une forme d'incertitude plane aujourd'hui sur l'ensemble des conventions fiscales signées par la France le 7 juin dernier les représentants de quelque 76 pays ont signé la convention multi-. Latéral de l'OCDE pour la mise en oeuvre mais mesures du plan Bex de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices cet instrument très ambitieux, la modifier en une seule fois les dispositions anti-abus de quelque 1105 conventions bilatérales dans le monde, dont la convention franco-portugaise, or, en l'absence de version. Consolider de la convention, il nous est impossible de mesurer précisément la nature et l'ampleur de ces modifications, nous en avons par exemple identifier une sur la notion très importante d'établissement stable si la France avec. C'était sans réserve les modifications contenues dans l'instrument multilatéral de l'OCDE, elle n'est pas le Portugal par conséquent cette clause ne s'appliquera pas intégralement, même si cela n'apparaît pas explicitement nulle part, des divergences de ce type très techniques sont susceptibles d'apparaître sur d'autres points et dans d'autres accords, monsieur le Ministre, pouvez-vous. Vous engagez à ce qu'à l'avenir, dans le cas de l'examen de conventions fiscales le Parlement dispose d'une information claire lisible et exhaustive sur ce que chaque instrument multilatéral pour chaque stipulations ce que change l'instrument multilatéral pour chaque stipulations et dans chaque accord cela nous sommes indispensables à une autorisation éclairé de du législateur. S'agissant ensuite de l'échange d'informations fiscales, la principale source d'information du législateur et du jaune a dunk c'est au projet de loi de finance de chaque année, qui permet de juger de la bonne ou de la mauvaise coopération coopération d'un État avec la France, or ce document n'a été publié, ni pour l'année 2015, ni pour l'année 2016, ni à ce jour pour l'année 2017, en dépit des engagements répétés du gouvernement précédent, et alors même que tout est en train de changer avec le passage à l'échange automatique, monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire si ce document sera publié pour l'année 2017 et si oui à quelle date. à l'avenir, si le gouvernement estime que ce document n'est plus le support le plus pertinent, quelles sont les alternatives envisageables pour améliorer l'information du Parlement je souhaiterais évoquer un autre sujet lié à la fiscalité, qui concerne la France et le Portugal, bien qu'il ne figure pas dans le président afghan, il s'agit du statut des résidents non habituel RN H. vous avez sans doute entendu parler de ce statut fiscal avantageux auquel nombre de reportages à des télévisions ou dans les hebdomadaires ont été consacrés, il permet aux particuliers qui réside au Portugal, plus de 193 jours par an, et notamment aux retraités de bénéficier pendant une période de 10 ans d'une exonération totale d'impôt sur le revenu sur le revenu de sources étrangères en principe. Bien sûr, untel régime relève de la souveraineté fiscale du Portugal qui tant qu'État de résidence peut choisir d'exercer ou non son droit d'imposer, il existe depuis longtemps un consensus international sur le sujet mais par 2 décisions de 2015 le Conseil d'État a jugé que pour se voir reconnaître la qualité de résident fiscal d'un État, il ne fallait pas seulement être imposables dans cet état mais il effectivement imposer ses décisions ne portait pas sur le Portugal, mais pourrait trouver acier appliquer, ainsi d'ailleurs que d'autres pays qui offrent des avantages similaires aux retraités les étrangers comme le Maroc, si telle était le cas, les Français ne pourrait de facto plus bénéficier du statut de résident monde habituel au Portugal, à vrai dire, le sujet est très complexe et devrait être appréciée au cas par cas, tant les situations sont diverses, ainsi, faudrait-il aller jusqu'à refuser les écrans exonération. Par cette Jetta en vertu de critères tels qu'une famille nombreuse ou de revenus modestes. Une entreprise exonérés en échange de la construction d'une route dans une zone géographique isolée doit-elle être traité comme un géant du numérique contre contre l'achat d'une boîte aux lettres, la France accepterait-elle qu'un autre etarra met en cause son choix d'exonérer les organisateurs des Jeux olympiques. De 2024, bref une clarification de la doctrine semble aujourd'hui nécessaire monsieur le Ministre, pourriez-vous nous donner ici quelques précisions sur la manière, dans l'administration fiscale, entend faire application de cette décision du Conseil d'État. Dans lequel cas estime-t-elle légitime qu'un résidant d'un autre État puisse être exonérées sur ses revenus de choses. Français, sans pour autant que cela entraîne un redressement équivalent en France, qu'en est-il, en particulier du cas du Portugal sait-on combien de personnes sont concernées, s'il s'agit surtout d'actifs ou de retraite. à à titre personnel, il me semble d'ailleurs pas forcément opportun d'imposer rétroactivement, ceux qui ont choisi ce statut car si car ils l'ont fait de bonne foi et en toute conformité avec le droit existant, de plus la fiscalité n'est pas forcément leur motivation principale car ce statut concerne de nombreuses binationaux reste qu'il y a bien là une forme de concurrence fiscale offensive d'ailleurs pleinement assumé par le Portugal, qui offre aussi des Golden visas aux étrangers hors Schengen est comprise comme telle par d'autres pays, à l'instar de la Finlande qui à négocier une nouvelle convention fiscale, mettant fin à cette possibilité, au fond, monsieur le ministre. Tout pourrait se résumer ainsi : comment le nouveau gouvernement entend-il impératif de lutte contre la concurrence fiscale agressive, d'une part et le respect de la souveraineté fiscale des États, d'autre part pour l'ensemble des raisons que j'ai évoqué, il me semble que l'avenant constitue un bon équilibre et qu'il est souhaitable de l'approuver, je vous remercie Monsieur si vous pouvez répondre mais différentes questions voilà madame. Merci monsieur Doligé la. je vous en prie, je vous laisse ce temps de boire sans aucun problème. Monsieur de lui je ne se représente. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Thierry Foucaud pour le groupe communiste républicain et citoyen pour 4 minutes. Présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, oui la convention fiscale dont nous débattons aujourd'hui vise à mettre en pratique la relation et relations et les modes d'imposition des revenus entre 2 pays membres de l'Union européenne à la nuance près que l'le Portugal n'était pas encore lors de la signature de la convention d'origine. Dans cette situation, oui, je pourrais aussi ici pour garder en mémoire les problèmes que nous abordons aujourd'hui de se rappeler l'apport essentiel de la communauté portugaise dans le développement de notre pays, au fil des années 60 et et la des gens du pays à la Communauté européenne au début des années 1980 donc à l'ancrage du Portugal dans le siècle,

merci facilitée par le statut de résident de résident non habituel n'a rien de commun avec d'autres montages et dispositifs utilisés dans certains paradis fiscaux plus connu que le Portugal, il n'en demeure pas moins qu'il conviendrait que les pays de l'Union européenne n'ait pas recours à ce type de mesure pour se rendre bien sûr plus attractif, alors il nous faut ainsi bannir dans notre législation, même ce qui pourrait en tenir lieu, pour le reste, les choses ont été dites, eu égard au 1000000 et demi aussi de Portugais de franco-portugais de toutes générations qui habite où habiter notre pays, nous ne pouvons que nous associer à la ratification de l'avenant de la convention fiscale. Mon cher collègue, la Pareto Monsieur Guillaume Arnell pour le, on perdait et ce pour 3 minutes-moi

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur de la commission des finances mais, chers collègues, la convention fiscale avec le Portugal, dont nous discutons ce soir renvoie tout débat plus large du mouvement de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, nous savons que les pratiques mises en oeuvre par certaines multinationales aboutissent à l'évaporation de plusieurs centaines de milliards de dollars chaque année dans le monde des agissements qui s'les dépenses publiques, de faire taire pays ou forces la concurrence économique dans cette lutte en juin dernier 76 pays ont manifesté l'intention de signer l'instrument multilatéral de l'OCDE qui concerne 4 domaines dont celui des conventions fiscales dès lors comme l'a souligné, notre collègue rapporteur monsieur Lollivier quelques incertitudes demeurent quant aux conséquences de cet accord, or sur les conventions fiscales bilatérales en attendant d'éventuelles réponses. Le projet de loi nous invite néanmoins approuvé cet avenant à l'accord ou bilatéral qui lie la France et le Portugal par la convention du 14 janvier 1971 mais mais Colin du RDS et moi-même approuveront ce texte qui vise à renforcer l'échange de renseignements mais aussi à répondre aux difficultés survenues depuis 2013 pour quelques quelques contribuables installés au Portugal, en effet, si les conventions fiscales bilatérales établissent des règles initialement accepté par chacune des parties contractantes le zèle soudain de l'administration fiscale peut conduire à des situations de redressement comme celle que connaissent aujourd'hui, quelques enseignants d'établissements français à Lisbonne ou à Porto, le texte a pas me semble-t-il, une solution équilibrée dans le respect des standards de l'OCDE, nous connaissons tous, mes chers collègues, les relations enfantine, le Portugal et la France, nous n'ignorons pas non plus les problèmes économiques de ce pays qui ont peut-être motivé une nouvelle interprétation de l'accord avec la France sur la double imposition et en dehors de cet accord, le développement offensif du régime fiscal des résidents non habituel, sans remettre en cause la souveraineté fiscale du Portugal, nos 2 pays étant partenaires au sein de l'Union européenne et partage à ce type, les valeurs de solidarité, tout ce qui pourrait conduire à une concurrence fiscale déloyale de la part de part et d'autre, doit être combattu, c'est l'esprit de ce texte et donc unanimement le groupe RDSE le vôtre.

Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord rappeler que cette convention fiscale année très ancienne puisqu'elle date de 1971 c'est-à-dire que les relations fiscales avec le Portugal sont anciennes et bien avant l'entrée en 1986 du Portugal dans la communauté européenne, le groupe de l'Union centriste, Monsieur le ministre se félicite que la France ait signé la convention multilatérale sous l'égide de loger tout simplement parce que nous estimons qu'effectivement la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale doivent constituer des priorités de l'action publique et il est important que l'on puisse agir en ce sens, alors ici, nous avons, nous pour quelle raison l'examinons nous bah tout simplement parce qu'effectivement cela était dit tout à l'heure, notamment par le rapporteur par vous aussi, monsieur le ministre, et se sont trouvées des difficultés pour un certain nombre de nos concitoyens, fonctionnaire au Portugal qui ont dû se trouver imposée au Portugal par l'application d'une partie des dispositions de la convention initiale qui pendant des années, n'avaient pas été appliquées alors pourquoi cela est survenu, notamment parce que le Portugal comme bon nombres de pays a dû subir les effets de la crise de de de 2008 et a dû pour cela prendre un certain nombre de mesures, parmi les mesures qui ont été prises il y a bien sûr celle de la rigueur fiscale mais ils se sont attachés à appliquer les conventions et dispositions qui avait été décidé, il faut que nous puissions nous en inspirer aussi parce que, grâce à ces mesures de rigueur fiscale, le Portugal a pu arriver en 2016, un déficit public de 2 pourcent je rappelle que l'audit de la Cour des comptes nous signons nous a signalé que pour la France si on ne fait rien, on n'est sur une tendance de 3,2 pourcent du du du des PIB en déficit public cette année, c'est dire le chemin qu'il reste à parcourir, mais je vous sais déterminer, monsieur le ministre, pour que nous arrivions, bien sûr en en-dessous des des le Portugal a aussi pris des mesures pour favoriser la croissance et là où, en début d'année en elle prévoyait une croissance de 1,4 pourcent hé hé bien, selon les chiffres observé au 1er trimestre on va arriver à 1,8 pourcent c'est c'est à dire là aussi l'effort que le Portugal fait quand nous la France nous estimons que nous devrions arriver cette année à une une croissance de l'ordre de 1,6 pourcent nous nous avons donc là aussi des efforts à faire, et puis cela a été évoqué par le rapporteur tout-à-l'heure également des dispositions fiscales tendant à renforcer l'attractivité du Portugal ont été prises, il faut aussi que nous puissions nous en inspirer donc pas pour faire échapper à l'impôt, bien sûr, ce qui viendrait s'installer en France mais peut-être prendre d'autres dispositions qui permettront de renforcer l'attractivité de notre pays, nous y en travaillé au Sénat pour ce qui concerne l'attractivité de la place financière, il n'apporte que des mesures puissent être prises en ce sens, alors cet avenant, monsieur le ministre, a été signé en août dernier, en août 2016, je voudrais féliciter l'ensemble des équipes des fonctionnaires que de la diplomatie qui a participé à à à à cette discussion et qui a permis d'aboutir effectivement un accord sur quelque chose qui n'était pas facile et et je ne pense pas que que ce résultat soit le résultat de, d'un enthousiasme que les Portugais auraient démontré à l'égard de la France à l'issue de la victoire qu'ils avaient obtenu dans l'Euro 2016, au Stade de France contre notre pays à 0, donc félicitations oppose équipe merci et le groupe de l'Union centriste votera, bien entendu, il se peut conventions fiscales.

La présidente, monsieur le ministre, mon groupe votera bien sûr ce cet avenant, et je crois que c'est une bonne chose que nous discutions les les conventions fiscales, il nous est arrivé même de nous opposer à certaines et l'accord qui est pour nous, et bienvenue en tant que sénateur des Français à l'étranger, j'ai été plusieurs fois au Portugal, j'ai rencontré les communautés concernées, il y avait une certaine émotion, bon qui question fiscale suscite de l'émotion, mais en fait, leur émotion était en partie de bonne foi, parce que de, de, de 71 73 prévoyait déjà un partage de la fiscalité directe entre la France et le Portugal, mais le Portugal ne s'en était pas préoccupé, autrement dit les Français ou les Franco-Portugais concernés n'étaient fiscalisés que sur la France et ceci a duré une une dizaine d'années, et tout le monde heureuse au bord du Tage quand tout d'un coup pour les raisons qui ont été indiquées le le Portugal s'est réveillée si j'ose dire, et avec une base juridique solide, a dit : mais comment ça se fait, il n'y a pas partage de la fiscalité, donc nous faisons des enquêtes des redressements et donc il y a eu de la tracasseries fiscales, fois encore une fois l'accord est bienvenue, je ne reprends pas ce qu'a excellemment expliqué le rapporteur sur l'imposition exclusif des Français. Franco-portugais en matière de rémunérations et pensions publiques de source française, c'est une dérogation au modèle de l'OCDE et on doit féliciter les négociateurs français de l'avoir obtenu, et je pense que tout le monde en se racontant puisque la fiscalité, un peu plus douce en France, au Portugal, c'est moins vrai, ce que je dis là est moins vrai sur les pensions, puisque, en matière de pensions le le Portugal n'a pas accepté que les retraités binationaux soit très fiscalement de la même façon que les fonctionnaires, ils seront donc fiscalisé au Portugal pour ceux qui sont de double nationalité je rejoins le rapporteur pour demander que l'application réelle rétroactive des nouvelles dispositions soient faits avec clémence par le Portugal, ça n'est pas évidemment une chose facile, ça veut dire qu'il faudrait que le gouvernement français discute avec la partie portugaise et demande et demande au fond une faveur, mais enfin, on comprend qu'elle, elle serait important et enfin sur l'ensemble des points que vous avez soulevé monsieur le rapporteur concernant. Des fiscalité douce que certains pays mettent en place, que ce soit des pays en dehors de l'Union. C'est C'est vrai, au Maroc, c'est vrai à l'île Maurice. On peut en discuter, encore que, mais à l'intérieur de l'Union, c'est quelque chose qui est choquant, c'est quelque chose qui est choquant, parce que c'est du dumping fiscal. à l'intérieur même de l'Union et c'est pas la voie que nous recherchons, nous recherchons au contraire une harmonisation et une cohérence dans la fiscalité, je pense, donc là, bon, on comprend que le Portugal cherche à développer son pays mais ce genre de ce genre de pratique n'est pas à encourager, bien au contraire, voilà et comme je l'dis donc, mon groupe votera cet avenant.

avec son son rapport évoqué évidemment la portée rétroactive jusqu'à 2013, mais pas de façon identique pour les binationaux j'entends votre demande de clémence,

jeudi 12 ans plus ce que j'ai dit avec monsieur le ministre en charge du Portugal des des relations très sympathique puisqu'il est venu me voir à peine la nomination en fait et on a parlé de cette convention,

et effectivement dans les bonnes relations que nous avons pour nos, nos concitoyens français et pour les concitoyens portugais je, je pense que le traité multilatéral et est très innovant en matière, en matière fiscale, il va avoir pour effet de modifier pour nos traiter une question très sensible que vous évoquez d'ailleurs la légitimité transparence ce que je, je peux m'engager puisque c'était de questions de monsieur rapportera à ce que

du droit et puis d'informer le Parlement est particulièrement les, les, les parlementaires qui s'intéressent à ces codification je propose M6, je sais qu'ici j'ai un gros travail de pouvoir travailler dans dans ce texte, ces textes consolider, texte de base et des avenants.

en général très bonne et le gouvernement s'engage publie le rapport avant la fin de l'année si vous en êtes d'accord c'est ça vous agrée, monsieur le rapporteur, et donc ainsi répondre à votre interpellation, vous dire que, aujourd'hui, un ancien résident de, de, de, de France, devenant résident ce territoire portugais, vous l'avez évoqué et personne retraite privés de source française pourra satisfaire des conditions pour être exonéré sur la pension au Portugal, selon la Cour, dite convention voilà donc il est vrai qu'une personne morale par ailleurs est considéré comme un résident fiscal au sens conventionnel, si et seulement si elle est assujettie effectivement soumises à l'impôt sur les sur les sociétés, à défaut, si c'est pas le cas, elle ne pourra pas bénéficier de l'application de la convention fiscale concernés, je pense que ça répond à votre interrogation, mais si cela n'était pas assez clair : je me permettrai de répondre pratiquement à votre à votre question, mais je crois que ça fait écho, moi je voudrais simplement répondre aux sénateurs, mais je pense qu'il est parti, malheureusement, du groupe communiste sur l'optimisation fiscale, moi je pense qu'il a a il tout à fait raison : la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale cette quelque chose que le gouvernement entend combattre, d'ailleurs nous avons particulièrement bien travailler avec nos, nos partenaires et la discussion est riche au niveau de l'OCDE sur ces questions, et la France évidemment sera totalement aux côtés de tous ceux qui souhaitent lutter contre cette mauvaise façon de de voir la fiscalité notamment des recettes en moins pour nous, pour nos finances publiques et de manière générale, nous aurons l'occasion d'associer les parlementaires à la lutte contre la fraude fiscale en lien bien sûr avec les les travaux conduits par l'OCDE, je pense que la convention le montrent particulièrement enfin sur la concurrence fiscale, bon, il paraît tout à fait normal que le Portugal dessert venir dans son pays des résidents qui, pour qu'ils puissent payer l'impôt, nous faisons pareil avec le système, notamment des impatriés, question, c'est une question à importante qui mérite d'être souligné qu'une question de souveraineté et je crois que nous sommes désormais dans un rapport qui, à la fois monsieur sénateur, vous l'avez dit, qui permet à chacune et à chacun de pouvoir vivre sans ses travaux tracasseries fiscales, nous verrons si on pouvait obtenir en plus cette clémence fiscale et désormais, nous aurons l'occasion de voir dans la Scion avec le Portugal que selon le du football, monsieur le sénateur et et plus selon des difficultés fiscales, je vous en remercie. Merci monsieur le ministre, je vais mettre on voit ticket l'unique constituant l'ensemble du projet de loi, le vote sur l'article voudra vote sur l'ensemble du projet de loi, il n'y a pas de demandes de paroles, je n'en vois pas je mise au voilà qui Cluny constituant l'ensemble du projet de loi qui est pour.

à 16 heures projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social et j'aurai l'honneur et puis-je me permettre de dire et en même temps, le plaisir de présider cette séance, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous retrouve lundi à 16 heures